La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal est donc adopté sur les réserves d'usage. Madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun sera attentif. Au cours des échanges au respect, à la fois des uns et des autres et et du temps de parole. Et je vais donner la parole au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le président vous avez la parole. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame, la Première ministre. De l'autre côté de l'Atlantique, les déboires de la si comme Valley Bank la signature banque nous renvoie au mauvais souvenir de la crise financière de 2008. C'est effrayant ça rapidement affolé les marchés. Suscita une crainte chez les citoyens américains qui ne voudraient pas voir exporter chez nous à l'Europe, depuis quelques jours, que ce soit à Bruxelles, par la voix du ministre des Finances de la zone euro ou parcelle de Jéhovah une aux États-Unis. Les commentaires se multiplient pour affirmer que l'on doit garder confiance. Certes l'fédérale américaine, le Trésor se sont mobilisés pour éviter le pire. Certes à l'Europe les règles prudentielles se sont durcies au cours de cette dernière décennie, en jouant sur le niveau de solvabilité et de liquidité de la banque, je mange de amener ma première Ministre socialiste. Et le moins de risque systémique. Au sein de l'Union européenne car le reconnaître serait l'encourager. S'il y a le problème des marchés financiers, pas le seul d'ailleurs. La fébrilité Salima des déclarations alarmistes certes si on peut espérer qu'il y a samedi soit éteint. Car ces banques reine américaine interroge quant aux effets de la politique monétaire menée par les banques centrales depuis plusieurs mois la remontée des taux d'intérêt comme principale boussole le point c'était le pas à montrer ses limites pendant ce temps nos concitoyens en particulier les plus modestes. Souffrent de plus en plus d'inflation, nous sommes à la veille de la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne doit-on s'attendre à la Première ministre a une nouvelle hausse des taux, au risque de restreindre encore la liquidité du du système. pensez-vous que les banques françaises soient suffisamment capitalisées et à mesure de continuer à jouer leur rôle de prêteur auprès des entreprises et des particuliers. Tout cela dans une situation économique européenne dégradé. Pour vous répondre. La parole est à madame la Première ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs le les sénateurs, monsieur le président, Jean-Claude Requier. Les raisons de la faillite de la banque californienne SVB sont bien connus. Une exposition au seul secteur de la technologie, une capitalisation insuffisante et un manque de fonds propres. Une supervision défaillante. Cette situation a amené les autorités américaines à prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour stabiliser la situation. Et je vous confirme, comme le ministre des Finances l'a rappelé hier que les banques françaises ne sont exposés à aucun risque à la suite de la faillite de la SVB elles respectent des exigences de fonds propres et de liquidités parmi les plus fortes au monde, elles sont soumises à une supervision européenne, elles ont des activités diversifiées, plus proche de nous, s'agissant du Crédit Suisse, dont les difficultés sont connus de longue date. Je tiens à rappeler que cette banque n'appartient pas à la zone euro. Elle n'est pas soumise donc à la supervision bancaire européenne et le ministre des Finances aura un contact avec son homologue suisse dans les prochaines heures. Ce sujet est du ressort des autorités suisses et doit être réglée par elle, donc vous le voyez, nous sommes très vigilants, mais la situation est très différente de celle que nous avons connu en 2008 depuis des nombreuses règles prudentielles ont été prises pour toutes les banques de la zone euro. Je vous remercie. Sur OK. Merci hein. Hier le Covid aujourd'hui la guerre en Ukraine. Espérons que le mais nous l'aurons pas une crise financière. À l'économie comme ailleurs, la confiance ne se décrète pas, elle se perd en litres mais ne se gagne quand goutte. La La parole est à notre collègue Mélanie Vogel. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci monsieur le président. Merci. Monsieur le Ministre, dans une démocratie parlementaire normale. Aujourd'hui, serait la journée de l'apaisement après des années de négociations avec les partenaires sociaux avec toutes les forces politiques un consensus sur l'avenir du travail et sur notre système de retraite aurait été trouvé et la réforme des retraites, seraient en voie d'être adopté largement et paisiblement. C'est le modèle décisionnel de tous les pays européens que vous aimez tellement prendre en exemple mais pas ici. Ah parce qu'ici c'est la France et qu'en France le gouvernement M. avoir raison tout seul en écoutant personne et en agissant contre tout le monde et qu'importe à son avis que personne ne soit d'accord avec lui personne, Monsieur le Ministre personne sauf une partie des républicains n'est d'accord avec vous, vous êtes tout seul 75% de la société française et contre cette réforme, 93% des actifs. Aucun syndicat, aucun syndicat ne défend votre réforme même la majorité parlementaire n'est pas certaine. Et pendant que les Français sont encore massivement dans la rue. Sept députés qui n'ont jamais voté ni même étudié tout le texte et sept sénateurs et sénatrices à qui le gouvernement a imposé un vote bloqué ont décidé à huis clos de prendre deux ans de repos aux plus précaires. Et vous, à ce moment-là vous hésitez entre une majorité de quelques voix arracher contre un pays transformé en poudrière où le 49.3, c'est-à-dire l'adoption sans vote d'une réforme minoritaire. Ces 2 options. Monsieur le Ministre ces deux options sont une folie. Ce n'est pas parce que des outils sont légaux que leur utilisation est légitime, ce n'est pas parce que des outils sont. Qu'il réponde aux standards démocratiques moderne des démocraties dignes de ce nom. Arrêtez les frais. À ce stade de tension sociale et démocratique. L'urgence, franchement c'est plus la réforme des retraites. L'urgence est de sortir de ce fonctionnement mortifère et d'organiser démocratiquement la transition vers une république vraiment parlementaire.

Au fond, si j'ai bien compris votre question est plutôt qu'une question c'était une interpellation vous considériez pratiquement que nous ne sommes pas dans une des dans une démocratie moderne. Alors nous sommes dans une démocratie moderne. Nous sommes dans une démocratie qui permet l'expression des oppositions qui permet l'expression des divergences et les mobilisations que vous avez évoqué en sont la démonstration les plus enfin les plus flagrantes. Elle permet l'expression des divergences. Elle permet l'expression des oppositions dans la limite du respect de l'ordre public et respecter l'ordre public, c'est à la fois éviter les débordements. Les organisations syndicales le font très bien pour l'organisation des manifestations, mais respecter l'ordre public c'est aussi condamné les coupures sauvages des coupures d'électricité qui vise les permanences et les habitations des élus dans des. Sénateur c'est éviter et c'est condamner aussi les coupures qui mettent en danger les commerces, les établissements scolaires. Les administrations qui mettent en danger. Celles et ceux qui sont hospitalisés chez eux et qui ont besoin d'électricité pour des respirateurs au pour des appareils médicaux et puis respecter l'ordre public c'est d'une certaine manière respecter le fonctionnement de nos institutions. Nous sommes au sénat et j'ai eu le plaisir de passer avec vous ici même 10 jours de débats, 10 jours pendant lesquels le Sénat puis évoquait chacun des Arctic chacune des dispositions, vous nous dites, madame la sénatrice. Il y a eu un vote unique oui comme sur la réforme de 2010, ici même, comme sur la réforme de 2013, à l'Assemblée nationale comme sur la loi pour la sécurisation de l'emploi, c'est une procédure constitutionnelle qui a un objectif et un mérite qui est de contourner l'obstruction parce que si nous nous posons la question il y a eu obstruction l'obstruction au Sénat n'a pas été de la même nature que celle de l'Assemblée nationale. Mais il y a eu obstruction vous avez méthodiquement par le dépôt de presque 9000 amendements et sous-amendements voulus paralyser le Sénat et vous lui retirez au Sénat, sa capacité à délibérer la majorité du Sénat le gouvernement ont su répondre pour permettre au Sénat de se prononcer et samedi soir, le Sénat a adopté la réforme adoptée la réforme avait toutes ces dispositions et je forme le voeu bien évidemment que la une commission mixte paritaire permette de trouver un texte de consensus entre à l'Assemblée nationale et le Sénat.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Laissez-moi vous lire une lettre d'un salarié de l'usine Buitoni à Caudry l'être à son employeur, le groupe Nestlé. Courant mars 2022. J'apprends que toute la production de pizzas et rappelé par Nestlé. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est inquiétant. On me demande de rester chez moi. J'apprends que le fruit de mon travail. Aurait handicapé et tuer des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait. Je suis aussi père. Je suis rempli de honte et je pleure. Le soir. Je vais au resto du coin en famille où tout le monde me connaît. À à mon arrivée, quelqu'un m'interpelle. Voilà ça de chez Buitoni. Je ne réponds pas, nous partons. Les chaînes d'info nous accable. Comment les salariés pour travailler dans des conditions ils sont sales, c'est bien fait pour eux. Je me demande pourquoi Nestlé ne prend pas la parole pour dire que ces employés ne sont pas responsables de ce drame. Début janvier, après une fermeture d'initiative et le tournage compét du site, les activités reprennent mais le commande les comment ne sont pas au rendez-vous. La direction suspend la production et arrête la fermeture du site. Voilà Monsieur le Ministre, en quelques mots la détresse que vivent depuis 12 mois. Les 150 employé d'usine de Caudry. La même semaine on annonce la fermeture de lits, l'usine Téréos à d'Oeuvres. Avec de nouveaux 150 emplois menacés. Cette usine produit sucre une des filières des chances françaises mais à force d'appliquer de façon drastique plus drastique que nos voisins les normes. Nous sommes en train de détruire notre filière betteravière. Alors que le gouvernement parle de réindustrialisation des territoires. Malheureusement je peux d'avance vous annoncer que d'autres fermetures vont suivre. Son énorme coup de massue pour le Cambrésis le code Rézi territoire déjà en grande difficulté. Aussi, Monsieur le Ministre, quels moyens entendez-vous déployés pour sauvegarder ses usines. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Wattebled d'abord merci d'avoir. Rappelé avec émotion réelle les mots que moi aussi j'ai entendu lundi quand nous étions ensemble à Caudry pour rencontrer les salariés de cette usine qui vous l'avez dit ont pris comme un coup de massue. L'annonce de la suspension d'activité de la chaîne de production et surtout ont pris comme une énorme injustice les accusations qui finalement leur ont été portées depuis un an, certains ont été traités. Vous l'avez dit d'assassin alors qu'évidemment ils ne sont en aucun cas responsable du drame sanitaire qui a affecté l'usine de production Buitoni, il y a maintenant un an. Ils n'en sont pas responsables, et donc il est hors de question qu'ils soient les victimes collatérales de ce drame sanitaire. J'ai rencontré la direction mes équipes travaillent avec la direction du groupe Nestlé pour trouver d'autres solutions. Je souhaite qu'on produit sur l'usine de Caudry des pizzas ou autre chose, mais je souhaite qu'on produise et je ferai tout pour. Vous l'avez dit, cette. Cette nouvelle extrêmement difficile. S'est accompagné d'une autre nouvelle, elle aussi. Vraiment triste à côté écho d'Oeuvres de la part de terreau, ce qui a décidé de fermer une de ses usines, vous le savez, vous l'avez dit d'ailleurs ça arrive et ça peut arriver encore à l'avenir des, des fermetures d'usines ça arrive mais pas quand une entreprise gagne de l'argent à la quand là qu'elle en perdait. Il y a quelques années, pas quand une entreprise se désendettent alors qu'elle étaient endetté. Il y a quelques années, pas quand une entreprise bénéficie d'un prix du sucre au plus haut et d'un marché en pleine expansion. J'ai demandé des explications à la direction. Nous avons une rencontre demain. Vous y êtes conviés avec le préfet et la direction et les élus parce que je souhaite qu'on ait des explications très précises sur les raisons pour laquelle une entreprise qui marche, une entreprise qui va mieux fermer une usine, avec un impact très important dans la région. Par ailleurs, je l'ai dit lundi avec vous dans le territoire, je le redis aujourd'hui, nous avons déployé d'ores et déjà annoncé le déploiement de 3 millions d'euros dans le cadre du programme rebond industriel. Qui va permettre aux entreprises industrielles du territoire qui souhaitent investir, et il y en a de pouvoir les accompagner dans la réindustrialisation du territoire, le Nord va mieux monsieur, le monsieur le sénateur, il y a des gigafactories à une heure ou 2h de Caudry qui monte et qui vont créer des milliers d'emplois conclure. Nous ne devons pas pour autant abandonner les territoires délaissés dans le vote vaudou seront à vos côtés, merci. Merci. La parole est. Notre collègue Jean-François Husson, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Ministre de l'économie. Depuis plusieurs années, nous ne cessons d'appeler votre attention sur l'absence de maîtrise de la dépense publique. Un constat qui est partagé par la Cour des comptes. Qui vient de vous adresser une sévère mise en garde pour ne pas dire un carton rouge. Elle dénonce parce que. Compte évidemment. Défalquer des des aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire à l'inflation, la dépense publique continue de dériver. Pouvez-vous nous confirmer que la France détient bien le niveau le plus élevé des dépenses publiques en Europe à hauteur de 58% de notre PIB. Et Monsieur le Ministre, comment avez-vous pu laisser ainsi dérivé nos comptes publics. Pour vous répondre. La parole est au ministre de l'économie. Des finances et de la souveraineté industrielle et numérique monsieur Lemaire. Je connais votre attachement monsieur le sénateur Husson pour rétablissement des finances publiques dont j'espère que vous me suivrez dans la méthode que nous avons proposé, qui nous a permis en 2018 de revenir sous les 3% de déficit public de rétablir les comptes publics et de sortir la France la procédure pour déficit excessif. Cette méthode, c'est d'abord un objectif, ramener les dépenses publiques de 57 à 50 pour 4% des dépenses plus ce qui suppose que tout le monde fasse un effort et qu'on s'abstienne de déposer des propositions qui peuvent augmenter la dépense publique mais qu'on fasse des propositions pour réduire la dépense publique. 3% de déficit repassé sous ses 3% dès 2027 et réduire la dette publique à partir de 2026, voilà les chiffres que nous vous proposons. Nous proposons aussi une méthode pour atteindre ses objectifs. Une revue des dépenses publiques comme cela n'a jamais été engagé dans notre pays consistant à regarder toutes les dépenses publiques de toutes les administrations, y compris en accord avec elle, celle des collectivités locales, celle des associations, celle de l'État parce que la dépense publique c'est 50% de dépenses sociales 30% de dépenses de l'État 20% de dépenses des collectivités locales et qu'il faut donc que chacun puisse participer à cet engagement collectif sur la base un diagnostic qui doit être partagée. Nous ferons ensuite à un séminaire sous l'autorité d'après Ministre pour examiner les dépenses de l'État et nous assurer que chaque ministère contribue bien à la réduction à dépense publique. Je proposerai à toutes les collectivités locales de participer également à cet échange et de s'engager dans dans cette direction-là, dans le respect de la liberté d'administration, des collectivités locales et nous ferons la même chose pour les associations et nous aurons des assises des finances publiques avant l'été, qui nous permettront d'établir le calendrier et le montant de réduction de la dépense s'agissant du calendrier. Je le redis, notre objectif, il est très simple dès le projet de loi le finance 2024, nous aurons des réductions significatives de nos dépenses publiques pour tenir les objectifs que je vous propose de soutenir. Monsieur le Ministre, en septembre dernier, vous aviez annoncé. Qu'elles allaient être les dépenses et puis vous aviez confié le travail à votre majorité pour trouver des économies. Vous avez rendu une copie blanche, c'est-à-dire 0. Comment voulez-vous aujourd'hui entraîné aussi doctement que vous le présenter à l'instant. Votre finalement votre méthode et votre stratégie. Jamais la France depuis la Seconde Guerre mondiale n'a connu un tel niveau d'endettement. Est-ce vrai ou faux. C'est juste une réalité nous allons emprunter 270 milliards d'euros. C'est du jamais vu cette année en 2023 avec des taux d'intérêt qui remonte donc on se retrouve en grande difficulté. La France se retrouve en difficulté au moment où nos partenaires européens ont eux conduit un certain nombre d'efforts. Nous sommes en queue de peloton sur un certain nombre de grands indicateurs d'aide publique record prélèvements obligatoires record déficit public qui nous mettent sur le podium européen envolée du déficit commercial. Ça ne peut pas durer. c'est l'affaire des Français, Monsieur le Ministre, je l'ai dit, vous avez pris finalement un carton rouge et la France. Par contre, on ne peut pas être hors jeu, elle ne peut pas rester hors jeu. Alors Monsieur le Ministre, faut conclure à quand des économies. La parole est à. Notre collègue Dominique Vérien pour le groupe de l'Union centriste. Madame la ministre. La terre est-elle plate. Cette question de paraît absurde et pourtant certaines voix estiment qu'après tout toutes les affirmations aussi complotistes et farfelue soit-elle, mérite d'être débattue. Pire encore, comme je l'ai entendu sur France Inter, hier matin, elles devraient être considérés comme des thèses minoritaires comme les autres qui seraient donc des thèses majoritaire, elles auraient ainsi leur place dans le débat public aux côtés de fait scientifiquement validée. Un mélange des genres particulièrement dangereux aux conséquences parfois désastreuses, en particulier dans le domaine de la santé ou certains vous explique que le cancer se soigne par le jeune ou que les vaccins sont un outil de contrôle mental des populations. Des charlatans profitent de certains pour leur vendre des pseudo-thérapies inefficace et dangereuse quand elle conduise à un refus de soins conventionnels des stratégies pernicieuse qui sous le prétexte du bien-être. Peut à peu à peu leurs victimes sous emprise et les entraîne dans un engrenage sectaire qui peut devenir mortelle. L'un d'entre eux a été récemment mis en examen mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt. Et que dire des mutuelles qui remboursent des médecines dites alternatives sans contrôle sérieux Madame la Ministre. L'État est-il suffisamment armé pour lutter. Notre position vis-à-vis de ces dérives sectaires quasiment unique au monde, peut-elle se conjuguer efficacement avec la législation européenne. Pour vous répondre, la parole. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Madame, Sonia Backès si Madame la Ministre, vous avez la parole. D'abord je vous remercie d'avoir participé à ces assises qui était extrêmement riche et à un moment important et attendu par tout. Toutes ces personnes qui défendent les victimes et ces dizaines de milliers de personnes qui sont touchées chaque année par ces ces dérives sectaires. Effectivement ces assises ont fait l'objet d'un certain ont donné un certain nombre de propositions et la première d'entre elles. C'est la question de la prévention, comment nos compatriotes peuvent-ils croire de la même manière le fait scientifique que un certain nombre de croyances pour répondre à ça, nous avons eu des engagements forts de la secrétaire d'État. Sarah El Haïry, qui, qui, sur le travail qu'on a à faire en matière d'éducation à l'information de nos plus jeunes pour lesquels, finalement, on n'a pas forcément. Évoluer du du passage de l'information traditionnelle aux aux réseaux sociaux. Un gros travail qui va être menée avec les plateformes pour éviter que celle-ci. Contribue. À soutenir ces ces dérives-là et puis un gros travail de communication et puis après il y a un travail particulier en matière de santé a effectuer puisque on sait très bien que l'explosion de ces dérives se passe surtout en matière de santé et il y a une une annonce forte qui a été faire pas fait pardon par le ministère de la, de la santé par la voix d'Agnès Firmin Le Bodo, avec l'encadrement absolument indispensable des pratiques non conventionnelles de soins puisqu'en fait, nos compatriotes ont accès à tout un tas de praticiens de naturopathe qui pour lesquels les les pratiques ne sont absolument pas vérifiées. Et puis il y a tout un travail pardon d'accompagnement des victimes qui attendent une indemnisation et puis il y a un travail de. Sur les hauteurs puisque les auteurs doivent être plus sévèrement punis vous l'avez dit il y a des mises en examen il y a des condamnations mais on a besoin de renforcer notre arsenal pénal et je compte sur vous. Les parlementaires et ici au Sénat, en particulier pour soutenir ce renforcement de notre arsenal législatif pour condamner ces ces gourous et ces charlatans. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre, de votre réponse, effectivement l'arsenal pénal et peut être à renforcé en France. Mais je crois qu'il faut réellement travailler sur la suggestion sur l'emprise et savoir convaincre probablement aussi la CEDH que une personne sous emprise n'est pas une personne libre. Que. Si on a effectivement toute liberté parce que de choisir une religion, c'est un droit fondamental. Il faut savoir que subir une suggestion. Par contre, peut être un vrai danger mortel. Merci. La parole est maintenant madame la présidente. Ceci pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, vous avez la parole madame la présidente. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre hier vous affirmiez devant les députés que chacun devait assumer ses choix. Je vous demande donc aujourd'hui d'assumer les vôtres celui du coup de force antidémocratique, celui de la régression sociale. Depuis 2 mois. Le peuple vous dit non. Les grèves et manifestations se multiplient sur tout le territoire et demeure ce qu'elles ont toujours été des outils du progrès social. Hier vous avez répondu avec nervosité à mon ami André Chassaigne en lui reprochant d'opposer la légitimité de la rue à celle du Parlement. Mais vous qui aimez vous rappelez rappelez votre passé de gauche. Dois-je vous rappeler que c'est la grève et la rue qui ont bâti des conquêtes sociales, sans remonter jusqu'à 1789 contestez-vous les grèves de 1906 pour la journée de travail à 8h contestez-vous la légitimité des grèves de 1936 et la victoire des congés payés contestez-vous les formidables progrès suite au mouvement de 68 à sa grève massive à la mobilisation de la jeunesse. plus proche de nous, les victoires de 95 face à la réforme des retraites de monsieur Juppé de 2006. Faut pour effacer le CPE n'ont-elles pas confirmé la force du mouvement social et sa légitimité. Oui madame, la Première ministre. Il existe une légalité résultant d'une élection, mais il existe une légitimité sociale que vous ne pouvez pas nier et qui aujourd'hui s'impose à vous. Oui, le recul de l'âge du départ à la retraite et refusé par d'autres peuples. Vous avez fait un choix de société, un choix de droite un choix de classe. Le débat a eu au moins le mérite de clarifier l'échiquier politique, l'union des droites de renaissance à LR minoritaire électoralement ensemble vous avez pris les rênes, par un acte d'autoritarisme dangereux pour la démocratie que devrait confirmer la CMP réunie depuis ce matin madame, la Première ministre. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne lâcherons rien y compris avec les moyens constitutionnels qui sont à notre disposition. Pour vous répondre. La parole est à madame la. La Première ministre Madame Élisabeth Borne. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la présidente, Éliane Assassi. Il y a quelque chose de grave à opposer systématiquement la légitimité de la rue à celle du Parlement. Il y a quelque chose de dangereux a tenté par tous moyens d'empêcher le débat. De le bloquer. La gauche sénatoriale a revendiqué un seul objectif, empêcher un vote sur le texte. Vous n'avez pas réussi de longs débats ont eu lieu. Tous les articles ont été examinés et le projet de loi a été adoptée à une large majorité. Madame la présidente associe évidemment j'aurais préféré plus de débats de fond et moins de procédure plus de débat d'idées et moins de posture. Vous en avez décidé autrement. Je le regrette mais c'est ainsi et c'est le fait unique de ce qui devient la NUPES sénatoriale.

Je veux à cet égard salué l'attitude responsable de la majorité sénatoriale pour la bonne tenue des discussions dans l'émission. Vous avez pu vous pencher sur tous les articles et enrichir le texte de nombreuses propositions notamment pour améliorer les pensions des femmes ou en faveur de l'emploi des seniors. Vous avez également pu faire votre de nombreux amendements déposés lors de l'examen à l'Assemblée. Madame la présidente Assassi quand j'entends, j'entends certains parlementaires de la NUPES qualifié le processus démocratique en cours de prise d'otages des Français. J'y vois une entreprise de disqualification de nos institutions particulièrement insupportable venant d'élus de la nation. Pour ma Pour ma part j'ai le plus grand respect pour le travail parlementaire qui se poursuit en ce moment même en commission mixte paritaire. Et je suis convaincu que le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent s'accorder pour un projet qui garantira l'avenir de nos retraites par répartition qui réduira l'écart de pension entre les femmes et les hommes qui augmentera les petites retraites qui fermera les principaux régimes spéciaux qui améliorera l'emploi des seniors qui protégera ceux qui sont usés par le travail qui permettra à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt. Cette réforme est nécessaire, elle a été enrichie notamment grâce aux travaux de votre assemblée et avec mon gouvernement. Nous sommes pleinement mobilisés pour que dans les prochains jours une majorité votent la réforme des retraites. La parole est à madame. Samantha Cazebonne pour le. Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre des Sports. L'institut de la jeunesse et de l'éducation populaire a rendu public jeudi 3 mars un baromètre national des pratiques sportives, pour l'année 2022 dont les résultats sont très encourageants, 60% des Français de 15 ans et plus ont pratiqué une activité physique et sportive en moyenne une fois par semaine au cours des 12 derniers des 12 derniers mois, soit 6 points de plus qu'en 2018. Malheureusement, ces résultats ont pu être occultée par les profonde crise de gouvernance qu'ont traversé certaines institutions du sport français depuis quelques années, notamment les Fédération française de rugby et de football. Le sport est vecteur d'unité et d'émancipation, il rend possible une société rassemblée autour de valeurs essentielles telles que l'équité, l'esprit d'équipe l'inclusion le respect la persévérance et rien ne doit entacher le projet politique et sociétal qu'il porte en lui. Alors que la France se prépare à accueillir des événements sportifs mondiaux majeurs. La Coupe du monde de rugby qu'à la fin de l'année et les Jeux olympiques et paralympiques. À l'été 2024. Il apparaît donc nécessaire de promouvoir des valeurs sportives irréprochable ma question Madame la Ministre porte sur la réforme de la gouvernance des fédérations sportives. Un comité national pour renforcer l'éthique dans le sport vient d'être créée et ses membres Pourriez-vous préciser quel va être le fonctionnement de ce comité, ainsi que ses missions précises et ses objectifs. Merci. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice, Samantha Cazebonne en effet les derniers mois ont été marqués par une série de crises. Dans le sport français qui ont mis en exergue la nécessité d'améliorer la gouvernance de ce sport, et notamment des fédérations sportives Il est clair absolument clair que ces errements constatés ne peuvent pas se reproduire. S'agissant d'organisation qui sont délégataire d'une mission de service public et qui ont la responsabilité d'une partie de notre jeunesse mais il est clair aussi et merci d'avoir rappelé que ça ne doit pas éluder les progrès dans la pratique sportive l'engagement remarquable des bénévoles des éducateurs et aussi que beaucoup de fédérations vont bien avance bien ainsi que les progrès la démocratie sportifs qui ont été notamment impulsé par la loi du 2 mars 2022 qui a instauré la parité au niveau des instances dirigeantes du sport français et aussi permis le vote des clubs pour les assemblées générales électives maintenant cette amélioration de la gouvernance, il faut la prolonger la poursuivent l'amplifier. C'est le sens de ce comité national pour renforcer l'éthique et la démocratie dans le sport que j'ai mis en place qui va être co-présidée par Marie-George Buffet et par Stéphane Diagana. Il va être composé de 10 autres personnalités qualifiées incontestable venant d'horizons divers. Je pense à Jean François Lamour. Je pense à Arsène Wenger. Je pense à notre arbitre pionnière Stéphanie Frappart, je pense aussi à une grande dame comme Isabelle Autissier ce comité aura la responsabilité de me faire des propositions pour l'Automne prochain en faisant un très grand nombre d'auditions et il aura la responsabilité à l'Automne de me livrer un certain nombre de conclusions autour de 3 axes une gouvernance du sport qui soit plus éthique, plus démocratique, avec plus de débats, plus de pluralisme et aussi plus protectrice des pratiquants et des pratiquants, notamment sur la thématique des violences à caractère sexiste et sexuel, je vous remercie. Merci, madame la Ministre Madame Cazebonne. La parole est à d'autres collègues Rémi Cardon. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame, la Madame, la Première ministre d'monsieur Dussopt disait hier devant les députés, je le cite, pour atteindre le port, il faut un cap. Ce cap, progrès, justice équilibre pour nos retraites, nous ne cherchons toujours et ce n'est pas le simulacre de démocratie que vous avez offert au Parlement qui nous a permis de nous en a rapproché. Premièrement les retraités ne verront jamais leur 1200 euros une homme de pensions de retraite longtemps promise. Voilà votre vision vision du progrès. Deuxièmement les femmes continueront de toucher des pensions de retraite inférieure à celle des hommes, en moyenne 39% voilà, votre vision de la justice. Troisièmement, vous faites reposer tous les efforts sur une seule génération sans jamais solliciter le patronat voilà votre vision de l'équilibre. Madame, la Première ministre. Une chose est sûre. Nous ne partageons pas le même cap. Et nous sommes des millions à refuser d'embarquer avec la droite sénatoriale sur ce radeau de la méduse. Vous faites l'unanimité et l'unité contre vous. L'unanimité des syndicats des travailleurs des millions de personnes qui descendent dans les rues chaque semaine qui vote la réduction des des grèves, la reconduction et qu'ne lâcheront rien. J'aimerais vous demander, madame, la Première Myst finalement pour qui et avec qui gouverner vous. Ce que vous proposez, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs c'est l'alternative mortifère, à savoir la préparation du terrain à la prise de pouvoir du Rassemblement national. Bref, il me reste à vous demander, madame, la Première ministre êtes-vous des inconscients ou des irresponsables. Ministre du Travail, du plein emploi d'insertion. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur cardan. Vous dites que ne partageait pas être sentiment que vous ne partagez pas notre réforme. Nous nous sommes convaincus que cette réforme a une majorité. Cette réforme a une majorité parce que elle peut être votée par tous ceux et toutes celles qui souhaitent sauver et préserver le système par répartition. Cette réforme a aussi une majorité parce qu'elle peut être voté par tout ceux qui sont prêts à aménager et faire en sorte de mieux protéger à la fois ce qu'ont les carrières les plus longues mais ce aussi ceux qui ont les métiers les plus exposés à l'usure professionnelle et la pénibilité. Cette réforme, elle a une majorité parce que tu ceux qui veulent a voté sont ceux qui veulent faire en sorte que l'emploi des seniors s'améliorer dans notre pays et que nous ayons un taux d'activité qui puisse augmenter et cette réforme, elle sera aussi voté par ceux qui sont attachés à la revalorisation des petites retraites vous en fait un cheval de bataille. Monsieur le sénateur. C'est la démonstration que la gauche aujourd'hui est déconnecté des classes populaires avec cette réforme, ce sont 1.800.000 retraités actuels qui vont bénéficier d'une revalorisation pouvant aller de 25 à 100 euros. Ce sont 900.000 parmi eux qui vont bénéficier d'une revalorisation de 70 Vous nous dites que nous serions inconscient et irresponsable l'irresponsabilité dans votre camp. Elle est dans votre camp quand vous ne faites rien alors que le système est en train de s'écrouler. Elle est en son quand quand elle est dans votre camp quand vous faites rien alors que ce que notre réforme permet de sauver le système par répartition. Monsieur le sénateur pendant le débat dont vous n'avez visiblement pas retenu grand-chose. Vous avez eu des mots assez assez outrancier, comme nous on a vu à l'instant à l'égard de la Premier Ministre c'est la démonstration, monsieur le sénateur. Que la mélenchonisation des esprits que j'ai évoquées. Elle vous a gagné comme elle gagne l'ensemble de la gauche française. Monsieur, monsieur Dussopt. Votre majorité c'est tout simplement le 49 3. Monsieur si vous voulez en tout cas sachez gouverner sans le peuple et contre lui et ses représentants, c'est dangereux pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe socialiste, nous allons déposer une demande de riz pour sauver la démocratie pour sauver la République de vos bâillon. La parole est maintenant à notre collègue Marc Philippe Daubresse pour le groupe Les Républicains. C'est monsieur le président, monsieur le ministre. De la transition écologique. La récente publication des chiffres de la construction neuve pour 2022 confirme ce que nous n'avons cessé de dire depuis plusieurs mois à plusieurs ici au gouvernement. La situation n'est pas dramatique elle est catastrophique. Rarement on a connu des chiffres aussi dramatiques. Moins 25% pour les promoteurs privés, moins 30% pour les constructions individuelles 350.000 unités prévues en 2023. Pour mémoire, après le plan de relance de Jean-Louis Borloo, on était à 486.040% de moins annoncé pour l'année qui vient et ça va continuer. Des faillites en cascade. Sont annoncés dans la promotion pour le logement social, la réforme funeste des APL de la loi élan à assécher les finances des offices d'HLM et on est pour la 3ème année consécutive en dessous des 100.000 logements sociaux. Sans parler des mesures que vous avez prise sur un certain nombre de sujets, par exemple le zéro artificialisation nette. Heureusement que le Sénat est en train de les corriger. Donc Monsieur le Ministre. Ma question est simple. Est-ce que vous avez prévu, enfin un plan de relance pour relancer la construction neuve dans notre pays, comme nous l'avons fait avec succès sous Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, est-ce que vous avez prévu des mesures fiscales de relance exceptionnelle comme nous avons réussi à le faire sous le gouvernement de François Fillon. On vous réponde. La parole est au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, Marc-Philippe Daubresse. D'abord quelques chiffres très récent et qui seront l'occasion de d'objectiver les choses. On a une augmentation des autorisations. En 2022, qui remonte à un niveau que nous n'avions pas connue depuis plus de 6 ans à plus de 480.000 en hausse de 3% mais dans le même temps on a une baisse des mises en chantier de 3% à 376.000 avec les indications que vous donnez entre les deux. On a des phénomènes structurels. Je vais revenir mais on a aussi un phénomène conjoncturel. Qui est la très forte augmentation des refus de prêts dans un double contexte où globalement les taux d'intérêt sont passés de 1 5 à 3, 20 sur 20 ans et où, dans le même temps le coût moyen de la construction a augmenté avec un effet d'inflation généralisée en 2022 particulièrement vrai dans le Champ du logement 1er sujet à côté de ça, par rapport à cette question des prêts et de la baisse de la demande puisque nous avons eu 39% de baisse de la demande au dernier trimestre. Et ça c'est pas un sujet gouvernementale. La baisse de la demande et les à des acheteurs qui cessent d'acheter pas à une absence d'offre. La réforme du taux d'usure en faisant en sorte de la mensualisé depuis le 1er février pour fluidifier une partie du marché. Le premier élément de réponse. Les réponses plus structurelles. Elles seront prises dans la continuité du CNR logements qui se termine au mois d'avril, nous discutons en ce moment, avec tous les professionnels, vous en avez cité un certain temps, il y en a d'autres et dans ses autres il y a les élus. L'ambition du président de la République, c'est d'ouvrir le chantier de la décentralisation, du logement, vous connaissez parfaitement ces questions vous les avez connu comme élu local, vous les avez connu comme membre du gouvernement. On a eu l'habitude de réfléchir sur un combien là où la disparité des situations fait que c'est le où est le comment qui mérite d'être questionnée. Et la décentralisation du logement. Elle est au coeur d'une ambition, y compris sur la rénovation énergétique dans un dialogue franc avec les communes avec les intercommunalités et avec les départements changement dézonage. Décentralisation des dispositifs soutien aux maires bâtisseurs. Ce sont ces ensembles sur lesquels nous travaillons. Monsieur Daubresse. Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, j'ai été en son temps ministre du logement, il faut que vous révisez vos chiffres. Les notaires viennent de sortir le dernier chiffre pour le dernier trimestre 2022 par rapport il y a un an, c'est moins 25%, les permis de construire, Monsieur le Ministre, moins 25% annoncés. Je vais prendre un seul chiffre si vous rapportez le nombre de constructions neuves à la population. Nombre de ménages français c'est le plus bas, chiffre que nous allons connaître depuis 1951 ça avait donné l'appel de l'abbé Pierre, Monsieur le Ministre, vous sous-estimer le problème parce que vous êtes confronté à des objectifs stratégiques contradictoires. Il est grand temps que le gouvernement se réveille. La parole est à notre collègue Catherine Conconne pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, madame la Ministre, chers collègues. Haïti pleurant tous les jours c'est mort ces blessés par dizaines Haïti affamé Haïti livré aux mains de gangs a été assistant au viol de ces femmes Haïti voyant ses enfants recrutés par des groupes armés Haïti sans gouvernement sans état s'enfonce inexorablement dans le chaos. Et pourtant, pas un mot de l'État sur la situation de ce pays à qui nous sommes tant redevable ce pays envers lequel nous avons une dette morale, comme le disait si légitimement François Hollande en 2015. 1er en colonie noire à prendre son indépendance en 1804. Haïti, à bien des égards a ouvert des chemins repousser les limites du possible et ce alors même qu'elle a été dès le départ, affublé du fardeau fardeau indigne d'une dette insoutenable pour acheter sa liberté. La résolution adoptée par l'ONU en octobre dernier constitue un pas symbolique mais elle ne peut servir de refuge pour justifier notre inaction collective. Certains pays comme le Canada, on fait le choix d'une politique plus active que fait la France à 1h30 de vol des pays français d'Amérique que fait l'euro il faut désormais aller plus loin que des sanctions face au massacre des Haïtiens devant le roi très des organisations humanitaires qui baissent les bras. Une à une, il faut organiser la coopération dans le bassin caribéen. Il faut oser l'envoi d'une force de maintien de la paix face aux massacres quotidiens de civils haïtiens la tireur la famine dans laquelle vit la population dans un état désormais inexistant. Dois-je rappeler qu'à la suite de l'assassinat du président Moïse en 2017, Haïti n'a plus de gouvernement. Combien de temps encore. Allons nous attendent. Combien de morts encore combien d'horreur qu'on met le viol. Combien de drames avant d'agir. Pour vous répondre. La parole est ministre délégué. En charge. Commerce extérieur. Les Français de l'étranger. Vous avez la parole. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Conconne. D'abord je vous prie de bien vouloir excuser la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes d'accord sur un point, la situation en Haïti qui est très grave à la fois sur le plan humanitaire. Sur le plan sécuritaire et bien sûr sur le plan politique. En revanche, il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est l'inaction de la France aux côtés des États-Unis et du Canada, la France et tu active, c'est l'une des nations les plus actives pour tenter d'aider les Haïtiens. Nous le faisons, notamment dans le cadre du soutien à la police nationale haïtienne et nous allons encore accroître cette coopération et ce soutien, nous le faisons également dans le cadre de l'aide humanitaire, 8, 5 millions d'euros d'aide humanitaire. Dont 5 millions d'aide alimentaire qui va directement aux enfin nous sommes vous l'avez dit actif dans le cadre de la diplomatie au niveau des Nations unies dans le cadre de la résolution 26 53 pour infliger des sanctions criminels qui sont les auteurs de ce que vous dénonciez. À l'instant, notamment ceux des gangs. Enfin, nous sommes à l'écoute de nos partenaires. S'agissant du projet de forces internationale d'appui à à la police nationale haïtienne sur la forme qu'elle pourrait reprendre et nous pouvons envisager d'y apporter un soutien matériel et puis je voudrais enfin terminé par le fait que la sortie de crise implique et vous le savez, un accord inclusif entre les acteurs La mise en place récent du Haut Conseil de transition doit permettre d'avancer vers des élections comme prévu dans le document de consensus national du 21 décembre dernier. C'est en tout cas ce que nous souhaitons, pour le bien d'Haïti. Merci. Madame cocotte. Vous avez quelques secondes. Je ne peux que déplorer. La discrétion, la très grande discrétion des actions que vous venez d'énumérer, mais c'est vrai. Haïti n'a ni pétrole, ni gaz. La parole est à notre collègue Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre de l'Intérieur depuis plus d'une semaine, Paris est devenue une ville submergée par des montagnes de déchets. Eh oui, mes chers collègues je ne vous apprends rien je pense. 7000 tonnes de poubelles non ramassées une reconduction de la grève qui est annoncé jusqu'au 20 mars. Alors cette situation peut entraîner des risques sanitaires conséquent bien sûr aggravé par la recrudescence de la présence des rats appelé les sur mulot à Paris dans les espaces publics de la capitale. Monsieur le Ministre, les parisiens sont en colère. Pourtant, à la mairie de Paris. Personne ne semble s'en émouvoir. Madame Hidalgo a même annoncé son soutien entier et total au mouvement social. Et oui c'est c'est la vérité. Constatant cette inertie. La chef de file de l'opposition à Paris. Madame Rachida Dati vous a saisi hier. Vous avez donc chargé Monsieur le Ministre, le préfet de police de demander à la maire de Paris de réquisitionner les moyens en matériel et en personnel nécessaires au ramassage des poubelles. En réponse, ce matin, le premier adjoint de Madame Hidalgo affirme que c'est le gouvernement qui a créé cette situation. Quel déni. Quelle mauvaise volonté. Alors Monsieur le Ministre, quand l'état va-t-il se substituer à la mairie de Paris pour régler cette situation et surtout dans quel délai. dans quel délai. La parole est. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer monsieur Darmanin. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs Madame la sénatrice. Vous connaissez déjà tout. À la suite de 9 jours de grève et chacun a pu constater qu'ils soient parisien d'occasion, Parisien d'habitude l'amoncellement dans certains arrondissements de Paris, d'un certain nombre de poubelles, que vous avez qualifié vous-de plusieurs milliers de tonnes poser question pour la sécurité évidemment de nos concitoyens. Avant même d'ailleurs où il y a des manifestations, mais pose aussi des questions de salubrité publique que chacun peut constater et pour avoir été comme beaucoup ici gestionnaire d'une collectivité locale, chacun peut voir ce que c'est qu'attendre neuf jours et voir des milliers de tonnes d'ordures et de poubelles effectivement être sur la voie publique. J'ai donc demandé mais au nom de la salubrité publique puisque le ministre de l'Intérieur est en charge de la tutelle. Sur le préfet de police. La préfecture de police et après avoir contacté évidemment madame la maire de Paris après avoir été saisi. Vous avez évoqué madame Dati en effet par plusieurs maires d'arrondissement mais aussi par plusieurs élus. Parisiens, quel que soit leur bord politique après avoir été saisi par eux j'ai donc demandé à madame Hidalgo, d'abord évidemment à l'oral et ensuite ce matin par l'intermédiaire, le préfet de police par écrit de pouvoir faire ce que le droit lui permet de faire notamment que la mairie de Paris a fait pendant 10 de la loi travail puisqu'il y a déjà eu. Effectivement une. Situation similaire de réquisitionner la question qui relève à la fois du. Relèvement là du du des poubelles qui sont relevés pardon de l'espace public comme de l'incinération parce qu'il s'agit bien des 2 sujets à l'oral. J'ai entendu en effet ce matin le premier adjoint, évoquer le fait qu'il ne serait pas favorable à cette situation. J'attends évidemment que madame la maire de Paris répondent par écrit à la demande par écrit du préfet de police et si ce soir cette confirmation été fait que la mairie de Paris, ne prenait pas ses responsabilités, je le dis ce soir, demain matin au plus tard le préfet de police propose procédera aux réquisitions au nom de la salubrité publique et je crois que tous les Parisiens, quelle que soit ce qu'il pense de la réforme des retraites en sont heureux.

ont plongé les Parisiens. Nous sommes aujourd'hui à moins de 500 jours de l'ouverture des Jeux olympiques l'image de notre pays et de sa capitale et durablement dégradée auprès des touristes et des observateurs étrangers qui sont sidérés. Il est donc grand temps d'agir. La parole est au président Laurent Lafon pour le groupe de l'Union centriste. Merci monsieur le président, ma question porte sur le devenir du Stade de France et s'adresse à Madame, la ministre des Sports, des Jeux olympiques et para-olympiques. vous avez annoncé il y a quelques jours que l'État travailler dans 2 directions, soit la session du Stade de France, soit le renouvellement d'un système de concessions déjà en vigueur depuis 25 ans, le gouvernement n'a pas arrêté à ce jour son choix entre ces 2 options qui sont significativement différente. De fait, le Trésor a engagé de manière inédite de procédures parallèles, l'une pouvant aboutir à la vente du Stade de France, l'autre pouvant aboutir au renouvellement de systèmes. De concession, alors que les 2 procédures sont lancées. Les objectifs du gouvernement quant à l'avenir du Stade de France n'apparaissent pas encore clairement aussi Madame la Ministre je souhaite vous poser 4 questions précises pour que vous nous éclairiez sur les intentions du gouvernement. La première, avez-vous eu des engagements de la part des 2 principales fédérations sportives utilisatrices du stade de France de football et le rugby quant à une autorisation a minima du stade et dans quelles conditions financières le souhaite-t-elle le faire la 2ème question porte sur l'athlétisme qui n'apparaît plus dans les consultations lancées par le Trésor. Les deux dernières porte enfin sur la cession concernant la cession, pourriez-vous nous préciser quels sont les critères qui pourrait vous amener à choisir la scission plutôt que la concession Est-ce que l'État français. Serait prêt à vendre le Stade de France à une structure appartements appartenant pardon à un État étranger, Stade de France qui est devenue depuis la Coupe du monde de 98 et avec les Jeux olympiques dans quelques mois un emblème du sport français. français. Pour vous répondre. La parole est à la ministre des sports, des Jeux olympiques et paralympiques Madame Oudéa-Castéra vous avez la parole. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. La font en amont de la fin de la concession à l'été 2025, le gouvernement s'est donné une boussole qui est de faire émerger le meilleur projet de long terme avec méthode et transparence pour le Stade de France avec 2 exigences préserver la vocation sportive du stade et une deuxième qui est de préserver les intérêts économiques et financiers de l'État. Alors vous l'avez dit de procédures ont été lancées en parallèle, vous m'avez posé 4 questions précises, je vais essayer d'y répondre. S'agissant des fédérations. Elles sont libres de candidater. Elles sont libres de s'associer à un candidat, ils sont libres de négocier les conditions d'utilisation du stade, ce qui est important c'est qu'elles puissent échanger avec l'ensemble des candidats dans le respect de l'équité et du droit de la concurrence s'agissant de la piste d'athlétisme les deux avis. Précise bien mentionne bien la capacité d'accueillir des grands événements sportifs internationaux. L'athlétisme est un exemple et là il faudra voir ce que proposeront les candidats s'agissant des meilleures solutions et des meilleures options prises sur ce terrain des grands événements sportifs sur les différents critères, il y en a deux qui sont expressément posée dans les deux avis un critère d'Avantage économique global pour l'État est un critère qui est plus commercial et relatifs notamment à l'amélioration de l'accueil du stade et notamment de l'attractivité de ce stade dans son territoire s'agissant de votre question sur. Un investisseur étranger, s'il devait y en avoir un qui répondent aux conditions protectrice qui dans le cas d'une session serait de toute façon fixé par la loi et Parlement ou si il devait cet investisseur étranger participé à un groupement plus simplement d'opérateur il y a pas de raison de l'en empêcher de l'écarter a priori et par principe mais ce que je veux vraiment dire ses projets ambitieux de long terme à la hauteur de la place de ce stade dans le récit sportif national des attentes des élus et des habitants de ce territoire. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Frédérique Puissat. Pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Ministre, de la Santé. 500 jours 500 jours c'est le nombre de jours qui nous restent avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. La parade nautique où défileront les 10.000 athlètes sur 6 kilomètres, est un lourd défi en matière de sécurité. Le budget que leur l'annoncer maîtrisé à hauteur de 8 milliards d'euros, 100 de plus en plus difficile à tenir. Et la France n'a pas droit à l'erreur. Mais ma question porte sur une autre difficulté, celle qui concerne la situation et la capacité d'accueil des hôpitaux pendant que se dérouleront les Olympiques cet été. Pour ce qui concerne les 15 mises athlètes et ceux qui les accompagnent. Un centre de centrer sera créé en lien avec l'AP-HP. Mais pour ce qui concerne les plus de 10 millions de visiteurs attendus que compte faire le gouvernement. Les hôpitaux de parisien, en temps normal, peine à fonctionner les services d'urgences sont débordés et trop de lits de chirurgie sont aujourd'hui fermées ajoutant de surcroît qu'en plein été, en raison des congés. Les équipes médicales sont réduites. Gouverner c'est prévoir. Alors Monsieur le Ministre, qu'avez-vous prévu pour assurer le fonctionnement des hôpitaux parisiens pour faire face aux soins courants et à l'affût de visiteurs pendant les Jeux olympiques. Merci. On vous pour la parole et communistes de la santé de la prévention. Monsieur François Braun. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Madame la la sénatrice puis ça. Autour de la Première ministre, le gouvernement est totalement mobilisé autour de la ministre des Sports pour faire de la Coupe du monde de rugby également mais des Jeux olympiques. Bien entendu et paralympiques. La grande fête sportive qui doivent être alors dans ce cadre plus global. Bon. Mystère et et concentrée sur 3 points, vous en avez appelé à Jean, Jean préciserez, 2 autres le 1er c'est bien sûr de maintenir l'accès aux soins, l'accès aux soins sur les territoires concernés par les Jeux olympiques, que ce soit à l'Île-de-France. Mais n'oublions pas aussi des Hauts-de-France et et PACA qui vont être directement concernés. Cet accès aux soins, il est pour les Franciliens par exemple bien entendu des des gens qui habitent à côté des des sites olympiques et pour cela nous mobilisons le public le privé la médecine libérale l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir assurer cette réponse qui a évalué, vous parliez des services d'urgence nous évaluant à plus 5% de fréquentation pendant cette période. À titre d'exemple. trois autres publics sont particulièrement concernés, nous sommes attentifs aux touristes qui vont arriver à ce moment-là il y a des questions de prise en charge bien sûr financière mais il y a aussi des questions de traduction, qu'il faut prendre en compte. Les sportifs et leur staff ont des parcours de soins qui vont être identifié pour il ne croise pas. Les les publics de spectateurs et puis enfin les personnes en situation de handicap doivent bénéficier de parcours de soins a parfaitement identifié le 2ème point que nous travaillons, c'est celui des situations sanitaires exceptionnelles, le risque climatique, nous serons été les risques infectieux, les risques NRBC et le risque également de cybersécurité de cyber attaque avec la mise en place de de contre-mesures enfin le 3ème point c'est celui de l'héritage des Jeux olympiques cet héritage, c'est le sport santé. Le président de la République a annoncé que 2024. Le sport serait grande cause nationale dans ce cadre-là le déploiement encore plus important du sport santé, en terme de prévention, parce que c'est un axe fort de la politique de mon ministère va nous permettre d'améliorer l'état de santé globale de nos concitoyens. Voici les 3 axes sur lesquels nous travaillons actuellement de façon extrêmement précis. Je vous remercie. Que le, le ministre, vous l'avez compris ma question est légitime et préventive légitime parce que le personnel de santé s'inquiètent. Préventif, parce que les Français ont trop souffert du fiasco du test du du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. Alors c'est vrai que mesdames et messieurs les Ministres, comme le président de la République. Nous souhaitons des médailles, mais nous souhaitons surtout être sur les plus hautes marches du podium en matière d'organisation, organisation des Jeux olympiques, organisation de la santé pendant les Jeux olympiques, organisation de la santé aussi dans nos territoires et dans nos départements au quotidien pour tous les Français. La parole est à notre collègue Jérôme Durain pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Vous avez écrit le 3 mars aux fonctionnaires de police pour répondre aux inquiétudes qui se sont exprimés derrière le slogan Sauver la PJ de Clémenceau, ce courrier a été rédigé avant même que le rapport du Sénat ne soient rendues publiques. La mission que j'ai eu l'honneur de mener avec ma collègue Nadine. Au nom de la commission des Lois avait pourtant émis 22 recommandations adoptée à l'unanimité pour vous aider à faire cette réforme nécessaire, vous ne les avait pas entendu. Vous les avez d'ailleurs à peine attendu vous vouliez aller vite. Mais vous n'avez pas réussi à rassurer les péquistes qui continuent à exprimer publiquement leur écoeurement. Vous deviez restaurer l'attractivité de la filière PJ vous conforter des envies d'émission. Vous n'avez pas davantage rassuré les avocats, les magistrats qui se joindront aux pigistes demain partout en France pour manifester devant les tribunaux mais surtout vous n'avez répondu à aucun des 4 rapports qui ont été rendus sur le sujet. Les inspections ont évoqué l'insuffisance du cadrage initial de l'expérimentation. Notre collègue Dominati pour la commission des finances, vous appeler à ne pas déshabiller la PJ à l'Assemblée nationale. Les deux rapporteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord monsieur Bernalicis craignant une mise à mal du principe d'indépendance de la police judiciaire ici enfin au Sénat où nous avons proposé un moratoire jusqu'aux Olympiques il vous permettrait d'améliorer votre copie tout en évitant de fragiliser notre appareil sécuritaire avant l'échéance de 2024. Pourquoi monsieur le ministre avait vous rejetez ce conseil éclairé du Sénat.

que c'est une réforme très importante que celle de la réforme de la police nationale. Vous même vous l'avez souligné dans notre rapport avec madame Bénureau comme l'Assemblée nationale a souligné puisque depuis 60 ans, il n'y a pas eu de réforme de la police nationale à ce point structurante et en effet, elle fait naître des interrogations, des questions et bien sûr bousculer des habitudes auxquelles le Vista d'intérieur et singulièrement le ministre que je suis est particulièrement attentif. Je constate d'ailleurs que le Sénat dans sa très grande majorité vous-même d'ailleurs ainsi que le groupe socialiste adopté le principe de cette réforme parce que vous avez voté, vous le savez bien la loi de programmation du ministère de l'Intérieur et je crois de la beaucoup construite ensemble singulièrement sur la question de la réforme de la police nationale. Alors vous dites que nous n'avons pas pris connaissance et et compte de vos propositions. Permettez-moi dire Monsieur le Sénateur, que c'est faux. Il est vrai que j'ai refusé d'attendre la fin des Jeux olympiques pour mettre en place une réforme qui est travaillé depuis le ministre-ce qu'il n'y aura je n'ira pas grand monde. Ici, bien évidemment, et qui par ailleurs travaillé depuis plus de 2 ans et demi par le ministre de l'Intérieur que je suis, qui avait déjà été imaginé par mes prédécesseurs dans le fameux Livre blanc sur l'intégralité des autres dispositions, nous vous suivons, monsieur le sénateur. Les OPJ devront hein systématiquement être OPJ. Bien sûr, c'est le cas, la formation particulière DDPN est prévu. Nous avons travaillé avec le ministre de la justice bien sûr pour que l'évaluation se fasse avec les procureurs de la République pour les DDPN. Nous travaillons d'ailleurs avec une lettre conjointe pour rappeler que l'article 12 du code de procédure pénale soit évidemment que les magistrats puissent saisir et sa mise d'enquête et ce ne sont pas des préfets qui le feront le la le fait que nous ne serions au rendez-vous des DZ PN qui pourront travailler en lien avec les DIPN que j'évoquais dans le courrier, je pense que c'est au rendez-vous également vous suggérer l'état des lieux du stock des procédures c'est à votre proposition numéro 1 avec nous avons confié une mission, suite notamment à vos interpellations les moyens spécialisés pour les directions régionales c'est votre motion no4. C'est effectivement le cas. Les magistrats devront saisir directement les offices centraux. C'est la proposition numéro 3, c'est déjà le cas faut conclure hé oui Monsieur le Président, j'attendais votre rappel pour dire qu'à quel point je ne peux de citer toutes les bonnes propositions que nous suivons de la part du sénateur du. Écoutez, Monsieur le Ministre, toutes ces bonnes propositions ne sont pas tombés dans l'oreille des pigistes et si nous imprimons si nous exprimons une une inquiétude c'est que notre conviction. Et notre crainte c'est que 100 PJ, nous ne gagnerons pas la guerre contre la drogue 100 PJ nous ne lutteront pas efficacement contre la criminalité organisée, notamment économiques et financières. Nous craignons que la dilution de l'expertise de la PJ que le tout voie publique ne soit une impasse, tout comme le rétrécissement départemental et la prend la prise en main de l'administratif sur le judiciaire. Alors oui, Monsieur le Ministre, comme les péquistes vous le disent comme les magistrats vous le disent pour la sécurité des Français. Sauver la PJ. Merci la parole l'état d'autres collègues. Bruno Sido. Pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre de la cohésion des territoires. La Cour des comptes dans son dernier rapport préconise la réduction du nombre de communes et notamment les plus petites d'entre elles. Les gouvernements successifs, par le biais de différentes lois se sont attaquées régulièrement au nombre de communes en France. Toutefois, je tiens à rappeler que le fait communal et le fait départemental précède le fait républicain. La loi de 10, 19.171, dite loi Marcellin a voulu faire fusionner les communes sans grand succès, et d'autres lois similaires ont été votées par la suite. J'ajouterai que comme on n'est pas prophète en son pays ne se mars cela a fait zéro fusion-association dans son département. Par exemple dans partout moi par contre le la Haute-Marne avec cette loi, 200 communes ont souhaité au départ fusionner mais la moitié d'entre elles ont divorcé. L'année suivante. Aujourd'hui, les communes sont attaquées sous l'angle financier afin d'assainir les finances publiques de l'État, en se basant sur les chiffres de 2021 années paradoxale où les investissements des collectivités ont été très réduits à cause de la crise Covid. Monsieur le Ministre, bien que ce que de a dit ce que dit la Cour des comptes soit rarement entendu par les gouvernements. Quelle est votre position sur l'analyse de ce qu'elle préconise. On vous répondre. La parole est au ministre de la. Cohésion des territoires. Monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bruno Sido. À l'évocation. Du fait que. Monsieur Marcellin n'a pas été prophète en son pays. Je veux convoqué la présidente de Roche, le sénateur noir le sénateur Bigot et le sénateur Emmanuel Capus puisque le département du Maine-et-Loire et celui dans lequel il y a eu de plus de fusions de communes. 48% des communes ont fusionné au point qu'il nous reste 186 communes sur les 358 que nous avions mais quand je vous aurais précisé qu'il ne s'agit, quand je vous aurais précisé qu'il ne s'agit que de mariage d'amour et que je vous aurais dit qu'en matière de fusion, je ne crois pas au mariage qui ne sont pas des mariages d'amour. Je vous aurais précisé ce qui est une partie de ma philosophie en pensant qu'il ne faut pas plaquer un modèle national sur ces sujets. Les constats, on les connaît les constats, c'est d'expliquer que nous avions en 1790 44.000 communes que nous n'en avions en que nous en avions encore 38.000 en 1960 et qu'on est rendu que à 34.000 et qu'il n'y a eu que 235 fusions de communes depuis 2014. Pourtant, un certain nombre de PPL je pense à la PPL. Je pense à la PPL Gatel se sont efforcés de regarder comment donner un statut aux communes associées aux communes délégué pour éviter que ce soit tout ou rien. Notre conviction et j'associe Dominique Faure dont vous savez l'attachement aux communes en particulier aux communes rurales en particulier, c'est que rien dans ce domaine ne se fera par la contrainte. L'intercommunalité est une chance, à condition qu'on ait les conférences des maires et les pacte de gouvernance dans certains cas il faut rendre possible effusion montrant ce qu'elles permettent. Mais il ne faut pas qu'elle soit forcée sinon elles aboutissent à la fin à des choses qui sont plus mauvaises qu'elle doit être notre obsession, c'est faire en sorte qu'on ait les mutualisations qui permettent d'améliorer la vie des habitants sur le territoire et le meilleur usage des deniers publics dans certains endroits, ça peut passer par des fusions dans d'autres par des coopérations intercommunales dans d'autres encore par des modes d'associations qui dépendent de ce que les élus veulent, on ne peut pas à la fois expliqué qu'on leur fait confiance et projeté un modèle qui sera le même partout en faisant fi de notre histoire et nos réalités locales. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, les Français sont plus, plus que jamais attachés à leur commune. La crise des gilets jaunes. La crise sanitaire sont passés par là et ont démontré l'importance de ces 500.000 élus qui travaillent, qui administre leur communes, les maires et leurs adjoints et les conseillers municipaux bien souvent tous ces élus sont bénévoles et font même beaucoup les travaux à titre gracieux. Rappelons-nous ce couple mère-préfet le Premier ministre Jean Castex vantait les le mérite des mères comme des piliers de la République. On les applaudissait pour leur implication. Mais aujourd'hui, face au poids des finances publiques. On voudrait les sacrifier. Alors je voudrais vous dire Monsieur le Ministre, que votre réponse ne m'a pas convaincu. Alors je repose ma question, allez vous faire payer aux petites communes le laxisme budgétaire du gouvernement en les supprimant. Merci. La parole est à notre collègue Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur Merci monsieur le président, ma question s'adressait à la ministre de la transition énergétique. En l'espace d'une année la problématique des coûts de l'énergie, vous le savez est devenue cruciale pour bon nombre de nos concitoyens et nos entreprises et même nos collectivités locales. Dans ce contexte le Parlement à légiférer, c'est son rôle et la loi du 16 août 2022, prévoit que le prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique la reine ne peut être inférieure à 49 euros 50 du mégawattheure désormais. Puis, curieusement, le gouvernement a introduit l'obligation de soumettre cette disposition à l'avis de la Commission européenne. Ce que le Conseil d'État dans son délibéré du 3 février dernier a formellement identifié comme inutile puisque ce prix de 49 euros 50 est largement inférieur au prix du marché. Et non seulement le gouvernement semble être sourd à cette objection du Conseil d'État. Mais vous n'avez à ce jour même pas solliciter la Commission européenne. Monsieur ou Madame la Ministre je ne sais pas qui me répondra, pouvez-vous donner les raisons de cette surdité gouvernementale mâtiné d'une pro Christian procrastination bien étonnante. Alors pour vous répondre là. Par l'État madame Olivia Grégoire ministre déléguée en charge et petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Monsieur le sénateur pieds-noirs, j'ai l'honneur d'essayer de vous répondre. Ma collègue la ministre Agnès Pannier-Runacher est en ce moment même à l'Assemblée nationale sur le projet de loi nucléaire et s'excuse de son absence. C'est pourquoi je vais essayer de répondre à votre question. Pertinente et technique avec les éléments dont je dispose et je ne doute pas qu'elle y apportera d'autres éléments à la suite dans cette fin de journée. Je veux quand même rappeler, indépendamment des des procédures que vous mentionnez et de la saisine et des réactions du Conseil d'État. La mobilisation du gouvernement français. À l'endroit de notre mix énergétique et nos travaux en cours avec la Commission européenne pour faire avancer aussi la réforme du marché du marché À quel point nous nous continuons à investir massivement dans le nucléaire. 4 à 5 milliards d'euros par an au niveau d'EDF. 50 milliards d'euros depuis 2015 pour le grand carénage six EPR de pour 50 milliards d'euros et à l'international, vous le savez avec le Hinkley Point, l'État n'a pas lésiné, il a recapitalisé par 2 fois depuis 2015, EDF près de 4 milliards en 2017, 3 milliards en 2022 et vous le savez, nous construisons des nouveaux réacteurs. Les travaux sont en cours et nous l'avons dit Agnès Pannier-Runacher là dit l'État sera au rendez-vous les Français dans cette situation d'envolée des prix de l'électricité sont protégés face à la hausse des prix de l'énergie. Vous avez mentionné la reine qui, peu importe. Ce qu'on dit le Conseil d'État est quand même un dispositif qui, aujourd'hui, protège massivement nos concitoyens mais aussi une bonne partie de nos entreprises. Je pense aussi au bouclier tarifaire, vous le savez, aux aides énergie. Je voudrais vous ajoutez quelques points. Nous n'avons rien lâcher sur la réforme du marché européen de l'énergie. Après un an de travail et de mobilisation notamment de Bruno Lemaire mais aussi d'Agnès Pannier-Runacher. La Commission a proposé formellement une réforme qui reprend trois demandes françaises majeur à la auquel vous êtes sensible des contrats pour différence entre les producteurs et tous les consommateurs, pour que l'électricité soit vendu à un prix proche des coûts de production nationale l'éligibilité du nucléaire à ces contrats l'éligibilité des installations existantes, comme c'est le cas pour la plupart des centrales en France, c'est une nouvelle encourageante, une bonne base de travail à 7h et notre objectif est qu'elle soit adoptée cette année. Je vous remercie. Mais. Cela passe par des moyens à consolider pour notre outil industriel qui doit accomplir cette ce programme nucléaire à savoir EDF qui doit faire face à une dette colossale de 64 milliards d'euros qui doit faire face à un mur d'investissements dans les années à venir et cela Luc Rémont déclarait lui-même que ce, ce ne sera pas possible si le prix de la reine reste fixé à 42 euros du Umaga Water à Agnès Pannier-Runacher reconnaissait elle-même que le prix de production par EDF était aux alentours de 58 euros. Donc on voit bien qu'il y a un Delta. qui est important et je demande au gouvernement un minimum de cohérence. Vous savez qu'il est encore temps de prendre les mesures nécessaires, d'une part pour ne plus bafouer les décisions du Parlement de piétiner ces décisions. Vous avez actuellement je vous le rappelle, un véhicule législatif à l'Assemblée nationale qui vous permet de les faire de le faire. Je vous invite à vous en saisir. Merci. Merci. Nous en avons terminé. Avec les questions d'actualité au gouvernement. Merci madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à adapter la défense extérieure contre incendie à la réalité des territoires ruraux dans la séance est suspendue.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs est parvenu à l'adoption d'un texte commun. Il y a des CMP qui. L'ordre du jour appelle à 10 la discussion de la proposition de loi visant à adapter la défense extérieure contre l'incendie à la réalité des territoires ruraux présenté par monsieur Hervé Maurey Madame Françoise Gatel et plusieurs de leurs collègues. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Hervé Maurey. Pour l'Union centriste, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à adapter la défense extérieure contre l'incendie à la réalité des territoires ruraux. Je remercie le groupe de l'Union centriste d'avoir demandé son inscription dans l'espace qui lui réserver. Ce texte est le fruit des travaux de la délégation aux collectivités territoriales initiée à la demande du président du Sénat qui a considéré je le cite, qu'il n'est pas normal que la quasi-totalité du budget d'investissement d'une commune soit consacré à la défense extérieure contre l'incendie. Quelle que soit l'importance de celle-ci. Ces travaux ont été menés con collègue Franck Montaugé que je salue et ils ont abouti à la publication en juillet 2021 du rapport défense extérieure contre l'incendie, assurer la protection des personnes sans nuire au territoire. Le Sénat a débattu en séance publique le 5 janvier 2022 à la demande de la délégation aux collectivités territoriales, présidée par notre collègue Françoise Gatel, également auteur de cette proposition de loi que je tiens à remercier pour son appui tout au long de nos travaux. Au cours de ce débat de janvier 2022. Nous avons malheureusement constaté à quel point le gouvernement n'étaient pas conscients de la situation et de ses conséquences sur un grand nombre de territoires ruraux. Ce constat nous a conduits à déposer la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. À notre initiative, l'article 32 de la loi du 21 février 2022, dite 3DS a prévu que le Gouvernement remette un rapport d'évaluation de l'impact de la défense extérieure contre l'incendie sur les communes et ce avant le 1er juillet 2022. Si celui-ci n'a pas été formellement remis par le gouvernement comme le prévoit la loi, ce qui est quelque peu surprenant. Une copie de ce rapport, daté de juin 2022 m'a été remise récemment à la demande du cabinet du ministre de l'Intérieur. Nous nous félicitons que ce document confirme. Une très grande partie des conclusions auxquelles nous sommes arrivés avec took Montaugé. Même si curieusement il a été élaborée sans aucune consultation des maires mais uniquement des préfets. Il est tout d'abord nécessaire de rappeler que la loi du 17 mai 2011 à substituer à la réglementation nationale en matière de défense extérieure contre l'incendie. Le principe d'une réglementation départemental établi par le préfet en concertation avec les élus locaux. L'objectif étant de mieux répondre aux spécificités des différents territoires que ne peut le faire. Une réglementation nationale. Comme le souligne l'excellent rapport de notre collègue Loïc Hervé, rapporteur pour la commission des lois que je tiens à remercier pour la qualité de nos échanges et de son travail. Cette réforme était attendue de longue date par les élus et les parlementaires. Malheureusement, près de 12 ans après l'adoption de cette loi, force est de constater que celle-ci n'a pas répondu à leurs attentes et à la volonté du législateur quant à l'adaptation de ces règles à la réalité des territoires. Elle a au contraire provoqué dans un certain nombre de départements un fort mécontentement des maires. Celui-ci résulte de la mise en application très inégal et souvent très insatisfaisante de la concertation prévue par le décret de 2015. Selon l'enquête que nous avons menée 70% des mères estiment en effet que la concertation n'a pas été satisfaisantes. Un autre aspect insatisfaisant de la réforme et l'absence d'évaluation de la mise en oeuvre au niveau local des règles de défense extérieure contre l'incendie. Celles-ci ont pu en effet être élaboré sans considération de leurs conséquences notamment financières pour les communes chargés de leur application. Il en résulte que ces règlements ne répondent pas toujours ou insuffisamment aux spécificités infra-départementale et ne sont pas proportionnée à la réalité des risques. Dans le département de l'Eure que j'ai l'honneur de représenter. Cela a conduit à édicter une règle particulièrement strict d'une distance de 200 mètres entre les habitations et l'installation d'un point d'eau sur l'ensemble du territoire, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale alors que le risque en termes de propagation n'est évidemment pas le même. Comme l'indique le rapport du gouvernement je cite il n'est pas concevable de demander à des communes peu peuplées de disposer d'une couverture de D. OCI identiques à celles des communes urbaines. Et pourtant, cela peut être le cas. Je sais de quoi je parle. Ce même rapport du gouvernement va plus loin en indiquant que ces règlements devraient même envisager l'absence de couverture plutôt je cite toujours qu'une des aussi coûteuse et pénalisante pour assurer la couverture incendie d'un bâti à risque très faible. Ces règles disproportionnées, ont des conséquences particulièrement préjudiciable sur les finances des communes se sont en effet parfois des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont nécessaires pour de toutes petites communes. Je me permettrai de citer l'exemple de la commune des Botero dans l'heure qui compte 380 habitants. Qui a un budget de 200.000 euros. Les travaux de mise aux normes sur son territoire s'élèverait à 3.600.000 euros. Le rapport du gouvernement rejoint ce constat en indiquant, je cite encore, la récurrence des sinistres en zone rurale et de faible intensité et les investissements demandés aux maires paraît souvent disproportionnés par rapport aux finances de leur collectivité. Je ne saurais mieux dire les maires pour financer ces dépenses de mise en conformité sont donc contraints de renoncer à des investissements importants pour la population et pour lesquels il s'était engagé lors des investi lors des élections municipales. Investissement, qui de surcroît bénéficieraient davantage aux entreprises locales que des bornes incendie ou des bâches. Cette situation conduit de nombreux maires à devoir refuser toute autorisation d'urbanisme enclenchant ainsi un cercle vicieux de baisse de population et donc de ressources et de fermetures de classes. Si certains préfets con conscient des difficultés ont modifié leur règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie pour tenir compte des attentes des élus, cela a été le cas notamment de fois en Seine-Maritime. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Une réponse législative pour remédier à cette situation est donc nécessaire et c'est le sens de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et qui a été enrichi par le travail du rapporteur et de la commission des lois. Ainsi le règlement deviendra un volet du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques pour renforcer encore la nécessaire articulation entre couverture des risques et moyens de lutte contre les incendies, mise à disposition du SDIS. La consultation des élus dans le cadre de l'élaboration du règlement de défense extérieure contre l'incendie sera renforcé et élargi le préfet devra ainsi recueillir l'avis des communes et les intercommunalités, lorsqu'elles sont compétentes en matière de défense extérieure contre l'incendie et prendre en compte ces avis. Une évaluation préalable de l'application du règlement dans le département permettant d'objectiver les difficultés devraient être faites. Par ailleurs cette ce document le règlement départemental n'ayant pas vocation selon l'expression du gouvernement que je cite à nouveau être figé. Il me semble nécessaire que ces règlements puisse être modifié à l'issue du vote de cette proposition de loi s'ils n'ont pas été révisées au cours des 5 dernières années. Cette clause de revoyure doit permettre l'intégration de bonne pratique l'évolution des techniques et des risques, notamment sous l'effet des dérèglements climatiques. Elle devra permettre l'édiction également de règles qui devront respecter plusieurs principes indispensables. Premièrement l'adaptation aux spécificités du territoire je proposerai ici de préciser qu'elles doivent avoir un caractère infra-départementale, le nécessaire équilibre et la complémentarité entre la les moyens des communes et ce des SDIS. La prise en compte de l'impact budgétaire et financier de ces règles sur les finances communales. Comme l'indique le rapport du gouvernement la fixation de ces règles en fonction du matériel et des ressources des SDIS malheureusement trop souvent observées ne peut constituer une règle absolue. Le règlement de défense extérieure contre l'incendie ne doit pas être la variable d'ajustement des moyens des SDIS mais doit également prendre en compte, je cite, une fois encore, le gouvernement la nécessité d'éviter de faire peser des investissements hors de proportion sur les Budgets des collectivités. Enfin ce texte proposera également l'institution d'une commission départementale chargée du suivi de l'application de ces règles. Il s'agira d'inscrire dans la loi la création de cette instance que le ministre de l'Intérieur a indiqué dans un courrier qu'il m'a adressé appelé de ses Celle-ci sera composée de mer et présidée par l'un d'entre eux et sera chargée de l'évaluation de la mise en oeuvre des règles en la matière et de leurs conséquences en matière budgétaire, d'urbanisme et de développement économiques. Cette commission pourra notamment proposer au préfet toute modification du règlement qui lui sera qui tels sont, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais partager avec vous pour vous présenter cette proposition de loi, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois. Monsieur l'auteur de la proposition de loi Madame la cosignataires donc cher Hervé Maurey, chère Françoise Gatel. Mes chers collègues. Pourraient problématisée cette proposition de loi autour de la question de savoir si la défense contre l'incendie est un sujet suffisamment grave pour qu'il soit confié qu'à ceux qui ont la maîtrise de l'art et finalement cette réflexion que nous allons conduire cet après-midi tourne autour de cette seule question. Cette proposition de loi, examiné cet après-midi entendre répondre à un problème lancinant que les communes notamment rurales ne connaissent que trop bien l'exercice particulièrement complexe de leur mission en matière de défense extérieure contre l'incendie. Les difficultés en la matière sont connus de longue date et elles sont connues de nous tous. La consultation du répertoire des questions écrites. De nos collègues députés comme de nos collègues sénateurs corrobore le sentiment qu'un État historiquement velléitaire en la matière des sollicitations lettre morte en promesses de réformes non tenues. Le sujet a trop longtemps constitué. Un irritant. Pour les mères de de de des zones rurales. Si aujourd'hui la passivité l'inertie de l'État en la matière ne semble plus de mise. Nous le devons tout particulièrement à notre collègue Hervé Maurey. Très mobilisés et de manière constante pour la défense des intérêts des communes rurales sur ce sujet, coauteur d'un rapport en 2021 avec notre collègue Franck Montaugé et auteur d'une proposition de loi qu'il nous revient d'examiner cet après-midi. Le cadre juridique applicable à ces missions avaient pourtant été largement revisité par la loi Warsmann en 2011. Pour mémoire, ce cadre prévoit une hiérarchie des normes entre plusieurs documents dont le règlement départemental de défense, secteur contre l'incendie. Le R D D ECI ce règlement départemental en constitue le noeud ces règlements départementaux établi en concertation avec les maires et arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS, doivent tenir compte d'un référentiel national le R et s'impose aux communes dont les arrêtés éventuelle schéma en matière de DEC, ils doivent être conformes au règlement départements. Outre le délai jugé excessif de mise en application de cette réforme. Les difficultés des communes n'ont pas trouvé de solution définitive dans cette réforme. et comme l'ont relevé. Hervé Maurey et Franck Montaugé. Dans leur rapport de 2021. Ces difficultés sont de 4 ordres, premièrement, la concertation est jugé. Allez, disons le mot inégal. la concertation à l'égard des élus dans l'élaboration des règlements départementaux. 2ème 2ème réflexion la couverture du risque et parfois qualifiée de défaillante. L'adéquation entre les prescriptions du règlement départemental et les risques réels. Les premières n'étant toujours pas proportionnée. Au second, en raison de l'évaluation insuffisante et de la complexité des règles surtout du défaut d'adaptation de celle-ci aux spécificités des territoires, notamment en milieu rural combien parmi nous ont entendu parler de la tristement célèbre règle des 200 ou 400 mètres il on parle ici de longueur de tuyau. On approche une des élections sénatoriales. Au mois de septembre mais ce sujet a occupé les élections sénatoriales de 2020 on est 3 ans plus tard et on continue de d'avancer sur ce sujet. sujet. 4ème réflexion le coût financier à la fois budgétaire et en terme de développement économique, notamment lorsqu'une autorisation d'urbanisme ne peut être accordé en raison du défaut de couverture du risque incendie. L'examen en commission de la présente, proposition de loi a permis de retravailler le dispositif initialement. Inventé par notre collègue Hervé Morin afin de le simplifier et de renforcer la portée du dispositif. Finalement on est allé au bout de la réflexion d'Hervé Maurey en faisant du REDD aussi un volet à part entière du Dacr. En effet, les personnes que j'ai auditionnés ont généralement convenu de l'incongruité que pouvait constituer la coexistence du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques le Dacr avec ce règlement départemental de défense et cetera contre l'incendie. De l'Assemblée des départements de France à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France en passant par des échanges avec le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le préfet Alain Taillon lui-même personne n'était vraiment en mesure d'expliquer l'intérêt de la l'existence de deux documents distincts, parfois même Madame la Ministre non pas seulement la coexistence l'hermétisme cité qui pouvaient exister entre les deux et certains travaux sénatoriaux ont démontré. Quelque chose qui paraissait complètement incongrue, je reprends ce terme. Tous portent ainsi à croire que la défense extérieure contre l'incendie. Constitue le parent pauvre de l'organisation des moyens de lutte contre l'incendie. Il a donc il était, je fais d'en faire un document annexe distincts et sans articulation avec le document stratégique que constitue le. Or il me, il me semble que la prise en compte des moyens et des difficultés rencontrées par les communes en matière de défense et qui soit contre un incendie doit justement constitué un n'élément de la stratégie des disent on veut on verra tout à l'heure dans les amendements mais a fortiori avec les changements climatiques nos forces que nous ne connaissons et à. Fortiori avec ces incendies importants que nous connaissons dans beaucoup de de département, même dans des départements qui n'étaient pas exposés jusqu'à la. La détermination et la location des moyens. Ne saurait faire l'économie d'une analyse des forces et faiblesses de la Défense et cetera contre un incendie dans un département le doit prévoir des adaptations de ses prescriptions en fonction des forces et des faiblesses en fonction des réalités du terrain. Ainsi ce volet défense etc contre l'incendie du Dacr constituerait ainsi à porter règlement départemental et sans qu'il soit besoin de le préciser dans la loi les arrêtés communaux et intercommunaux en matière de défense extérieure contre l'incendie qui devraient être conforme à ce nouveau volet du schéma départemental. Cette mesure constitue également une simplification des documents organisant les services d'incendie de secours qui n'ont jamais fait l'objet d'une réforme globale portant vision d'ensemble et stratégique de ses compétences. La procédure d'adoption du volet spécifique de la Défense secteur contre incendie au sein du s'inspire très largement de celle aujourd'hui applicable pour les l'élaboration du règlement départemental. Elle conserve néanmoins 2 apport du dispositif initial. Le projet de document ferait l'objet d'une concertation élargie.

Et d'une évaluation préalable du service public de la Défense extérieure contre l'incendie. Conformément au souhait de l'auteur de la proposition de loi, Hervé Maurey. Le principe d'une révision concomitante du Dacr et son volet relatif à la défense, c'est contre l'incendie serait également conserver. Ce dispositif a été ah harmonieusement complétée par un amendement en de de notre collègue Hervé Morin que nous avons repris en en commission lors de son examen tendant à créer une commission départementale de suivi de la Défense Sector contre l'incendie constitué d'élus, elle aurait pour mission d'une part, de procéder à l'est l'évaluation régulière de l'état de la couverture des risques au regard des points d'eau situé sur le territoire dont elle ferait état dans un rapport annuel et d'autre part de formuler toute proposition d'évolution qu'elle jugerait pertinente cette piste d'évolution évoquées par la direction générale dans un rapport de juin 2022 me paraît consensuel et permettrait aux élus de disposer d'un espace et de, d'écoute et de dialogue avec le service départemental d'incendie et de secours. Nous avons tellement. Été. Attentif à cette proposition de d'Hervé Morin et que nous on avait même prévu une incompatibilité. Entre les élus siégeant dans la commission. De défense contre l'incendie et ceux qui siègent au sein du comité. Ce conseil administration du SDIS pour bien qu'on ait un dialogue éclairé entre d'un côté les maires de communes nous avons rural et d'un autre côté, ce qui dans le département sont en charge de. La lutte contre l'incendie au sein. Du Conseil administration. Des services d'incendie et de secours. Nous avons enfin prévu que le rapport annuel de cette commission puisse faire fonctions sur décision du conseil administration du SDIS d'évaluation préalable du service public de la Défense et cetera contre un incendie l'année précédant la révision du Dacr. Cette modification me paraît de nature à renforcer la place de cette commission qui pourrait se voir attribuer un rôle majeur dans l'élaboration du volet défense extérieure contre l'incendie du Dacr. Elle constitue ainsi une mesure de simplification des évaluations des évaluations aux objectifs similaires n'ayant passé assez nécessairement vocation à être multipliés. Le texte qui vous est proposé. Mes chers collègues. Cet après-midi et donc équilibrée pragmatique et consensuelle pour finir, je tiens à saisir l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de remercier nos collègues sénateurs qui, sur tous les bancs ont permis de cheminer ensemble vers une amélioration significative de la vie des communes rurales en matière de défense extérieure contrôle incendie, je vous remercie. La parole est maintenant Madame Dominique Faure Ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, cher Jean Noël Buffet. Monsieur le rapporteur. Chers Loïc Hervé, monsieur le sénateur cher Hervé Maurey. Mesdames, et messieurs les sénateurs, nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de la niche du groupe UC pour étudier cette première proposition de loi du sénateur Hervé Maurey visant à adapter la défense extérieure contre l'incendie dites des. À la réalité des territoires ruraux. Ce texte résulte notamment d'un important rapport d'information réalisée au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales sur le sujet que je tiens à saluer. Vous l'avez rappelé la DEC il qui est une responsabilité ancienne des maires puisqu'elle date de la fin du XIXe siècle a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle concourt ainsi directement à la sécurité, la protection des populations, c'est son 1er Roger. Elle participe aux bonnes conditions d'intervention des services d'incendie et de secours. Les six en garantissant la sécurité des sapeurs-pompiers engagés, c'est son second objet. Nos travaux doivent donc concilier ces impératifs absolus avec une organisation et un financement de la DEC ECI réaliste efficace et adaptée à nos réalités de terrain. Le déploiement de la DEC, il doit aussi s'inscrire dans un contexte d'évolutions climatiques défavorables. Périodes de sécheresse périodes de forte chaleur propice au développement des feux d'espaces naturels. Ces feux peuvent menacer des habitations désormais partout en France et pas seulement dans les régions méridionales ou dans le Sud-Ouest. À titre d'exemple, un feu de chaume et de Bosquet sur 90 hectares, a détruit des maisons d'habitation cet été 2022 dans l'Essonne communes des Molières pendant une vague de chaleur. Le régime juridique de la DOCX, issues d'une réforme opérée par voie législative et réglementaire achevée en 2015. Vous l'avez dit, qui remplace de simple circulaire datant des années 50. Désormais et ceci constitue un indéniable progrès la DEC il ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée bah basé sur l'analyse des risques et des objectifs de sécurité. Ainsi, les valeurs de volume ou de débit des points d'eau d'incendie ou la distance entre ces points sont précisées dans un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie dit RD déci. Arrêté par le préfet après avoir été élaboré par le six en concertation obligatoire avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DSI. Il doit s'inscrire en cohérence avec le règlement opérationnel du six et le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Le Dacr. Le cadre a donc évoluer vers plus de décentralisation et de prise en compte des spécificités locales. Mais je ne peux que rejoindre les avis exprimés par les différents orateurs, il reste très largement perfectible. La DOCX souffrent d'un déficit de suivi approfondi et régulier. Les élus peuvent rester ainsi sans réponse et sans appui face à de légitimes interrogations sur ce sujet, techniquement complexe. Ce n'est donc pas satisfaisant. La proposition de loi telle qu'elle est issue des travaux de la commission et de son rapporteur comprend de dispositions qui visent à améliorer l'articulation entre le RD des si et le Dacr. Et à créer une instance de concertation de l'ensemble des acteurs concernés notamment les maires avant l'édiction des règlements départementaux. Alors nous souscrivons la philosophie de ces mesures. Mais nous vous proposons de les mettre en oeuvre en intégrant certaines modifications par voie réglementaire. S'agissant de l'article 1, la rédaction du texte aboutit à transformer la nature même du Dacr en créant un volet dédié à la DEC y'prescriptif directement intégrer en son sein. Néanmoins, le Dax hein. Selon le gouvernement. Pas vocation à devenir un document opposable mais doit rester un document stratégique qui vise à effectuer l'inventaire des risques de toute nature auxquelles doivent faire face les 6 et à déterminer les objectifs de couverture de ces risques. La distinction entre le Dacr documents d'analyse et d'orientation et le REDD ECI textes réglementaires spécifiques à la défense contre l'incendie et pertinente. S'agissant de l'article 2, le gouvernement a également fait le constat qui rejoint celui de la commission des lois d'une insuffisante concertation de l'ensemble des acteurs concernés et notamment des mères avant l'édiction règlements départementaux ce défaut ne concerne que certains territoires. Toutefois il n'apparaît pas indispensable que la loi institute une nouvelle commission pour améliorer la concertation alors que le constat de l'existence d'un trop grand nombre d'instances de ce type est unanimement partagée. Je vous propose donc, concrètement, que le gouvernement fasse évoluer le dispositif dans l'esprit de ce qui est proposé par cette proposition de loi suivant 4 axes de travail pour un lancement avant l'été 2023. Ce plan d'action comprend tout d'abord de mesures directement inspirée de cette proposition de loi que nous pourrions travailler en étroite concertation avec Hervé Maurey et le rapport, le Le 1er point de ce plan d'action. Je propose que la question de la DOCX soit discuté au sein d'une instance départementale qui existent déjà. Plutôt que dans une nouvelle structure, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ces SA. Donc je propose que nous élargissons les compétences par voie réglementaire. Je m'engage à ce que la création par décret simple de cette nouvelle prérogative de la CCD. Ça interviennent très rapidement et prennent pleinement en compte cette exigence d'association de l'ensemble des acteurs concernés. Point de de ce plan d'action. Je propose également que nous mettions en place par voie réglementaire. Une liaison entre le RD des si et le Dacr comme vous le demander, sans donner toutefois de porter opposable hausse Acre. Et puis en outre les points III et IV de ce plan d'action. Le point trois, nous allons lancer la production d'un guide méthodologique à destination des six basé sur des bonnes pratiques relatifs à la stratégie de déploiement de la DEC précisant l'appui que les que les six doivent apporter aux collectivités en la matière, notamment pour favoriser le développement des schémas communaux ou intercommunaux de. ECI et puis le dernier point le quatrième enfin nous allons améliorer les synergies entre la réglementation de l'urbanisme et la DRCI afin d'en clarifier les conséquences sur le droit à construire sous la forme d'un référentiel technique. Pour toutes ces raisons. Nous émettons un avis défavorable sur cette proposition de loi. Mais je vous propose d'acter ensemble cette stratégie et ce plan d'action en 4 points en lieu et place des 2 articles proposés. Vous pouvez compter sur ma complète détermination à faire évoluer avec vous le dispositif avant l'été en répondant pleinement aux préoccupations plus que légitime évoquée par le Sénat. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Dans la suite de la discussion générale donc la parole est à madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union centriste pour six minutes. Monsieur

Traitement des urticaire et des irritants, puisqu'hier nous avions Lausanne et aujourd'hui nous avons la défense incendie qui correspondent quand même aux 2 irritant majeur que nous trouvons sur nos territoires et notamment les plus ruraux than plus défense incendie c'est le blocage de toute velléité de construction. Découragement renoncement chute de la. Population et je ne vous fais pas la litanie de moins d'habitants, plus de commerces, pas d'école et cetera et cetera. Vous connaissez ça Shanon cas à remercier Hervé Maurey et Franck Montaugé, auteur d'un rapport à la commission. Des collectivités territoriales. Françoise Gatel, la bonne fée des dits de collectivité. et notre rapporteur Loïc Hervé, cette proposition de loi a été largement. Cosigné. Le constat est sans appel, la réforme engagée en 2011 de la défense extérieure contre l'incendie n'a pas tenu ses promesses, 70% des mères. Interrogée par la délégation estime que la concertation n'a pas été suffisantes, 81% considèrent que leur territoire. N'est que partiellement couvert ce qui signifie que près d'un habitant sur 3 serait hors du Champ de couverture avec 6 à 7 millions de concitoyens. la déci fait peser des contraintes souvent excessive sur les communes sans que celles-ci soient suffisamment impliquée dans sa définition. Depuis 2011, les communes sont chargés du service public mais reste soumise au règlement départemental arrêté par le préfet et doivent contribuer au financement, le règlement départemental et porteur d'un certain nombre de normes inspiré par un référentiel national qui s'applique ensuite au territoire. Or l'évaluation on vous l'a déjà dit des risques en matière d'incendie dans le département. Procès d'un document distinct, ça aurait été évidemment trop somme d'en faire un seul. C'est d'ailleurs ce que la proposition de loi propose les normes définies par les règlements départementaux retrouve donc parfois en total décalage avec les besoins réels et les spécificités. Et on vous a parlé tout à l'heure des 400 ou des 200 mètres nous l'expérimentateur dont tous les jours dans nos départements, et ces coûts sont évidemment. Ces mesures sont évidemment porteuse de coûts importants qui obère la DETR qui devrait servir à autre chose qu'à compenser. C'est D'ailleurs la concertation des élus en vue de l'élaboration de ces normes se relève hein se révèle évidemment insuffisante l'élaboration du règlement départemental rédigé par le SDIS ne requiert qu'une concertation des maires menée de façon très inégale. On vous l'a déjà dit. Quant à la révision, elle est à la discrétion des préfets et le rapporteur vous a expliqué qu'elle était tout à fait aléatoire. Ce constat. Un peu les donc une une réforme, c'est ce que propose la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui l'intégration du règlement départemental de Dessy au schéma départemental je vous ai entendu Madame la ministre et je ne peux pas adhérer à la proposition réglementaire. Sachant les difficultés d'application d'un département à l'autre des mesures réglementaires. Je pense que la loi doit intervenir pour modifier ses dispositifs qui sont des dispositifs légaux et je ne vois pas pourquoi on irait dans un dans une hiérarchie des normes qui est inférieur puisque c'est la loi, il faut que la loi en raison du parallélisme des formes. Le modifie ça supposera que ce texte soit inscrit à l'Assemblée nationale mais j'imagine qu'avec la position que vous venez défendre vous devenez de défendre à la tribune. Ça ne va pas être chose facile mais on peut quand même. Essayer. D'autant que cette proposition est vraiment. Tout à fait intéressante et tout à fait indispensable. Pour rendre les choses plus faciles pour nos départements ruraux. Rien ne vous empêche dans l'intervalle, de prendre une circulaire. montrez-nous votre bonne volonté, prenez votre circulaire et puis laissons la loi parcourir son chemin. Les deux choses ne sont pas incompatibles entre elles. Donc je pense qu'on peut mener les 2 combats de front, plus ce sera utile pour nos territoires ruraux plus ça rendra la vie facile aux communes les plus rurales moins ça leur coûtera d'argent et plus ça donnera des lignes de conduite aux préfectures et mieux ça ira. Je voudrais simplement ben la Ministre dans la minute qui me reste à peine cette ce texte à la discussion budgétaire que nous avons eu lors de la discussion budgétaire. En 2022 pour le budget 2023. J'ai été extrêmement surprise que des amendements de bon sens de la première partie de la loi de finances de notre collègue à Catherine Loisier notamment sur des mesures fiscales d'aménagement et d'entretien des forêts ne soit pas du tout pris en considération. Je pense qu'il faut travailler en commun avec le ministère de l'agriculture et des forêts pour ajuster avec votre ministère et le ministère du Budget. Des mesures intelligentes et coordonnée parce que la défense incendie. C'est aussi l'entretien des forêts et je pense que les 2 sujets sont liés et que là aussi il y a un travail qui doit être fait en amont pour préparer la prochaine loi de finances parce que je ne vois pas comment on peut dissocier les 2 sujets, à la fois la défense incendie c'est normal à la fois la protection puisque vous avez vous-même annoncé et et donner l'exemple d'un cas qui, je crois, se trouve dans le département de notre président bien-aimé et donc en conséquence de quoi, je pense que les sujets sont liés je. Je pense que la loi est importante, si vous prenez une circulaire ou un règlement dans l'intervalle très bien les deux, les deux procédures doivent se poursuivre en parallèle et en attendant notre groupe votera avec enthousiasme cette proposition de loi, je vous remercie. La parole est à la présidente Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues je ne surprendrai personne en disant combien les incendies dramatiques qui ont eu lieu au cours de l'été dernier ont marqué les esprits et très singulièrement la population girondine et Madame la Ministre, vous étiez d'ailleurs venu sur place pour rassurer la population et les communes de votre soutien. Ces incendies ont imposé pour certains une prise de conscience abrupte des risques encourus sur nos territoires et le réchauffement climatique pour le dire très sainte éthiquement va démultiplier ses risques recommandant toujours plus de vigilance et d'anticipation et risque qui vont nécessiter en 1er lieu des moyens matériels et humains et c'est en ce sens que nous aurons bientôt à examiner ici une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Parce qu'au Sénat, nous avons cette culture de l'anticipation toutefois en préalable du volet opérationnel. Il existe aussi un volet planification qui nécessite de mobiliser et d'actualiser des outils juridiques au enfin que ces dernières répondre au mieux à la réalité de nos territoires. Je tiens donc à saluer l'initiative des auteurs de cette proposition de loi, Hervé Maurey et Françoise Gatel. Nous avions débattu au mois de janvier 2022 sur les conclusions du rapport d'information défense extérieure contre l'incendie, assurer la protection des personnes sans nuire au territoire rendu par Hervé Maurey, ainsi que Franck Montaugé et je profite de cette prise de parole pour saluer leur investissement sur ce sujet. Il avait souligné que de nombreux maires nouvellement élus reconnaissait ne pas être en capacité de s'approprier la matière relevant de la DSI et de porter une appréciation sur cette politique à l'échelle de leur territoire par manque de compétences techniques. Mon collègue Éric Gold étaient d'ailleurs intervenues au nom du RDSE pour souligner que l'une des principales difficultés que pose la DSI réside dans ces règles complexes et insuffisamment adaptée aux réalités de nos communes. Ce fut une remarque largement partagée par notre assemblée nos administrations locales font donc face à un régime juridique particulièrement exigeant lequel résulte du caractère périlleux de l'activité qu'elle a des, si, il faut néanmoins trouver les moyens de le simplifier et de permettre un meilleur enchevêtrement des outils. Je pense que cette proposition de loi et participe, et c'est l'occasion de souligner le travail d'orfèvre du rapporteur notre collègue Loïc Hervé, plutôt que de prévoir la concomitance de la révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, comme le prévoit le texte initial la réécriture par la commission de l'article 1er vient intégrer le REDD si hausse Acre afin d'assurer effectivement une concomitance des 2 documents. Bien entendu, il est à ce stade. Difficile de mesurer l'impact de cette modification mais je ne doute pas qu'elle participera à l'effort de simplification et d'efficacité de notre droit dans ces conditions et pour ces raisons, le groupe RDSE se prononcera unanimement en faveur de cette proposition de loi, je vous remercie.

monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Assurer la protection des personnes sans nuire au territoire. Voilà tout l'enjeu de la défense extérieure contre l'incendie depuis l'application du décret de février 2015. C'est une conciliation difficile que j'appelle sincèrement de mes voeux dans mon département grâce à grâce à cette proposition de loi. Dans l'heure, il ne se passe pas une semaine sans que je ne sois confrontée lors de mes visites de communes à l'impossibilité de mise en oeuvre du règlement départemental de défense incendie soit parce que c'est foncièrement irréalisable soit budgétairement intenable. Ce règlement élaboré en 2017 prévoit uniformément pour nos 585 communes très rurales. Un point d'eau tous les 200 mètres sans prendre en compte la diversité de l'habitat qui peut être souvent diffus dans la plupart des communes de l'heure. Pour l'une, le manque de débit rend impossible l'installation des points d'eau supplémentaires pour d'autres c'est l'absence de foncier disponible qui va bloquer l'installation des bâches citernes et pour d'autres encore. L'installation de toutes les préconisations de la défense incendie va littéralement siphonné le budget d'investissement de la commune pour plusieurs années. Enfin quand la mise aux normes n'est pas possible. Les élus sont contraints de bloquer, de nombreux permis de construire, source d'incompréhension et de conflits avec leurs concitoyens et vivent leur mandat avec la crainte de l'engagement de la responsabilité de la commune en cas de sinistre. à l'origine, c'était d'abord élaboration déconcentrée des règlements départementaux était voulue pour mettre en oeuvre une défense incendie évolutive au plus près de la réalité des territoires et en concertation avec ceux-ci. Force est de constater que l'objectif a manqué sa cible, dont certains dans un certain nombre de départements. Le dernier rapport d'évaluation du gouvernement de juin 2022, en application de la loi 3DS liste Sedif dysfonctionnements reconnaît des situations de crispation dans certains départements essentiellement runo ruraux et préconise pour ces cas emblématique la révision et l'adaptation des règlements au niveau infra-départementale. L'heure Lulu est l'illustration parfaite de l'imposition d'une défense incendie je cite coûteuse et pénalisante pour assurer la couverture incendie d'un bâti à risque très faible et où les distances et d'intervention la rendent parfois inopérante. Mon département avait déjà été tristement cité il y a plus d'un an dans un débat que nous avons eu. Dans cet hémicycle avec madame bah. Le montant des dossiers de TER à ce sujet, 20 fois supérieur à la moyenne des autres départements témoigne du poids disproportionné de la défense incendie pour l'État, le département et les communes pour un résultat très en-deçà des objectifs du règlement départemental alors que d'autres départements ont pu trouver des issues à ces situations de blocage par des systèmes de dérogation d'évolution des doctrines de lutte ou tout simplement une révision de leur règlement départemental comme 17 d'entre eux l'ont déjà fait. Je déplore que cette situation reste bloquée dans l'Eure. Vous le comprendrez mes chers collègues, je suis donc favorable pour établir l'esprit d'une défense incendie déconcentré évolutive à ce que la loi encadre et prévoit la concertation avec une une périodicité enfin qu'il existe des issues en cas de règlement trop uniformes et trop rigide. L'intégrer dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est une mesure cohérente, tout comme l'obligation de révision dans l'année qui suit la l'adoption. L'adoption de ce texte pour ceux dont la révision est trop ancienne. Comme le souligne à propos le rapport. Du gouvernement l'effort en matière de défense incendie doit être pondéré par l'analyse pragmatique et locales du risque, la prise en compte de la disponibilité de la ressource et par la nécessité d'éviter de faire peser des investissements hors norme sur les Budgets des collectivités. Enfin, la récurrence des feux d'une ampleur que nous n'avions pas l'habitude de voir nous invitent à repenser le modèle de défense incendie afin qu'il soit adapté à nos ressources et à nos moyens pour garantir la sécurité de nos concitoyens et de nos sapeurs-pompiers et je soutiendrai donc sans réserve ce texte cette proposition de loi de mon collègue Hervé Maurey. Si cher collègue. La parole est à monsieur Pierre Jean Vergnes, Eulen pour le groupe les indépendants pour 4 minutes. Monsieur le président. Madame la ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission et notre chère collègue qui a qui est l'auteur de de la PPL. La défense extérieure contre l'incendie et. Parfois mal identifié souvent assez mal comprises. C'est pourtant ça a été dit un enjeu essentiel de sécurité publique qui permettrait concrètement aux pompiers qui se rendent sur un feu d'effectuer dans les meilleures conditions possibles. Leur mission. Elle a pour objectif de garantir la ressource et une alimentation correcte, des points d'eau incendie d'assurer une localisation et une répartition efficiente de ces points d'eau. Il revient aux maires et aux présidents d'intercommunalités d'assumer cette compétence et cette responsabilité elle doit se faire main dans la main entre les élus locaux et les SDIS. Jusqu'en 2011, la déci relever d'une logique nationale avec des normes applicables 2 fassions uniforme et qui pour le coup était extrêmement éloigné des spécificités locales et du terrain. En 2011. Comme président d'un SDIS comme maire. J'ai apprécié d'avoir eu la souplesse de bâtir des documents à l'échelle départementale. C'était une première avancée extrêmement importante, ce fut et c'est toujours un gros travail entre les pompiers, les maires ou les présidents d'interco pour aboutir à un arrêté communal. Les résultats sont plus ou moins probant comme l'dit le rapporteur sont assez inégaux selon selon les départements et le les travaux qui ont été menées par les SDIS. Les maires n'ont évidemment et surtout dans les communes rurales pas toujours les moyens humains et matériels nécessaires pour la la réalisation d'un tel document qui reste, même pour les spécialistes, reconnaissons-le, assez complexe. Et avec différents interlocuteurs notamment quand la distribution de l'eau et confiée à d'autres sociétés en affermage des difficultés pour avoir des informations, des difficultés pour engager un dialogue sur ce sujet. Si cette réforme a permis de vraies avancées. Elle n'a pas eu tous les effets escomptés. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, une grande partie des maires ont estimé à juste raison, ne pas avoir été assez associés en amont à l'élaboration des nouvelles règles. Ce qui fait que sa mise en oeuvre. On a été. Compliqué, dans un certain nombre d'endroits. Puis il y a le volet financier. Les communes évidemment font face dans ce cas là, des coûts d'investissements très importants et si on prend une commune qui a des hameaux où il faut mettre des points tous les deux les 400 mètres. on comprend bien, tout ça engendre des coûts qui des fois ne sont pas tenables alors pardon de la comparaison, mais il y a il y a il y a des systèmes tels que les investissements sur les églises au Patrimoine ou les préfectures permet des déplafonnement pour avoir des financements à hauteur de 100%. C'est peut être vers ce type de solution qu'il faut se retourner aussi. Nous saluons le travail qui a été menée et les dispositions de la proposition de loi modifié par la Commission, qui prévoit de remédier à ces difficultés en incluant le règlement départemental au sein du schéma. Départemental d'analyse et de couverture phallus Dacr fameuse. Tout en associant davantage les maires à leur élaboration. Ces dispositions vont apporter une plus grande souplesse notamment sur les territoires ruraux. La création de la commission permettra davantage de cohérence dans la couverture des risques. Un bilan annuel servira des vieux d'évaluation préalable qui facilitera à terme l'application de ces mesures. Ce texte répond aux attentes des élus locaux mais nous devons et je sais que c'est l'esprit de chacun ici rester vigilants à ne pas perdre de vue l'objectif 1er de la défense extérieure contre l'incendie, c'est-à-dire améliorer la sécurité publique et les capacités des pompiers à lutter contre le feu. Les sénateurs du groupe les indépendants voteront en faveur de la proposition de loi. Merci de votre attention. Merci cher collègue. La parole est à madame Monique de Marco pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans son dernier bulletin, le Bureau de recherches géologiques et minières alertent sur le faible niveau des nappes phréatiques. 80% d'entre elles auraient un niveau inférieur à la moyenne et 45% des nappes ont rejoint le niveau inquiétant de niveaux bas voire très bas. Depuis l'Automne, les pluies ont été insuffisamment insuffisante pour reconstituer ses nappes. La situation ne va pas s'améliorer d'ici le printemps et le renouveau végétale sans qu'on puisse compter sur la contribution Ingrid du manteau neigeux dans les Pyrénées qui est trop faible. Fait nouveau, cette situation touche l'ensemble du territoire. Et laisse augurer un été 2023 encore plus sec que ne fut l'été 2022 et ceci dans toutes les régions. Ce n'est pas sans incidence sur le risque incendie dans les espaces naturels mais également dans les communes bordant ces espaces. En Gironde, nous avons fait la douloureuse expérience. L'été dernier. Dans ce contexte, l'importance de la défense extérieure contre incendie doit être réaffirmée. C'est donc dans cet état de vigilance que nous abordons l'examen de cette proposition de loi visant à adapter la défense extérieure contre un incendie à la réalité des territoires ruraux. Il est vrai que depuis sa modification pas la loi de simplification du droit de 2022 1011. L'application du nouveau cadre de la DEC, il n'est pas satisfaisante. Le rapport d'information de 2021 souligne la faible mise en conformité des communes, la loi faute de schéma communaux nécessaire. Cela en raison du déficit de concertation observée au moment de l'élaboration des règlements départementaux des défenses extérieure contre l'incendie mais aussi et surtout en raison du coût de la mise en conformité largement démontré dans le rapport. Il est indéniable que pour de nombreuses petites communes la création ou l'entretien des bouches d'incendie est une charge exorbitante. Elle s'ajoute à cela l'entretien des canalisations d'eau courante auquel sont rattachés. Cette proposition de loi n'offre aucun instrument financier aux communes. Nous considérons qu'un plan national d'accompagnement financier devait être mis en place pour répondre à cette problématique transversale de la compétence communale de l'eau. Sans cela, toute initiative, quelle qu'elle soit semble vaine. Et je ne vous ai pas entendu Madame la Ministre aborder justement ce sujet de financement donc vos propositions. En définitive, l'efficacité des mesures proposées par nos collègues centristes pour l'amélioration. L'application de la DEC y'dans toutes les territoires et très difficile à évaluer. D'un côté la clarification des procédures de concertation la création d'une commission consultative dédié et l'obligation d'information des communes en amont de l'adoption du règlement réglementation départementales vont d'évidemment dans le bon sens et vont permettent de mieux accompagner les mères. Mais d'un autre côté. Les dispositions qui permettent aux communes rurales de déroger aux normes de sécurité aujourd'hui prévue par le référentiel national il risque de faciliter la délivrance de permis de construire en zone non sécurisée et donc l'étalement urbain. Ce référentiel Fisc fixe les besoins objectifs en point d'eau et bouche d'incendie pour les pompiers. Il y introduire des dérogations territoriale ne risque-t-il pas d'affaiblir la capacité d'action. Quel est le sens également de la création d'évaluation préalable des coûts financiers urbanistique et de développement économiques. Si ce n'est de justifier les dérogations pour les communes aujourd'hui moins que ça se poser au risque incendie. Mais seront-elles à l'abri, demain. Cette solution reporte la charge sur les générations futures. Nous avons donc déposé un amendement visant à clarifier cela. Dans l'intérêt des communes. Nous proposerons enfin une piste alternative destinée à alléger leurs charges. Il s'agirait comme le proposait d'ailleurs le rapport d'information de faire l'inventaire de tous les points d'eau incendie privatifs pour les intégrer au schéma communaux. Et les substituer à des bornes communal. Cela y intégrer les piscines privées ou toute étendue d'eau non potable à condition qu'elle ne porte pas atteinte aux réserves non. Nappes phréatiques, en tout état de cause nous abstiendrons donc de voter. Je vous remercie. La parole est à monsieur Dominique Théophile pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. La proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey. Entend adapter la défense extérieure contre l'incendie à la réalité des territoires ruraux. Elle s'inspire du rapport d'information que vous avez commis en août 2021 avec le sénateur Franck Montaugé. Au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Ce rapport consacré à la réforme de la défense extérieure contre l'incendie, la déci intervenu en 2011 formulé une série de recommandations permettant de faciliter son application dans les territoires ruraux recommandations dont certaines trouvent ici leur traduction législative. Dans sa première mouture, le texte prévoyait une révision du règlement départemental de défense accès au contrôle incendie dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi et après chaque révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Il prévoyait également une meilleure concertation entre les élus et les acteurs concourant à la DSI et proposé de faire procéder. L'établissement de ce règlement d'une évaluation de ses conséquences financières urbanistique et économiques. La commission des lois a profondément remanié ce texte qui propose désormais une fusion du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie et du schéma départemental d'analyses de couverture des risques en faisant du premier un volet du second. La commission a également voté la création d'une commission départementale de suivi de la DSI chargé de procéder à l'évaluation régulière de l'état de la couverture des risques au regard des points d'eau situé sur le territoire et d'adresser aux préfets de département des propositions d'évolution si l'ambition de ce texte nous semblent parfaitement louables hein. Pour ne pas dire nécessaires au regard des difficultés rencontrées dans de nombreux territoires et par de nombreux maires et alors que le risque d'incendie se fait de plus fort chaque année en raison du réchauffement climatique et des sécheresses à répétition. Notre groupe est partagé sur la méthode proposée. Outre les quelques doutes que nous avons sur ce qui pourrait relever du domaine réglementaire plutôt que du domaine législatif, je pense notamment à la création à la création d'une commission départementale de suivi à l'article de d'autres nous semblent plus contestable. Je pense notamment à la fusion des 2 dispositifs de nature et de fidèles finalités différentes, le SIDA et le R D. Par ailleurs, et c'est là peut-être que ce qui nous retient le plus. Il nous semble que ce débat trouverait sa place lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre Lindt Tisley intensification et l'extension du risque d'incendie, porté notamment par notre collègue Jean par notre collègue Jean Bacci. Ce texte d'une petite quarantaine d'articles et d'une portée plus large que celui que nous examinons cet après-midi et qui s'inscrit par ailleurs en cohérence avec la stratégie nationale et territoriale de lutte contre les incendies de forêt voulue par le président de la République nous apparaît être le véhicule législatif le plus adéquate et le plus à même de prospérer. Car la multiplication des textes sur le sujet. S'ils ont ambitionne. Tous de rendre la défense extérieure contre l'incendie plus lisible dans les territoires ne concourent pas à la lisibilité de nos travaux. En conséquence, le groupe RDPI s'il salue le travail de ses auteurs s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie.

C'est le président, madame la Ministre. Monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur, madame et monsieur les coauteurs et permettez-moi d'y associer un coauteur putatif mon ami et collègue Franck Montaugé au Sénat nombres de nos travaux sont transpartisan. Et le sujet de la lutte contre l'incendie. Et de la protection de nos concitoyens contre le risque incendie fait partie de ceux-là. En tant qu'acteur majeur de la lutte contre l'incendie. L'action des pompiers est propice à un travail consensuel au sein de l'hémicycle et il faut le dire nos leurs valeurs, leurs engagements. La reconnaissance que nous souhaitons leur apporter et partager sur tous les bancs de la Haute Assemblée. Outre les nombreuses PPL, mes chers collègues qui irriguent notre travail parlementaire. J'en ai dénombré au moins 4 entre 2000. Le 21 dès 2022. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le statut des sapeurs-pompiers. Je voudrais saluer le travail de notre collègue Roland Courteau sur le régime de retraite, ce qui permet d'ailleurs de vous, de vous rappeler que nous avons eu beaucoup d'amendements. Dans le cadre du PLFSS rectificatif. Que nous avons examiné pendant ces 10 jours et 10 nuits sans désemparer et cela a été je crois par nos collègues notamment de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers. Alors madame la ministre. Vous nous dites, dans votre intervention. La ministre, ce qui est moi. Vous nous dites, dans votre intervention que bon finalement vous allez vous inspirer de ce de ce travail et que vous allez le transformer en décisions gouvernementales à caractère réglementaire. Permettez au législateur que nous sommes. De poursuivre leurs travaux et je tiens à vous dire que je ne doute pas, nous ne doutons pas de votre bonne volonté, en l'espèce mais finalement nous préférons décider par nous-mêmes ce qui est l'intérêt. De notre pays et en l'occurrence des communes concernées. De missions donc ont été. Également créer une mission de contrôle sur la prévention, la lutte contre une intensification et l'extension du risque incendie et la coupe de la commission affaires économiques et de la commission de l'aménagement des territoires. 70 propositions ont été traduits dans une PPL qui arrive en séance début avril et cette mission d'information par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Cette dernière a abouti à un rapport de Franck Montaugé, Hervé Maurey Hervé Maurice son compte j'ai vous le mettrez dans l'ordre que vous voudrez. En juillet 2021 une PPL a également été rédigée pour reprendre les mesures d'ordre législatif et cette une de ces mesures que nous examinons en particulier, une des 4 mesures que nous examinons aujourd'hui un débat était organisé en janvier 2022 suite à la remise du rapport et c'est vrai que le gouvernement à l'époque. Avait indiqué avoir mandaté la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour la réalisation d'un audit dont la publication, sans faire de ma part est encore attendu mais aucun engagement précis du gouvernement n'a été formulée pour prendre en compte les constats et les propositions du rapport sénatorial. en revanche mis en exergue la déconnexion une sorte de déconnexion de l'exécutif. Quant à la réalité sur la situation. Qui nous intéresse. Mais j'ai bien entendu Madame la Ministre vos engagements en l'espèce. En effet, mes chers collègues, de nombreux élus locaux font état d'une inadaptation à leur territoire des obligations en matière de défense extérieure quand un incendie il y aurait d'ailleurs plusieurs millions de nos concitoyens qui ne serait pas. Correctement protégés contre le risque incendie, bien que nous ne bénéficions d'aucune statistique sérieuse sur la couverture effective du risque incendie. Il est probable il est probable fort probable que les zones rurales qui est qui connaissent l'habitat le plus déconcentré soit plus particulièrement affectés par cette réforme quand l'on sait qu'un tiers de la population vit dans une commune rurale, le nombre d'habitants concernés donc forcément inquiétant, la compétence de la défense extérieure incendie comme la police spéciale qui est rattaché relève du maire ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Si elle a été déléguée les difficultés soulevées par les élus locaux sont surtout liés à la prise en charge, cela a été dit à plusieurs reprises de cette défense pour des petites collectivités, qui ont du mal à faire face finalement aux dépenses d'investissement absolument nécessaire. Les impacts financiers pour la mise aux normes de la DSI ont conduit certaines communes à reporter des projets pourtant attendu par leur population, et les impacts en terme d'urbanisme a également été pointé il convient pour cela de revenir sur l'évolution de la politique de la DSI reposant sur une logique nationale indifférencié. Elle a été réformée par la loi de 2011 qui a mis en place des déclinaisons départementales. Cela été aussi rappelé à plusieurs reprises l'organisation néanmoins de la concertation n'ayant pas été prévu par la réforme de 2011, elle a été laissé de facto à l'appréciation. Souveraine, mais parfois inégalitaire des préfets. Il y a effectivement des des expériences très différentes en la matière que nous connaissons de département à département le texte. Mes chers collègues qui nous est soumis à ce jour prévoit la révision du règlement départemental dans un délai restreint avec une meilleure concertation des élus et acteurs de la DSI donc. Ce texte est un progrès par rapport à la situation. Actuelle c'est une mise en cohérence qui permettra d'apporter une vision plus globale et d'optimiser les moyens de lutte contre le l'incendie. Le dynamisme des travaux du Sénat témoigne de l'engagement de notre chambre consciente du service de sécurité rendu à nos concitoyens à défendre ardemment les conditions de travail des sapeurs-pompiers et à protéger notre population contre le risque incendie. Nous sommes très attachés. Madame la Ministre à la concertation et notre groupe est nécessairement favorable, favorable aux dispositions contenues dans ce texte néanmoins avec notre collègue Franck Montaugé qui a fourni un excellent travail. Nous allons essayer encore par nos amendements, de l'améliorer, mais je le dis à l'ensemble des bancs de cette assemblée, hé bien le groupe socialiste sera à la hauteur de l'ambition qui a été porté par les coauteur de cette proposition de loi, je vous remercie. Merci monsieur le président. La parole est à madame Céline Brulin, pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Cette proposition de loi de nos collègues. Gatel est la bienvenue et je le dis d'emblée nous la soutiendrons. Car la défense extérieure contre l'incendie peut considérablement empoisonner la vie des communes rurales. Elle contribue. Au sentiment que plus l'État abandonne ses propres missions, en particulier celle d'assurer l'égalité républicaine, plus il se fait exigeant et procédurier à l'égard de nos communes. Les maires souhaitent assurer la protection des populations. Mais comme le dit le rapporteur Loïc Hervé, à juste titre la déclinaison départementale. Du référentiel national de défense extérieure contre l'incendie sans concertation avec les élus restrictif dans son schéma et parfois disproportionnés par rapport aux risques réels va à l'encontre même des objectifs de protection de la population. Cela a été le cas dans mon département de la Seine-Maritime avant qu'avec de nombreux maires nous obtenions précisément une révision de ce règlement départemental dans de trop nombreux départements en effet la déclinaison départementale du référent national ne prend pas en compte les réalités de terrain alors que c'est précisément sa vocation, il nous a fallu initié une consultation des communes, ce qui n'avait pas été fait ou si peu, par les services de l'État. Madame la ministre, il nous a fallu multiplier les interventions auprès du préfet comme auprès du gouvernement, gouvernement, trop souvent sourd à ces interpellations en prenant appui sur le témoignage de près de 180 communes et l'expertise des mères. Il nous a fallu pointer les aberrations comme celles écoutez-moi bien que subissait par exemple des communes du bord de Seine, se voyant refuser la prise en compte du fleuve et la possibilité de s'y alimenter en eau dans leur schéma communal ou encore le refus de prendre en compte la densité de l'habitat considéré comme urbaine dès lors qu'elles étaient entre les poteaux d'entrée et de sortie de bourse qui a évidemment des conséquences sur les 200 ou 400 mètres. Il nous a fallu alerter sur l'impossibilité objective. De se conformer à la DSI faute de débit d'eau suffisant de foncier nécessaire pour installer bâches ou citernes enterrées et plus encore sur l'impossibilité financière. Certaines communes étant contrainte d'y consacrer le budget d'investissement d'au moins un mandat entier, il nous a fallu mettre en avant des propositions simples, pragmatiques facilement réalisables et peu coûteuse dans un recueil remis au préfet au SDIS pour faire la démonstration que des solutions de bon sens exister, bref il nous a fallu beaucoup d'énergie et plusieurs années de mobilisation mais malheureusement ce que nous sommes parvenus à faire en Seine Maritime ne l'est pas partout. Or je viens d'entendre enfin d'où l'utilité à mes yeux de cette proposition de loi. Alors je viens de vous entendre madame la ministre et je souhaite vous alerter sur la manière dont risque d'être accueilli votre refus d'apporter votre soutien à cette proposition de loi au profit, si je peux le dire en c'est à terme de vagues engagements à travailler sur des mesures réglementaires car voilà des années maintenant que les élus de tous bords vous alerte sur ce sujet. Suite au rapport qui a été évoquée de nos collègues Montaugé. Est mort et nous avons eu ici même un débat où nous avions tous alerter vos de vos prédécesseurs sur la nécessité de donner consigne aux préfets de faire brûler. J'ai les choses, rien n'a bougé. De même, le rapport que le gouvernement de par la loi et censés remettre au Parlement ne l'a toujours pas été on s'en étonne bref. Je crois qu'il est nécessaire d'en passer par la loi, ça n'épuisera pas tout le sujet Madame la Ministre assurez-vous parce que je crois que demeure le sujet financier parce que même avec les assouplissements que nous pouvons apporter à la défense incendie ce ça reste extrêmement lourd pour les communes et nous aurons là aussi de nombreuses propositions à vous faire pour que ça pèse moins sur les communes et peut être par exemple plus sur les compagnies d'assurances qui ont tout à gagner au fait que la défense incendie soit mieux assurée partout dans le pays. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. 10 ans seulement après l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit, de nombreuses insuffisances ont été relevés en matière de défense extérieure contre l'incendie. Conduisant le Sénat évaluer la réglementation applicable travaux qui ont fait l'objet en juillet 2021. Du très bon rapport de nos collègues Hervé Maurey et Franck Montaugé, que je salue et qui dans la continuité de celui-ci, ont conduit à la proposition de loi d'Hervé Maurey et de Françoise Gatel, que je salue aussi que nous nous apprêtons à examiner. Du fait des enjeux juridiques et financiers importants qu'elle revêt pour les communes en particulier pour celles qui sont rurales la DSI est une préoccupation sensible pour les élus locaux. Les règlements départementaux de défense extérieure contre l'incendie, adoptée en 2017, dans la majeure partie des départements ont permis des avancées. Il s'avère néanmoins que les mises en conformité impacte fortement les communes par une responsabilité accrue des maires chargé des pouvoirs de police administrative spéciale par la nécessité d'identifier les risques de dimensionner les besoins en eau par la mise en oeuvre d'un service public de la DSI chargé de la création de l'Aménagement et du contrôle des points d'eau incendies par la prise d'arrêtés communaux ou intercommunaux listant a minima les points d'eau incendie et enfin par la création de nouvelles charges dévolues aux communes notamment financières. Les enjeux de la réforme était important. L'objectif étant de diminuer le recours à une gestion nationale de la DSI et de privilégier une approche réaliste et opérationnel mettant en adéquation les risques identifiés localement et les besoins en eau. Les règles sont toutefois jugés localement comme sévère et difficile à mettre en oeuvre. D'où la nécessité d'adapter le cadre actuel. Qui plus est dans un contexte de réchauffement climatique et de recrudescence des incendies. La mutualisation, à l'échelle des territoires constitue un véritable levier. Elle est une source de rationalisation pour la planification et les achats, la maintenance et le contrôle périodique des points d'eau incendie. ce levier peut présenter l'Avantage, de rapprocher au même niveau la gestion du service public de l'eau et de la DSI enfin il réduit le nombre d'interlocuteurs facilite l'échange et le partage de données notamment avec les SDIS. En conclusion, le texte que nous examinons constitue une avancée que je salue. L'amélioration de la réglementation applicable à des si est une nécessité pour faciliter son exploitation il y a lieu d'inciter à l'effort de mutualisation dans l'Ain territoires ruraux pour assurer la déci par la mise en commun des ressources que chacune des communes. De son côté consacre à ce domaine. Juste le moment opportun aussi de renforcer l'éligibilité des travaux en matière de ici aux dotations de l'État et pourquoi pas de redéfinir un outil d'analyse de risques des 6 communal qui soit plus accessible. Je voterai bien sûr avec enthousiasme ce texte. Je vous remercie. La parole est à monsieur Édouard Courtial pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Merci monsieur le président. Monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues alors que notre pays a connu son année la plus chaud depuis le début des enregistrements, causant une sécheresse exceptionnelle et que 80% des nappes phréatiques atteigne un niveau inquiétant, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et que j'ai cosigné un écho bien particulier. Elle fait suite à la saisine par le président du Sénat de la délégation aux collectivités territoriales. D'une mission d'information sur un sujet que les communes rurales ne connaissent que trop bien celui de la Défense extérieure contre l'incendie. Là. Aussi, comme on l'appelle vise à garantir l'alimentation en eau des moyens des SDIS par l'intermédiaire des points identifier spécialement pour cela. Cette politique publique a longtemps été encadré par voie réglementaire et a ensuite été réformé réformé en 2011 par voie législative avec la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit disons après l'entrée en vigueur de cette loi, de nombreuses insuffisances ont été relevés ainsi que. La nécessité de mieux associer les communes conduisant le Sénat a procédé à l'évaluation de la réglementation applicable dans ce rapport du 8 juillet 2021. Notre collègue Hervé Maurey. Dans la continuité de ce rapport et pour répondre aux difficultés d'application de des règles rencontrés sur certains territoires. La PPL 3 à modifier les modalités de révision des règlements départementaux de UCI qui quatre cet exercice pour prévoir une meilleure prise en compte des intérêts communaux Avec l'auteur de la proposition de loi la nécessité de renforcer la cohérence entre le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie et le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. La commission a néanmoins estimé le dispositif proposé insuffisamment opérationnelle. Là en conséquence simplifié et renforcer sa portée ont prévoyons que la RD, quatre organisations départementales de défense extérieure compte l'incendie constitue un volet à part entière du SDA un document stratégique pluriannuel de la couverture des risques de toutes natures présentant les garanties nécessaires d'associations et de concertation des élus locaux pour son établissement. Chers collègues, nous le savons, l'eau devient au même titre que l'énergie. Un enjeu majeur, y compris pour les collectivités locales pour faire face à sa pénurie. En outre, toute mesure qui peut conduire à. Une plus grande prise en compte des réalités locales à une simplification et à davantage de concertation doit être. C'est pourquoi j'appelle évidemment à l'adoption de cette proposition de loi. Merci, chers collègues, la discussion générale est Close. Nous allons examiner le texte de la commission en commençant par l'article premier jet de demandes de parole, monsieur Montaugé. merci Monsieur le le président. Cher collègue, Madame la Ministre mon nom a été. Évoqué plusieurs fois au cours de cette discussion générale à ça m'était jamais arrivé. Je ne suis pas signataire de ce de ce texte. Donc je voudrais rassurer tous ceux ici qui pourraient penser que j'ai voilà du dédain peu d'intérêt pour le sujet vous vous en doutez tout tout le contraire a notamment par rapport au travail que j'ai pu réaliser avec. Mon confrère Hervé Maurey sous sous l'égide de la présidence de la délégation. Aux collectivités locales et la décentralisation, conduite par par Madame Gatel. Voilà je je regrette je je le dis sans acrimonie, sans amertume ni quoique ce soit. Je regrette ne n'avoir pas été sollicités. Pour signer ce texte.

Mon petit cas personnel et sans importance. Mais je trouve que c'est c'est embêtant par rapport à l'esprit. Que que moi je me fais et que j'ai compris hein. Travaillant depuis près de 10 ans dans cette institution. L'esprit qui préside à nos travaux. La reconnaissance. Que nous avons, les uns à l'égard des autres quand même, même nous ne faisons pas partie. Voilà nous avons pas pris les mêmes engagements partisans, je crois que ça c'est très très précieux et ce qui s'est passé là cette, c'est un coup de canif.

Monsieur le Président. Juste un mot pour Franck Montaugé pour lui dire que comme il le sait, on est aujourd'hui dans un espace réservé au groupe de l'Union centriste et c'est ce qui a conduit à ce que finalement cette proposition de loi qui reprend en grande partie, celle qu'on avait signé tous les deux ne ne soit présenté que que par mois. Moi je voudrais surtout répondre à, à Madame. La ministre. Madame la Ministre. Vous partagez le constat je m'en réjouis. Vous souscrivez à la philosophie, je m'en réjouis toujours mais malheureusement vous n'êtes pas favorable au texte, c'est quand même assez dommage. Et vous proposez c'est un grand classique depuis Clémenceau de créer une commission. Qui examinera le le problème. Autour de 4 points sur lesquels je reviendrai pas en totalité parce que j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais juste dire 2 choses sur ce vos propositions, vous êtes contre la, la commission d'élus que l'on propose. écoutez vous devriez parler avec monsieur Gérald Darmanin parce que j'ai ici un courrier de lui du 24 octobre où il est écrit en toutes lettres qu'il proposera par décret. La commission d'une instance départementale spécifique et quand vous renvoyer donc je l'invite à rencontrer le ministre de l'Intérieur et quand vous renvoyer à la Commission. D'accès. D'accessibilité pardon c'est tout ce qu'on ne veut pas pourquoi la commission d'accessibilité. Elle est composée de 3 maires. Et de 9 représentants de l'administration. Pour représenter la voix des élus à mon avis on peut faire beaucoup mieux. Et puis dernier point que vous oubliez dans votre axe de travail et qui est essentiel c'est un des des de hein. C'est le coeur de ce de ce texte. En tout cas c'est un point important, c'est la nécessité de réviser le schéma, vous n'en parlez pas. Qu'est-ce qu'on fait dans les départements où il faut faire une révision, il y a il y a plus de 70 départements qui en 2022 n'avaient pas entamé la la révision, qu'est-ce qu'on fait, je pense qu'au bout de 5 ans, c'est utile qu'il y a quand même un bilan de Il y a des évolutions en terme de risques, il y a des évolutions risque en terme technologique, un certain nombre de préfets ont engagé cette cette révision d'autres je suis bien placé pour le dire, ne le veulent pas ou ne le peuvent pas, donc c'est important que cette révision, elle soit prévue par le texte

profondément les, les élus locaux et merci à nos collègues Maurer Montaugé d'une part et aux signataires du présent texte, d'autre part. Alors il y a toujours une tentation de préférer voir la règle s'appliquer pour les autres et de considérer que sa collectivité a droit à une exception, c'est assez français. C'est même peut être assez humain. Or il faut sur un sujet aussi sérieux que la sécurité incendie, une règle claire, c'est une exigence républicaine. Mais à cette exigence, il faut répondre en tenant compte des réalités sur lesquelles les règlements actuels se fracasse. C'est le cas dans le département de la Charente-Maritime, que j'ai l'honneur de représenter qui connaît tous les types d'habitats comme d'autres départements des villes denses des lotissements des bourdes et hameaux ou des habitat très diffus. Je salue donc cette proposition de loi ainsi que les amendements proposés, notamment par mon groupe. La concertation entre élu. SDIS et préfet et le meilleur moyen d'atteindre l'optimum entre les exigences de sécurité et la réalité des moyens de nos communes pour partager intelligemment la responsabilité parce que c'est une sacrée responsabilité. Le diagnostic mais aussi le coût c'est le maire qui connaît le mieux sa commune mais c'est le SDIS qui connaît le mieux la réalité du risque et c'est le préfet. Quand on lui en laisse la marge de manoeuvre qui s'est appliquée efficacement la loi et le règlement. Faisons-leur confiance pour travailler ensemble et sortant d'un carcan qui n'a pas convaincu. Ce nouveau cadre est très attendu en Charente-Maritime en Haute Saintonge comme dans le Nice mais aussi au SDIS qui pour calibrer l'achat de ces engins doit savoir ce qu'on attend de lui car les plans d'investissements sont conséquents. J'invite donc le Sénat a adopté le texte, quelles que soient les amendements retenus et au gouvernement à s'en saisir, il faut écouter le bon sens de la Haute assemblée Madame la Ministre ne réinventer pas l'eau tiède, c'est tout court, dont il est question et le Sénat vous amène une solution clé en main. Je vous remercie. Nous passons à l'amendement huit monsieur Montaugé. Que la question, ça a été évoqué par. De multiples reprises par les orateurs la la question de fond reste quand même celle des moyens. Des moyens, on a essayé plusieurs fois. Un projet de loi de finances. des des des des crédits. À l'effet. De, de mise en conformité des réseaux de de de essayer on n'y est jamais parvenu. Ça n'a jamais été retenu par le gouvernement et moi je suis inquiet d'une chose qui a peut-être pas été évoquée, c'est l'état des lieux des réseaux de défense extérieure contre l'incendie. Au plan communal au plan départemental au plan national, on n'a pas réussi dans le quart de, du travail avec Hervé, on n'a pas réussi à avoir une une vision précise cet état des lieux de conformité la conformité par rapport à ce qui existe, elle est très très préoccupante, je vous le dis et elle met en question la responsabilité juridique des mères en tout cas de ceux qui sont en charge en responsabilité de cette compétence-là, ça reste un problème je je vous renvoie à la question des ponts qu'on a su traiter qui est engagée. Oui voilà ça se pose dans les mêmes termes et peut être avec plus d'acuité encore concernant la DSI

La commission des lois du Sénat a aussi donner une valeur législative o Ernest au au règlement national. Le texte de la PPL, elle ne met pas suffisamment en évidence le lien fonctionnel entre le règlement national et les règlements départementaux donc l'objet de cet amendement c'est de confirmer hein suppression.

Je comprends l'intention que vous avez. Chers collègues. Et je tiens à remercier l'auteur de l'amendement pour sa vision sur le texte établi par la commission que votre intention. Que l'intention de la commission dans la rédaction était beaucoup plus modeste. Il s'agissait moins de permettre au règlement départemental de c'est qu'ils ont pris de la conformité aux référentiels national mais de ne pas prévoir l'existence obligatoire de celui-ci dans la loi afin de ne pas rehaussé toutes les dispositions réglementaires relatives à ce dernier dans la loi, c'est-à-dire ne pas remonter le référentiel national au niveau législatif, ce qui aurait des conséquences bien plus importante que celle que vous imaginez mon cher collègue, si nous avions prévu la conformité du règlement départemental. Un document national. Que nous ne définissons pas dans la loi. Cela m'aurait aurait pu pour couvrir le risque de ce qu'on appelle une incompétence négative. Mais je crois que c'est ça, c'est la réponse technique. La vraie question qu'on doit se poser, c'est la valeur du règlement départemental et la valeur du référentiel national. Est-ce que vous avez vu ce que c'est. Mes chers collègues, que le référent national. C'est un guide pour écrire le le règlement départemental. Ça n'est jamais un super règlement national c'est un référentiel, donc c'est un guide des bonnes pratiques et cetera donc je pense qu'il est si tu le lis l'intention je la comprends, je peux même la partager. Je pense que par contre le faire serait. Beaucoup plus dangereux et beaucoup et créer beaucoup plus de conséquences juridiques qu'on ne veulent le faire et donc c'est monsieur le président. Une demande de retrait à défaut un avis défavorable. Merci madame la ministre. Merci monsieur le. Président donc. Même avis que la commission les termes, pour nous, le cas échéant vise la nature même du référentiel national. De de ce des CI qui constitue en fait comme ça a été très bien expliqué un guide méthodologique. Ce point justifie l'avis réservé du gouvernement sur l'article 1er et sur la volonté de conférer. Hausse Acre un caractère réglementaire alors que ce n'est pas sa vocation. Merci cher collègue. Il est maintenu le l'amendement. Il est retiré il est retiré le huit. Donc on passe au IV monsieur Moret. Oui, merci Monsieur le le président comme cela a été souligné notamment par le rapport du gouvernement le règlement national OCI n'a, n'a jamais exigé une couverture uniforme des de de de la couverture du risque, je cite qu'il n'est pas concevable de demander à des communes peu peuplées de disposer d'une couverture identique à celle des communes urbaines. C'est pourtant ce qui se passe dans un certain nombre de départements dont celui dont je que je représente ici même l'objet de de cet amendement. Et de préciser que lorsque l'on élabore un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. On prend en compte les spécificités départemental mais aussi les spécificités infra-départementale et les spécificités des risques de chaque territoire quand on est en bordure d'une forêt, forcément il faut par exemple plus de de protection que quand on est dans un cas différent, donc c'est vraiment pour qu'il y ait des des règlements qui soit adapté à la situation de chaque territoire composant le département et pas seulement au département dans son ensemble. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cet amendement prévoit que le volet. OCI du Dacr soient désormais tenus d'adapter les règles et les dispositifs. Et ainsi que les procédures du dossier au niveau infra-départementale. C'est une bonne idée. C'est une intention que je partage chaque territoire devant voir les règles s'appliquant à lui-différencier autant que faire se peut et se voir appliquer le principe de différenciation que nous essayons de d'infuser. Au Sénat, sur bien des dispositifs législatifs. Dans notre pays. Toutefois il me semble que seule une vraie appropriation par les acteurs locaux de ces documents permettra aussi de faire vivre effectivement cette différenciation. Ça permettra cet amendement d'Hervé Maurey, de mieux prendre en compte notamment la question de la ruralité et dans la ruralité, la question de la densité de la population des. Des spécificités en terme d'urbanisme. C'est pourquoi la commission des lois ce matin a rendu un avis favorable à l'amendement monsieur Moret. Merci ma main Ministre. Donc le monsieur le président. Merci le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Le gouvernement partage pleinement la préoccupation du sénateur Maurey sur la nécessaire prise en compte dans la définition des règlements départementaux de céder ECI de la grande diversité des situations qu'il s'agisse du niveau de risque à défendre ou de la densité de l'habitat. Toutefois, au fond, le gouvernement rappelle son avis réservé sur cet article 1er qui conduirait à conférer hausse un caractère réglementaire alors que ce n'est pas sa vocation. Merci ma ma Ministre Monsieur Lemoine. Merci beaucoup monsieur le le président. Oui dans la philosophie, c'est vrai que c'est utile et intéressant de pouvoir avoir cette appréciation qui colle au plus près des terrains du terrain. Je veux le le signaler parce que j'ai en tête. Chacun a en tête des cas particuliers. La situation de la commune de de Saint-Martin Ardon dans le département de l'Yonne à qui on refuse effectivement un certain nombre de de DP pour l'implantation de panneaux photovoltaïques. Parce que le point d'eau qui est bien à moins de 100 mètres pour le coup un débit légèrement inférieure aux 30 m3 bon qui est une règle effectivement, fixé dans le règlement départemental, pour autant il y a pas que les bornes. Physiquement, situé à proximité qui peuvent permettre de venir. Comment dire éteindre telle ou telle incendie il y a aussi les moyens prépositionnés dans certain nombre de centres de secours qui parfois sont à proximité. Il se trouve que cette commune et près d'une autoroute près de 2 sites Seveso et cetera et donc nous avons aussi hé bien là très vite peut se rendent sur place et donc je pense que l'appréciation fine comme ça hé bien également des moyens et donc ça on peut le faire à travers cette vision infra-départementale. Hé bien, ne peut qu'aider à avoir. Hé bien une analyse juste. Et permettant de concilier la sécurité et puis également le développement de ces territoires. C'est un point que je voulais signaler à l'occasion de cet amendement qui du coup me semble assez. Comment dire frappée au coin du bon sens. Merci cher collègue dont je le mais voit cet amendement quatre avec un avis favorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté le trois monsieur Moret. Oui, merci Monsieur le Président, j'ai évoqué tout à l'heure le le fait que dans certains cas, il y avait des coups littéralement insoutenable pour les communes en matière de d'application des des règles qui leur sont imposées donc cet amendement vise à a préciser que le règlement départemental doit à l'avenir prendre en compte les moyens financiers des communes et des établissements de coopération intercommunale lorsqu'ils sont Donc c'est pour s'assurer que l'on aura plus demain des règlements qui impose aux communes des charges tout juste tout tout simplement insoutenable pour elle. Oui, monsieur le président. Le le présent amendement tend à prévoir que le volet dit aussi du Dacr prend en compte les moyens financiers des communes et le cas échéant des EPCI compétents. Je comprends l'intention de l'auteur, mais j'ai une nuance sur ce sujet-là, pas sur les autres mais dans celui-là qui est importante et que je voudrais expliquer qui qui justifie un avis défavorable de la commission cet amendement. Mes chers collègues, est satisfait. Dans son intention par l'amendement que j'ai proposé, qui a été adopté par la commission. Des lois. L'amendement adopté donc dans le texte, déjà la Commission prévoit que le vol été aussi dû s'Dacr favorise je cite un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et lorsqu'ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l'incendie et par le Service d'incendie et de secours. Nous avons non déjà prévu la, dans dans la. Le texte de la commission, la nécessité d'un équilibre avec une disposition quantitative et une complémentarité c'est la disposition qualitative entre les moyens du SDIS et les moyens déployés par les communes. C'est important que nous ayons cet équilibre-là et. Si nous allons sur des termes aussi aussi précis que ce que propose Hervé Maurey, alors à ce moment-là, nous aurons nous aurions besoin aussi de mettre d'autres termes, je parle notamment au moyen aux questions des moyens techniques. Des des services départementaux d'incendie et de secours de retrouver un nouvel équilibre, il faut qu'on nous soyons sur une loi. Précise et si possible. La moins. Qui utilise le moins possible de périphrases et de rester sur un dispositif qui soit juridiquement. A fortiori mon, mon cher mon cher collègue Hervé Maurey si nous visons un une adoption par l'Assemblée nationale, et peut-être d'une adoption conforme puisque moi je porte cette ambition Madame la Ministre que cette ce texte soit voté par l'Assemblée nationale à ce moment-là, je pense qu'il faut que nous restions à l'adoption à l'adoption du texte adopté par la commission des lois si Madame Laberge retrait ou défavorables. Je m'en remets à la sagesse de la commission des lois sur cet amendement. Merci. Il est maintenu ou retiré parce que Monsieur Maurel est maintenu ou retiré. Écoutez, je vais, je vais le retirer et puis pour faire confiance. Au rapporteur puisqu'il m'a dit que ma préoccupation a été prise en compte dans la rédaction de la commission des lois. J'estime que que l'amendement est satisfait donc je le retire.

Et territoires ruraux m'est apparu important de préciser que le volet relatif à la défense extérieure. L'incendie du schéma d'analyse et de couverture est élaboré avec les maires et avec les maires ruraux notamment, je vous remercie. Monsieur le président. Il va sans dire que dans cette assemblée, nous chérissons la ruralité et les maires qui sont les élus des communes rurales. Prévoir la prise en compte particulière des communes rurales. Les maires des communes rurales sont d'ores et déjà inclus dans la mention la proposition de loi telle que nous l'avons re-réécrite et dans un département rural Les maires ruraux sont ultra-majoritaire, y compris dans les instances de concertation que nous avons prévu. Je ne crois pas utile de préciser. Encore plus cette. Cette notion, donc c'est un avis défavorable de la commission des lois. Monsieur Blanc il est maintenu. Pardon, pardon. L'avis du ministre. C'est rien j'arrive. Merci monsieur le président. Le gouvernement s'en remet à l'avis du rapporteur de la commission des lois sur cet amendement. Très bien. Monsieur Blanc. Monsieur le président je je vais le maintenir, parce qu'il y a des départements où les maires ruraux ne sont pas spécialement. Représentés. Et. Espèrent être associés à ce type de décision.

Qui est contre.

d'accord bon alors comme il y avait un équilibre quand même entre les pour et les contre. C'est pour ça que j'espérais un peu sur les abstentions. Recommence lever vraiment nettement la main qui est pour. Là c'est plus net. Ah ben voilà. Regardez. Et ben voilà il fallait le dire bon elle est très bien il est adopté. Le neuf. Monsieur

Du conseil d'administration du du Cassis. Et cet avis conforme du du Cassis de devant lui-même tenir compte des avis du conseil départemental des conseils municipaux des communes compétentes et le cas échéant des organes délibérants des EPCI qui sont situés sur le territoire du du du département. Donc en fait il s'agit notamment à partir des des constats que nous servions fait dans le le rapport avec Hervé Maurey. Précité. Il s'agit de de tirer les conséquences des défauts constatés par le passé à la suite de l'adoption des règlements départementaux de de Et Les REDD si donc des communes ont été confrontés. Ça, ça a été dit à de multiples reprises. Hein hein. Discussion générale a des conséquences. Budgétaires très lourdes qui excède largement leur capacité financière et qui obère leur marge, marge de manoeuvre sur d'autres projets communaux qui sont attendus par la population. ce dispositif permettrait quand même avec cette exigence de conformité de faire les choses comme il faut. Antonin compte des possibilités des communes. Des territoires plus plus largement. Merci avis la commission monsieur le rapporteur. Monsieur le président. Je comprends l'intention de monsieur Montaugé. Je suis défavorable à cet amendement viendra ajouter une condition qui n'existe pas à l'heure actuelle pour le règlement départemental. De défense contre l'incendie, puisqu'il est aujourd'hui adopté après un avis simple du Ducasse 10 l'ajout d'une telle disposition nuirait à la cohérence de notre position qui tend justement à mieux inclure les élus

Pas toujours. Le défenseur du du pouvoir préfectoral mais en l'espèce, je pense que c'est quand même une responsabilité qui est importante et je pense que la vie simple est préférable à l'avis conforme donc demande de retrait ou avis défavorable. Avis du gouvernement, d'un ministre. Merci monsieur le président. Le gouvernement souhaite aussi le retrait de cet amendement. En effet. Si l'association des représentants des collectivités territoriales dans la définition de la stratégie. De décide cette défense doit être amélioré, cela passe avant tout par son inscription dans la durée au travers notamment d'une instance départementale de suivi et ne décide pas d'assortir les avis recueillis d'un caractère conforme. Je rappelle enfin l'avis réservé du gouvernement sur une partie de la substance même de cet article 1 qui conduirait à conférer hausse d'Acre un caractère opposable alors que ce n'est pas sa vocation, je vous remercie. merci monsieur le président. Les l'intention de se, de, de cet amendement est aussi d'attirer. L'attention pour le coup. Sur sur la dimension financière de cette affaire. on demande aux collectivités d'engager des investissements par rapport à la défense extérieure contre samedi. À un moment donné il faut que l'ensemble des responsables ou des parties prenantes prennent leurs responsabilités sur le sujet. Voilà pour que, au bout du compte. Et au regard des règlements. On est des réseaux qui soit conforme à ses règlements et qui surtout permettent de défendre nos qu'ont nos concitoyens nos compatriotes quand contre le risque incendie. C'est ça la difficulté dans laquelle on est en réalité. c'est ce que pose le le texte, c'est aussi l'ambition du texte et cette cette exigence de conformité où cette demande de conformité d'avis conforme. Aurait permis une plus grande responsabilité. Responsabilisation des acteurs pour aller dans ce sens-là. Voilà, ce texte ne va pas résoudre le problème de fond. Je regrette. Voilà on aura légiférer une fois de plus on sera toujours à côté du du du sujet par rapport à la question des moyens et de langage demande des moyens au regard de chars que partie prenante qui voilà et responsable du parti du sujet à la place qui est la sienne et conformément aux responsabilités qui lui sont comme Ferré. Merci. Pas de demande d'explication de vote je mais aux voix l'amendement 9 avec 2 avis défavorable qui est pour.

Excusez-moi monsieur le président. Cet amendement propose. La possibilité de transférer la aussi la police spéciale

cette faculté, peut être mise en oeuvre dans une perspective de rationalisation de mutualisation et de plus grande efficience de la de la défense extérieure contre l'incendie je pense qu'il faut, il faut vraiment le permettre. Il y a pas de contrainte il y a pas d'obligation encore une fois unanimité pour arriver à à à cela. Voilà je ça irait dans le bon sens. Il me semble. Monsieur manteaux ai le 17 en discussion commune c'est le vôtre.

merci Monsieur le le président et chers collègues, il s'agit là de, de, de permettre d'autoriser le transfert de la police spéciale de des Dessy vers les syndicats compétents. le but étant de de d'améliorer en fait l'articulation de la DSI entre communes et groupements. De la sorte. Voilà. Merci avait de la commission sur ces deux amendements en discussion commune. Monsieur le Président, sur l'article l'amendement cette de Monsieur Montaugé. C'est une demande de retrait car il nous apparaît. Que cet amendement est parfaitement satisfait par le droit existant, notamment. Depuis l'adoption par le parlement de la loi 3DS. En effet, l'article 52. Tiret 61 du CGCT dispose qu'en matière de défense et cetera contre l'incendie à l'État les ont publics de coopération intercommunale à fiscalité propre on établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte surtout tout partie de son territoire ou à plusieurs syndicats située chacun sur des parties distinctes de son territoire. Donc ça me paraît parfaitement satisfaits. Quant à votre amendement monsieur Montaugé. L'amendement 10. C'est un moment qui tend à prévoir que le président d'un syndicat des eaux pourrait exercer un pouvoir de police en matière de défense et ça compte l'incendie lorsqu'il exerce la conférence que la compétence. C'est une bonne idée. Cette disposition à laquelle le rapport de la direction générale est d'ailleurs favorable me semble tout à fait de bon aloi. Elle permettra une meilleure efficacité de l'action publique en la matière. C'est un avis favorable. Avis du gouvernement. Hein défavorable aux deux amendements.

Merci monsieur le président. Non, madame la ministre, on aurait quand même aimé avoir quelques explications par rapport à la position. Que vous vous exprimez au nom du du gouvernement mais bon ça ça viendra peut-être. Monsieur le président. Sur sur le premier amendement à l'écoute des des propos du du du rapporteur j'ai j'entends effectivement que la droit des la loi 3DS intègre ça il y a une petite notion dans cet amendement qui figure pas dans la loi 3DS c'est l'unanimité.

on votera pour le neuf. Au nom de mon groupe mais. Voilà on aime. Quelques explications de Madame la Ministre je vous remercie d'avance Madame. Monsieur manteaux j'ai, soyons clairs, le sept, vous le maintenez ou vous le retirer au profit des explications du rapporteur le cet homme a le. Le retirer.

Alors. En fait, cet amendement vise à créer. J'ai reprendre une partie des éléments cités par le rapporteur de la commission, cet amendement vise à créer et je parle bien du 10. Une nouvelle possibilité, transfert de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie au président d'un groupement de collectivités territoriales, compétents en matière d'eau actuellement la police spéciale de la dissiper transféré facultative ment aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de d'ici ce présent amendement a pour objet d'étendre la possibilité de ce transfert au Président des groupements compétents en matière d'eau, un tel transfert devrait nécessairement. Conditionné par le fait que le groupement dispose de la compétence en matière de service public de Dessy, laquelle est distincte du service public de l'eau en effet l'amendement proposé risquerait de permettre la séparation entre l'exercice de la compétence et celui de la police spéciale. Par conséquent, je vous confirme que le gouvernement est défavorable à cet amendement. Oui voilà. Parfaite information de madame la ministre et des, des collègues. Cet amendement a été rectifiée. Dans l'intervalle, donc il il prend en compte toutes vos observations. Absolument, à la police rectifié. Alors je vous fais confiance. Monsieur le rapporteur de la commission, monsieur le sénateur, parce que je n'ai pas la la bonne version probablement et donc je m'en remets

Qui est contre. Il est adopté. Nous passons à l'article de avec une demande de parole de monsieur Seguin. Merci, monsieur le Président Madame le Ministre. Il existe aujourd'hui un impératif légal pour les communes, on vient de le répéter, d'avoir des réserves d'eau de minimum 30 m3. Pour répondre aux risques faibles isoler leurs distances oscillant de 200 à 400 mètres des habitations dans mon département de l'Orne. Ce sont, ah tiens des communes qui ne sont pas aux normes. Comme de nombreuses communes rurales partout en France. Une solution pourrait être mise en place pour compenser ses manques qui représentent des dangers notamment pour les sapeurs-pompiers, la fourniture de camions citernes de grande capacité de 10 à 15 m3 ce que les préfets n'osent pas mettre en place, n'ayant pas de cadre législatif ou réglementaire qui leur permet explicitement. Ces camions viendrait en complément des réserves d'eau des communes seraient en nombre suffisant pour quadriller le département et ne ferait pas l'objet d'un transfert de responsabilités. Il conviendrait par là d'élargir les moyens pour parvenir aux objectifs opérationnels de la DSI ainsi le recours au camions citernes de grande capacité doit être précisé clairement dans le référentiel national prévu au R 2225. De du CGCT qui a été introduit par le décret du 27 février 2015 relatifs à la défense extérieure contre l'incendie. L'ouverture de ce dispositif serait une décision simple et efficace, attendu par les acteurs de terrain, il n'appartient qu'à vous Madame la Ministre par voie réglementaire de le faire. Et pour votre information si vous souhaitiez exprimant expérimenter cette mesure. Sachez que le département de l'Orne se porte volontaire. Je vous en remercie.

à ce que le rapport annuel qui sera rendu par la commission départementale chargée du suivi de la défense extérieure contre l'incendie soit adressé aux parlementaires du département. Monsieur le président. Chers collègues, c'est un avis défavorable pour une simple raison, c'est que cette commission. Nous sommes en train de la créer que nous laissons une liberté, la plus grande possible d'organiser leurs travaux, que l'idée d'un d'une transmission de ce rapport parlementaire est une bonne idée pour autant en faire une obligation législative. Je suis pas sûr que ça contraignent ce soit une idée qui soit une idée de contraindre. Moi je préférerais que étant donné que ce sont des élus locaux qu'ne sont pas membres du du conseil administration du SDIS. On va peut être une fou pour une fois leur faire totalement confiance dans la manière d'organiser leurs travaux et la publicité qu'ils vont donner à ceci, c'est la raison pour laquelle mon cher collègue, c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement. Merci monsieur le président je propose très brièvement de répondre au sénateur Maurey en introduction de cet article de pour vous rappeler, et peut être clarifié ce que je vous propose, ce que je vous ai proposé, la problématique de la DSI soit évoquée au sein d'une instance départementale qui existe déjà. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui est présidé par le préfet, cette commission traitait déjà de sujets liés au risque incendie associent les acteurs locaux dont les maires et donc ce que je vous ai proposé c'est de créer au sein de cette ces CDS DSA une formation spécialisée. Une sorte de sous-commission. Sur la DSI qui pourraient remplir les mêmes missions que celle envisagée par votre proposition de loi. Donc je pensais nécessaire de clarifier peut être mes propos ensuite mon plan d'action, c'était de vous proposer que cette extension des compétences de la ces CDS a institué par un décret du 8 mars puisse s'effectuer par voie réglementaire. Je pense que vous l'aviez compris associe l'ensemble des acteurs territoriaux de la DSI et demeure placé sous la présidence du préfet en effet ce dernier tu à l'échelon départemental, détenteur de la compétence de police générale au titre de laquelle il arrête le règlement départemental de ici dont l'instance de concertation a créé aurait pour but d'assurer le suivi Pour ce qui est en est de l'amendement numéro 5. Nous nous en remettons à l'avis de la commission avis défavorable. Monsieur Moret.

à laquelle vous proposez de donner la compétence que le, que l'on donne à cette commission concret conformément à ce que souhaite le ministre de l'Intérieur. Encore une fois cette commission, elle ne nous convient pas pour la simple et bonne raison qu'elle est composée je me répète deux 3 élus et de 9 fonctionnaires. Je suis tout à fait respectueux des fonctionnaires mais je ne pense pas que nos fonctionnaires et 3 élus se soit de nature à représenter. La volonté des des des communes et notamment des communes rurales comme la, comme l'a dit notre excellent collègue sur mon amendement qui propose simplement encore une fois que l'on transmette. Le rapport de cette commission aux parlementaires, je le maintiens et je le maintiens. Pour une raison très simple, on est tous à se plaindre dans cette assemblée, matin, midi et soir, qu'aujourd'hui, notamment du fait de la suppression du cumul des mandats, on est plus au courant de rien on sait plus ce qui se passe dans les commissions dans les différentes réunions qui se tiennent. Là il s'agit d'assurer le le suivi de de d'un d'un règlement qui a une implication sur l'ensemble des le tout en application d'une d'un texte qu'on est en train de voter, donc ça me paraît important que l'on écrive noir sur blanc que ce rapport devra nous être transmis qu'on soit pas obligé d'aller lever le doigt et et mendier supplier pour avoir communication de ce rapport. Monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président. Hein. Une réponse. Hervé Maurey, ça pourrait faire l'objet d'une autre PPL, l'association des parlementaires, dans les départements depuis la fin du cumul des mandats. On ne, on ne le dit jamais assez. Les parlementaires même au type de leur pouvoir de contrôle de la Constitution ont énormément de difficultés. Madame la ministre, à être au courant de ce qui se passe. Le problème c'est que si on commence à mettre dans tous les textes que tous les documents qui sont élaborés par toutes les commissions départementales doivent être transmis aux parlementaires à ce moment-là on alourdit le droit et a fortiori au moment où nous vous proposons ensemble monsieur Moret et la commission des lois de créer une commission d'élus locaux qui est pas du tout votre idée Madame la ministre hein, c'est vraiment une commission à part indépendante qui va vraiment éclairés les les la la les travaux du d'illustration du SDIS du préfet. À ce moment-là. Laissons un peu de liberté, nous qui sommes qui chérit sont à la fois la décentralisation mais aussi la liberté locaux pour ne pas rajouter ça dans le texte. Ma foi, si le Sénat le votent, c'est c'est c'est pas c'est pas la plus grande difficulté mais c'est vraiment un élément qu'on doit avoir pour. Pour la suite de nos travaux parce que si si on met ce mot, ce mot là dans tout ça, on risque d'alourdir vraiment le droit. Je vous en prie, allez-y. Merci le monsieur le Président, je pense que j'avais une collègue qui avait levé le doigt avant mais on lui donnera la parole, la parole après. Non, simplement pour souscrire à l'argumentation du du rapporteur. On va pas. Utilisées ou instrumentalisées, un texte qui vise à, à renforcer les, les élus locaux et leur capacité de faire. En essayant de corriger le besoin de d'information des. Des parlementaires. Alors je comprends tout à fait l'intention, mais je pense que c'est un autre sujet. Et nous on on souscrit à l'argumentaire de du du rapporteur. Madame brûle Merci, monsieur le Président, j'entends les arguments du rapporteur mais peut-être Madame la Ministre que le signe que vous devriez donner. Dès à présent. C'est de vous engager à fournir le rapport que le gouvernement de par la loi 3DS. Devait porter à la connaissance du Parlement sur cette question de défense incendie. Et qui ne l'a pas été. Parce que. On n'a pas un plaisir particulier à lire des rapports je crois les uns et les autres. Mais on voit bien que c'est un sujet qui préoccupe de nombreux départements qui préoccupe encore plus de nombreuses communes qui tente. De se mettre en conformité avec les exigences de la défense incendie et qui n'y parviennent pas. Malgré toutes les volontés du monde. Et je soupçonne. Et je le dis volontairement sans l'avoir lu puisqu'il ne nous a pas été remis. Je soupçonne que ce rapport conforte ce que nous disons, les uns et les autres et qu'ils. Qu'ils fournissent. Comme l'avait déjà fait le rapport de nos collègues Montaugé Maurer des pistes. Qui permettent non seulement de contrôler le gouvernement mais d'améliorer cette affaire parce que je me j'ai en tête. Que le rapport de nos collègues disait qu'il y avait encore ça c'est sûrement amélioré depuis. Mais il y avait encore 7 millions de nos concitoyens qui n'étaient pas couverts. Par la défense incendie en raison de l'impossibilité des communes de répondre aux exigences. Et donc c'est un vrai sujet et donc Madame la Ministre, nous souhaitons que ce rapport ne soit remise vous en remercie d'avance. Madame la ministre. Madame la ministre, vous avez tort de soupçonner madame la sénatrice. Le rapport a été transmis à la commission des Lois il sera transmis à tous les parlementaires bien sûr.

tous les groupes sont partagés, là c'est assez curieux. Alors on recommence. Qui est pour lever nettement à la main.

Merci. Qui est contre. Il est rejeté. Allez le 13 Madame de Marco. Merci j'ai précédemment évoqué des inquiétudes quant aux conséquences de cette proposition de loi sur les normes d'installation des points d'où incendie dans les communes. C'est précisément le cas du remplacement des règlements départementaux par le vol et incendie dans les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques. Mais aussi de la rédaction d'évaluation préalable des conséquences financières, rumeurs mystique et de développement économiques visant à permet des dérogations pour les communes les moins exposés aux incendies. Dans les prochaines années, sous l'effet du réchauffement climatique en cours, de la multiplication des sécheresses et de la raréfaction des ressources anneaux le risque incendie va croître sur l'ensemble de notre territoire afin de s'y préparer, il convient que des études préalables sur l'installation des bouches d'incendie communal intègre ces perspectives climatiques telles telles le sens de cet amendement. de défense et cetera contre l'incendie est éteint un des endroits où on a pu relever ça l'avis de la commission que nous avons rendu ce matin est un avis de sagesse sur cet amendement Madame de Marco. Merci. Il y avait du gouvernement qui aimait aussi un avis de sagesse. je mets aux voix l'amendement très avec 2 avis de sagesse qui est pour. Ce qui est contre. Adoptée. Le 12 Madame de Marco. Cet amendement durement vise à compléter la proposition de loi d'une des recommandations du rapport d'information. 18 juillet 2021 consacré à la défense extérieure contre l'incendie. Je lis page 46. La proposition de recensement de l'ensemble des points d'eau je cite ici les rapporteurs la DEC, il repose sur une équation à plusieurs variables à pondérer parmi lesquels la disponibilité de ressources en eau, le débit de cette ressource et la distance entre celle-ci et la zone à défendre l'enjeu consiste à trouver le point d'équilibre entre ces différentes contraintes a optimiser la combinaison de ces variables. Dès lors, l'un des leviers sur lequel il apparaît judicieux de jouer réside dans la prise en compte de l'ensemble de la ressource en eau en effet optimiser cette ressource permet d'alléger les exigences sur les autres variables en particulier la distance. Fin de citation. Telle est l'objet de cet amendement qui permet de remplacer les obligations communales de création de bouche d'incendie par la meilleure prise en considération de l'ensemble des ressources nous y compris privés déjà présente sur le territoire. Merci. Avis de la commission. Non monsieur le président. La visite de la commission est défavorable. On va, on va laisser peut-être les commissions départementales et les et les élus et les techniciens départ. Manteau avec un peu de liberté sur la capacité qu'ils ont à à identifier les points d'eau, on va pas on va pas lister ici les lacs, les mares les étangs, les cours d'eau et je veux dire, on retrouve on tomberait dans une rédaction quasiment du code civil, dit à plus de 200 ans. Donc soyons dans quelque chose de de large ne ne ne ne ne mettons pas ce genre de disposition dans dans dans la loi de grâce. Je comprends l'esprit. Il a dit il a du sens, mais il est beaucoup trop précis. Pour être repris. Dans le texte de loi. Madame la Ministre. Nous comprenons aussi l'esprit mais nous émettons un avis défavorable aussi. Hé bien je mise aux voix l'amendement 12 avec 2 avis à monsieur Richard. pour pour faire sourire à l'heure tardive. Est-ce que les piscines privatives doivent être pleine d'eau ou est-ce qu'elles peuvent être vide.

Merci, monsieur le Président Madame la Ministre sur le rapporteur monsieur l'auteur dans le même ordre d'esprit que précédemment. C'est un amendement. Qui précise qu'il propose de préciser que les membres de la commission départementale de suivi soit désigné sur proposition des associations des maires du département. Dont l'Association des maires ruraux. Merci commission. Oui, monsieur le président tout à l'heure, le Sénat a adopté. Un joli notamment dont la commission des lois strictement horreur. On est un peu dans le même esprit, mon cher collègue sur cet amendement, premièrement, il n'y a pas d'association des maires ruraux, dans tous les départements. Deuxièmement si nous créer nous mettons l'association départementale des maires ruraux au même niveau que l'association départementale des maires. Alors nous aurons des demandes. Des communes forestières des des petites villes, de villes moyennes des intercommunalités et de toutes les associations d'élus qui serait légitime a demandé à être autour de la table donc dans un département rural, je reprends le même argument que tout à l'heure où les maires ruraux sont très majoritaires, ils sont aussi très majoritaire de l'association départementale des maires qui sont fédérées au sein de l'association des maires de France et c'est la raison pour laquelle la maître-ces 2 associations mais au même niveau ne nous est pas apparu comme quelque chose de père pertinent sauf encore une fois à élargir complètement à toutes les associations d'élus, de tous ceux qui voudraient. Donner un, un avis en la matière donc l'avis de la commission des lois et défavorable sur cet amendement même si on comprend encore une fois la nécessité de bien représenter les maires ruraux à la hauteur de la la représentativité qu'il mérite. Madame la Ministre. qui ne réunirait pas l'ensemble des acteurs territoriaux de la défense extérieure contre l'incendie. Merci Monsieur Blanc. Merci, monsieur le Président, je persiste dans mon désaccord mais il se trouve que j'ai été saisi de très nombreux cas où des règlements départementaux dont nous parlons, n'ont pas été soumis à la consultation des maires ruraux, alors comment ça fonctionne, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Il y a les nombreux endroits où ça ne fonctionne pas donc il me paraît important de le faire figurer dans la loi. Que les élus ruraux sont représentés. Je ne vois pas où est le problème. Merci Monsieur Lemoine. Merci président. En lisant attentivement donc le le le 5ème alinéa de cet article. Il est bien dit que ce serait sur proposition des associations des maires du département. Il me semble que quand on parle des associations. Ça ne couvre pas qu'une et qu'il peut y avoir au sein des départements effectivement parfois plusieurs associations l'AMF d'un côté la AMRF de l'autre et donc finalement je me demande si le texte tel qu'il est rédigé. au bénéfice des débats qu'on peut avoir là présentement ne peut pas englober aussi en fait d'autres types d'associations de maires qui peuvent être parfois plus sectorielles en tous les cas la rédaction. Ne me semble pas l'exclure. Merci monsieur le président. Il y a des. Départements de divers. Genre il y a le département urbain. Il y a un département rural. Il y a le département. Dual. C'est le cas par exemple du département d'où je viens. C'est un département qui est à la fois urbain. Et à la fois rural et l'expérience a montré sur la base de ce que propose systématiquement notre préfet. d'inviter les 2 associations de maires qui ont toutes les deux à caractère général qui ne sont pas des associations thématiques. C'est pas la forêt. les les cours d'eau c'est 2 associations qui ont une compétence générale mais qui se distingue par la taille des communes qu'elle représente et force est de reconnaître que c'est un vrai sujet et donc. Moi j'invite en tout cas je voterai l'amendement proposé par notre collègue blanc parce que il va dans le bon sens, il est respectueux de la diversité des situations que connaissent nos communes. Merci monsieur le président et moi dans mon département, il y a il y a effectivement une association des maires ruraux, une association des et bé pendant de l'Association des maires de France. Et le président de l'association départementale des maires de France siège. L'Association des maires ruraux est le président de l'association des maires. Siège à l'Association des maires de France dans le département du Doubs. Donc il serait incompréhensible que effectivement. L'un puis siéger et et pas l'autre. Donc je pense l'argument effectivement développé sur le fait qu'il y a peut être pas dans tous les départements. Des associations de maires ruraux peut s'entendre. Mais c'est pas parce qu'il y a quelques départements. Qui où il n'y a pas d'associations de maires ruraux qu'il ne faut pas les entendaient moi je voterai. L'amendement de monsieur Blanc.

Alors les communes forestières dont nous sommes un certain nombre à être membre ici pourraient tout à fait légitime à vouloir être membre de cette commission sur qui traite des questions de défense et va contre l'incendie il y aurait rien, il y aurait rien de d'illogique donc habituellement habituellement au Sénat on on reconnaît la juridiction de l'Association des maires de France et de leurs déclinaisons départementales que sont les associations départementales, soit on ouvre complètement comme l'a dit Jean-Baptiste Lemoyne à tout un tas d'associations qui sont effectivement des associations générales comme l'Association départementale des maires ou l'association départementale des maires ruraux mais qui peuvent être tout un tas d'autres associations qui pourraient là ou ailleurs, avoir une légitimité à à agir donc je c'est un débat qu'on a eu d'ailleurs la commission des lois, je m'en souviens, je m'en souviens très bien encore récemment, je préférerais qu'on en reste à une une acception la assez restrictive qui est celle de l'association départementale des maires qui couvre le plus la le la plupart des communes de notre département la pardon mais c'est pas une hostilité vis-à-vis des maires ruraux. Mais si on ouvre la porte,

que vous y alliez par voie de circulaire. Prendre des dispositifs. Oui, tout à l'heure. Oui, enfin que vous alliez prendre des mesures réglementaires qui correspondrait peu ou prou et qui pourrait remplacer la proposition car vous étiez David avoir des mesures réglementaires. Je pense que dans ces dispositifs inciter à consulter l'ensemble l'ensemble des associations présentes dans chacun des départements parce que chacun de nos départements ont des structures différentes, et peuvent avoir plusieurs démembrement de différentes donc ça ça peut être déjà une instruction qui peut être donné. À vos services dans les départements et qui devrait permettre de de régler ce problème. Merci.

Il est rejeté. Je mais voit l'article 2. Qui est pour. Qui est contre. Il est adopté après l'article de un amendement six Monsieur Oui, merci beaucoup monsieur le président. Bien cet amendement vise à ce que soit prévue dans l'année qui suit la promulgation de la loi, une révision de l'ensemble des schémas qui n'aurait pas été. Révisée depuis leur élaboration c'est-à-dire au au cours des 5 dernières années, on l'a évoqué dans dans nos débats cet après-midi il y a encore beaucoup de de département où les règlements n'ont pas été mises à jour. Or, ça nous semble utile de faire un bilan de de ces règlements, et d'autant plus qu'il y a des situations qui ne peuvent pas perdurer comme on a eu l'occasion de de l'évoquer, donc voilà c'est simplement prévoir cette cette révision de l'ensemble des schémas qui n'ont pas encore été. Avis

la la loi était promulguée. Nécessité de prévoir ce type de dispositif donc c'est c'est tout à fait bienvenue. Je je ne ne serait pas plus long puisque je reprendrai pas la parole pour explication de vote. Monsieur le Président, je voulais simplement dire, Madame la Ministre que si nous divergeons sur. La manière dont vous voulez le faire par le règlement et nous par la loi. On doit saisir au bond votre votre proposition. De travailler sur les 4 thématiques. Vous avez évoqué dans votre discours, je vous demanderai s'il vous plaît de prendre en compte les différentes. Éléments de la discussion générale d'un certain nombre de nos collègues, je pense notamment. À Nathalie Goulet je pense notamment à l'intervention de Vincent Segouin tout à l'heure sur la des l'adéquation des moyens matériels dans les départements. Je crois que c'est vraiment des éléments de réflexion qui sont importants, on pourrait éviter et faire des économies énormes, si nous avions simplement une adaptation de la norme en matière, en matière de de de matériel, notamment des matériels roulants. Tout à fait adapté désormais donc vraiment, on est d'accord pour travailler avec vous. Mais mais prenait en compte un certain nombre d'observation que les collègues ont fait dans la discussion générale. monsieur le rapporteur. Madame la Ministre votre avis sur l'amendement six. Sur l'amendement si je m'en remets à la vie de sagesse de la commission et je réponds à monsieur le rapporteur, que je suis ravi que vous acceptiez de travailler avec nous. Je voulais proposer et on va travailler ensemble, en prenant en compte les propositions intéressantes qui ont été faites par. les différents sénateur, merci beaucoup. Qui est contre. Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, y a-t-il des demandes d'explications de vote. Oui monsieur Montaugé Madame Goulet, allez-y.

y a quiétude. Quant à la difficulté que rencontrent beaucoup de territoires et beaucoup d'élus qui sont responsables directement, personnellement. Dans la mise en conformité de leur réseau de défense extérieure contre l'incendie, les moyens. Ne sont pas. À leur disposition pour pour se faire, je profite de l'occasion pour saluer. Et services d'incendie et de secours qui, malgré cette situation sur laquelle certaines. D'entre nous ont alertés. Font face. Situation de de feu de lutte contre le feu. Voilà je tenais aussi à le à le souligner, il se débrouille toujours, ils arrivent toujours à trouver des solutions pour minimiser les les les les dégâts et évité la plupart du temps les dégâts humains, mais l'inquiétude demeure. je veux attirer. L'attention. Du gouvernement là dessus. Certains préfets accepte que de la DETR soit consacré puisse être consacrée à la mise en conformité de ces réseaux, il faut aller bien au-delà.

de budgétisation et et au niveau national je terminerai sur un point, nous avons avec Françoise Gatel et Hervé Maurey, à l'occasion de notre travail de 2 rapports rencontrer le ministre de l'Intérieur monsieur Darmanin, qui nous a indiqué et il a donné suite à ça. Vouloir faire un audit interne à la direction de la sécurité civile sur ce sujet il y a procédé parce que j'ai été interviewé, moi en tant que en tant que rapporteur, il serait intéressant pour autant que ce soit possible que nous ayons un retour sur ce rapport d'audit interne un relatif à à la DSI sur la note à l'ensemble du territoire national. Du point de vue de la sécurité civile donc nous voterons favorablement ce texte c'est même pas dans le bon sens. Merci. Il en faudra beaucoup d'autres. Merci Madame Goulet. Oui, monsieur le président, ma la même ministre vous dire évidemment qu'on soutenait le texte qui était défendu qu'on soutient que soutiendront aussi vos initiatives. Revenir sur la proposition d'expérimentation qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une demande de vent. Lors de la discussion budgétaire ce dispositif. Était d'ailleurs tellement intéressant que j'avais proposé au rapporteur d'entendre le président du du département. Je ne l'ai parfait lors de cette proposition, mais mon collègue second à la fait donc c'est parfait. C'est un dispositif qui est cher mais je suis sûr que. Il y aura un moyen de, d'y arriver. En attendant, les maires attendent vraiment Madame le Ministre des dispositifs urgent je l'ai dit en commençant la discussion générale c'est un irritant supplémentaires c'est un frein à l'urbanisation dans nos départements et à la construction dont on a impérativement besoin dans les territoires ruraux. Donc vous avez fait des propositions et vraiment on vous attend. Vraiment sur ces sujets. Merci. Madame brûlant. Merci monsieur le président. Je l'ai dit nous allons voter ce cette proposition de loi qui va. Améliorer un certain nombre de choses et je pense que de nombreuses communes vont s'en réjouir. Le sujet ne sera malheureusement pas épuisé et j'entends dans ce qui est dit par les uns et par les autres et y compris par vous Madame la Ministre de la volonté de continuer de nous associer aux améliorations à apporter au titre de celle-là. Je voudrais moi aussi insisté sur le coup qui reste extrêmement important pour les communes, même lorsqu'on trouve des solutions de bon sens et de bonne Intelligence. Et que la DETR ne peut pas être le seul vecteur de financement. Notamment parce que c'est au détriment d'autres projets locaux et que, par définition, les communes qui ont, n'ont pas pu avancer sur la défense incendie ben vont devoir retarder d'autres projets. Je pense que ça mérite d'être examinée. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui attendu c'est. La possibilité de nos données, un genre d'agrément au bureau d'études qui accompagne les communes parce que pour le dire de manière un peu triviale, certains ont la main un peu lourde. Autant dans les études qu'ils fournissent que dans le nombre de points incendie qu'il propose de, de mettre en oeuvre. Et que un agrément ministériel comme ça se fait dans d'autres domaines. Pourrait permettre de juger de la probité ou pas de ces bureaux d'études le mieux. Étant encore et c'est ce que nous avons obtenu en Seine-Maritime. À force de revendications que le SDIS mettent à disposition des personnels pour accompagner mieux les communes dans la définition de leur schéma communal. Il me semble aussi et je crois que c'était une des pistes qui étaient évoquées dans le rapport de nos collègues qu'il faut aussi évaluer et comparer le coût que représenterait pour les SDIS comparé au coût que ça représente pour les communes tout ça et de l'argent public et nous veillons tout ça ce qu'ils soient utilisés le mieux possible, parfois il est préférable d'équiper.

Qui est contre. Qui s'abstient. Elle est adoptée. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 est parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires présenté par Madame, Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues dans la discussion générale. La parole est à madame Françoise Gatel, auteur de la promotion de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois. Madame le rapporteur, mes chers collègues, l'égalité de représentation des femmes et des hommes est un principe constitutionnel depuis 1999. Ainsi pour les communes de plus de 1000 habitants. Le législateur. A instauré une règle de parité pour leur représentation au conseil municipal mais aussi au conseil communautaire. Ces dispositions ont montré leur efficacité puisqu'à l'issue du renouvellement de 2020 le nombre de femmes conseillère communautaire a augmenté de plus de 4 points et atteint désormais. Près de 39%. Alors le sujet de la parité dans l'intercommunalité son amélioration ce est souvent évoquée. Il convient toutefois de rappeler que l'intercommunalité n'est pas une collectivité mais un établissement public de coopération et que ses conseillers sont donc directement issu des élections municipales puisque les conseillers ils sont les représentants de leur commune. De ce fait comme dans les syndicats. La composition de l'Assemblée communautaire se doit de respecter chaque élection municipale. Cependant la règle de la parité prévoit qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire au cours du mandat, le respect du principe de parité continue à s'appliquer et le siège de conseiller communautaire devenu vacant doit être obligatoirement pourvu par un élu communal du même sexe dans les communes disposant de plusieurs sièges. Au conseil communautaire cède règle de parité peut donc aboutir à une vacance durable du siège, provoquant une sous-représentation problématique et contestable d'une commune au sein de son EPCI. Ces situations de représentation commencent à émerger. Elles existent à Reims au Havre à Fécamp mais aussi dans des petites communes de la Nièvre ou de Vendée comme à Talmont Saint-Hilaire. Ce problème est particulièrement aigu pour les petites communes qui ne disposent que de peu de conseillers communautaires mais peut donc toucher aussi toutes les communes de plus de 1000 et peut ainsi aboutir à une grave diminution de leur représentation au sein du conseil communautaire. La loi avait d'ailleurs perçu dès le départ. Ces difficultés en prévoyant une dérogation au principe de remplacement par un élu du même sexe. Pour les communes ne disposant que d'un seul conseiller communautaire. Il convient donc et c'est l'objet de cet humble, proposition de loi de corriger cette rupture de l'égalité d'égalité pour les autres communes. C'est-à-dire celles de plus de 1000, car pourquoi l'amoindrissement de la représentation serait-il toléré dans certains cas et pas dans d'autres et je voudrais ici rassurer mes collègues qui pourraient craindre que ce projet de loi ne soit une atteinte à la parité. La plupart des exemples que j'ai cités, que j'ai cité laisse penser que dans beaucoup de cas, ces dispositions risquent de bénéficier aux femmes car à ce jour, il y a je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait diagnostic plus de démissions d'hommes que de femmes. En outre, cette application stricte du principe de parité peut aboutir à ce que j'appelle des accidents démocratique fâcheux. Comme un amoindrissement des droits de l'opposition, celle-ci pouvant perdre toute représentation au conseil communautaire quand elle n'a qu'un siège alors même que le pluralisme des courants d'idées a acquis valeur constitutionnelle. Donc je le disais tout à l'heure si aujourd'hui ces situations peuvent être encore peu nombreuses. Nul ne peut ignorer le risque de multiplication de ce type de situation. Dans cette crise de l'engagement, je rappellerai l'augmentation préoccupante des démissions d'élus municipaux depuis 2020 le nombre de démissions des maires depuis 2020 célèbre aujourd'hui, mes chers collègues à 930 et je ne connais pas à ce stade, le nombre de démissions de conseillers municipaux mais il y a la gravité. Monsieur le président, mes chers collègues permettez-moi de remercier très chaleureusement notre rapporteur Nadine l'euro pour la très grande qualité de son travail et son écoute et n'oublions pas mes chers collègues, que l'intercommunalité nécessite encore beaucoup d'abaissement et que l'engagement comme la démocratie sont aujourd'hui tous les deux d'une grande fragilité avec humilité. Madame la rapporteur Monsieur le Président Madame la Ministre disons que ce petit pas législative qui vous est proposé aujourd'hui peut être considéré comme un grand pas pour la démocratie. Je vous remercie. Merci cher collègue.

Merci. Monsieur le président, madame la ministre. Monsieur le président de la commission des lois, chère Françoise, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui entend répondre à un problème comme vous l'avez dit ponctuel mais qui mérite toute notre attention. Les vacances durables de sièges au sein des conseils communautaires faute de candidats de même sexe pour remplacer le conseiller démissionnaire. Dans un contexte de crise des vocations et de désintérêt croissant pour le mandat communautaire les exemples locaux de telles vacances se multiplient et aboutissent parfois à des situations ubuesques comme cela a été rapporté par l'auteur de la proposition de loi. Ce constat semble d'ailleurs partagé par certains de nos collègues députés Élodie Jacquier-Laforge et Raphaël Schellenberger dans leur rapport sur la parité dans les fonctions électives et exécutive du bloc communal rappelait les marges de manoeuvre nul des des élus locaux fassent une telle obligation. L'ancien ministre des collectivités territoriales Joël Garreau, répondant à une question écrite de Madame Gatel avait lui-même constaté que ces situations qui sont certes exceptionnel pourrait faire l'objet d'une attention particulière à l'occasion d'un prochain vecteur législatif, hé bien nous y voilà. Cette situation de vacances et particulièrement préjudiciable. Cela a été dit aux communes et aux intercommunalités à 3 égards. Premièrement la vacance d'un siège aboutit à un amoindrissement de la représentation des communes au sein du conseil communautaire, alors même que les intercommunalités sont désormais titulaire de nombreuses compétences qu'elles exercent souvent sur l'ensemble de leur périmètre. Deuxièmement, dans certains cas une telle vacances conduit à un amoindrissement des droits de l'opposition qui peuvent se retrouver privés de représentation au sein du conseil communautaire, faute d'avoir un réservoir de candidats de même sexe fléché ou non suffisant. Troisièmement des vacances durables sont préjudiciable au bon fonctionnement des EPCI Afsca. À fiscalité propre eux-mêmes dont les décisions pourraient être considérée comme entâchée d'un défaut de représentativité et de légitimité en particulier s'agissant des équilibres fragiles de représentation, nous connaissons tous cela entre d'une part la ville centre et les communes de plus petite taille. La solution aux difficultés des élus semblent pourtant parfaitement simple une fois qu'il est constaté l'impossibilité, faute de candidats du remplacement d'un conseiller communautaire par un conseiller municipal de même sexe, alors pourquoi ne pas ouvrir la faculté de le remplacer par un conseiller d'un autre sexe la présente, proposition de loi apporte donc une solution pragmatique et encadré en prévoyant. Pour les seules communes de plus de 1000 habitants représentés par plusieurs sièges communautaire et lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal de même sexe candidat à ce siège de le pourvoir par le suivant de liste fléché est est élu conseiller municipal sans tenir compte de son sexe et si il n'y a pas non plus de conseiller municipal fléché sur la liste concernés le siège serait alors pourvu par le 1er conseiller municipal élu sur la liste n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire sans tenir compte de son sexe ce dispositif me paraît constituer un point d'équilibre satisfaisant entre l'exigence d'égale représentation des hommes et des femmes et l'indispensable représentation juste et continue des communes au sein des conseils communautaires. Ce dispositif n'étant applicable qu'aux communes de plus de 1000 habitants représentés par plusieurs. Sièges au conseil communautaire. Se représente environ 30% des communes. Je souhaite être clair sur ce point, il ne s'agit pas ici de modifier les situations des communes de moins de 1000 habitants. Ainsi n'enlevant rien au droit existant. Ces assouplissements éviterait par tout moyen une vacance de sièges qui n'est jamais souhaitable et opérerait une nouvelle conciliation des principes de parité et de représentation des communes au sein des conseils communautaires communautaires afin d'éviter que comme c'est le cas actuellement, l'un de ses précis PFAS. Échec à l'autre. La principale originalité du dispositif et de n'être applicable qu'à l'issue de la première année du mandat. Ce faisant, elle permet d'écarter toute possibilité de contournement du dispositif pour affaiblir l'application du principe de parité par des démissions en cascade, dès les élections passées. La rédaction de la proposition de loi initial a été retravaillé. En commission afin de s'assurer que le dispositif ne s'applique qu'à compter d'une année suivant la date d'installation du conseil municipal, qu'ils soient issus du renouvellement général ou d'un renouvellement local aucune vacances intervenu dans le délai d'un an à compter du début de mandat ne pourrait donc se voient appliquer les dispositions de la proposition de loi. Je souhaite terminer mon introduit Pour remercier Françoise Gatel pour la qualité aussi de sa rédaction. Et pour le travail que nous avons pu accomplir ensemble. Durant cet examen de cette proposition de loi, je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Là. La parole est maintenant Madame Dominique Faure Ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, j'en aurai le buffet madame la rapporteure Nadine. Madame la sénatrice Françoise Gatel mesdames et messieurs les sénateurs, nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de la niche du groupe UC pour étudier la proposition de loi de la sénatrice Françoise Gatel visant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires continuité de la représentation des communes au sein des EPCI qui pour la chambre haute, que vous êtes est un sujet de préoccupation légitime. Comme vous le savez bien sûr l'article L 273 tirer 10 du code électoral prévoit que lorsqu'un siège de conseiller communautaire est devenu vacant pour quelque cause que ce soit ce dernier pourvu par le candidat de même sexe. Élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire sur laquelle le candidat démissionnaire a été élu. La loi prévoit également. Que lorsqu'il n'y a plus de candidats de même sexe pour pouvoir ce siège, il est fait appel au 1er conseiller municipal de même sexe sur la liste des conseillers municipaux non candidat au mandat de conseiller communautaire. Et puis enfin, lorsqu'il n'existe plus aucun conseiller satisfaisant aux conditions précitées. Le code électoral prévoit que le siège concernés restent vacants jusqu'au prochain renouvellement du conseil du conseil municipal de la commune et c'est précisément de ce dernier point que la PPL de la présidente Gatel nous invite à débattre aujourd'hui. Elle souligne en effet. Que telle qu'est conçue la loi. Elle peut conduire ponctuellement et malheureusement à ce qu'une commune ne soit plus représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale auquel elle appartient. Ce dispositif législatif vise bien entendu en première intention et conformément à ce que prévoit la Constitution à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives objectif que je partage totalement et dans tout mon parcours d'élu local me permet de savoir à quel point il est cardinal pour la vitalité et la diversité démocratique de nos territoires. Il est important néanmoins d'affirmer que l'absence de représentation d'une commune au sein du conseil communautaire de son EPCI représente une difficulté significative pour la dite commune. Le cas n'est pas complètement d'école si nous ne disposons pas de chiffre consolidé permettant d'établir que le phénomène serait massif. Et je ne croit d'ailleurs pas qu'il le soit quelques situations ponctuelles, nous ont été remontés et témoigne du fait que l'hypothèse peut se présenter. Bien sûr, la parité est un objectif que nous devons poursuivre sans relâche et avec ma collègue, Isabelle Rome, nous savons à quel point cette parité fragile. Les propositions formulées par la mission flash madame la rapporteur que vous avez cité d'Élodie Jacquier-Laforge et de Raphaël Schellenberger sous la précédente mandature démontre d'ailleurs que notre dispositif électoral présente encore quelques angles morts et que nous devons donc achevé le mouvement entrepris par la loi du 6 juin 2000 qui avait prévu pour la première fois la prise en compte de la parité dans les élections communales. Et à ma connaissance la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le sujet nous invite aussi au pragmatisme. Ce dernier considère en effet qu'il est loisible au législateur d'aborder des des lits des dispositions contraignantes ou incitatives pour atteindre l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Ce qui signifie que nous avons une obligation de résultat, mais que nous sommes libres des moyens que nous donnons aux collectivités pour y parvenir. La jurisprudence du même conseil constitutionnel rappelle d'ailleurs que le principe de parité doit être concilié avec d'autres impératifs. Il doit en particulier s'articuler avec le principe inscrit à l'article 4 de la Constitution, lequel prescrit de ne pas porter atteinte aux expressions pluralistes des opinions. Eh bien je crois que le principe de parité doit aussi s'articuler avec l'exigence de représentation effective des communes au sein des organes délibérants des EPCI auxquelles elles appartiennent. Il y a là un enjeu de continuité de leur représentation et de leur participation à la délibération collective, une commune qui ne plus aux décisions de son EPCI. C'est une commune qui dans tous les domaines de compétences de cette PC il ne pourra plus se faire entendre. C'est une commune qui aura donc le sentiment d'être dépossédés d'une partie de ses choix et je suis trop attaché à ce que la gouvernance locale fonctionne bien pour admettent que cette hypothèse puisse même dans un nombre de cas limités se réaliser. Vous le savez aussi bien que moi mais la coopération intercommunale et construite pour fonctionner sur la base de la participation effective et active des communes. Si nous n'étions pas persuadé de la nécessité de favoriser une association effective des communes au fonctionnement de leur établissement de coopération intercommunale. Nous n'aurions pas adopté dans la loi Engagement et proximité les dispositions relatives au pacte de gouvernance ou celle. Relative à la conférence des maires. Soyons cohérents. Si nous voulons que l'intercommunalité fonctionne bien et cela doit être un objectif partagé, nous devons garantir à chaque commune qu'elle pourra en toute hypothèse participer effectivement aux délibérations de son EPCI. En sens inverse. J'ai écouté attentivement ceux d'entre vous en commission qui ont exprimé leurs doutes et je salue l'engagement qu'il marque en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas sûr néanmoins que la conséquence logique de cet engagement, doivent être d'en venir à priver une commune de sa représentation au sein de l'EPCI. La proposition faite par la présidente Gatel qui consiste seulement dans le cas résiduels dans lequel plus aucun conseiller de même sexe ne pourrait occuper le siège vacant à admettre qu'un conseiller de sexe différent l'occupe. Me semble en tout état de cause, tenir la Crète, elle n'a aucunement pour objectif de revenir sur nos ambitions en matière de parité. Mais elle permet de traiter le cas dans lequel l'application des règles en matière de parité, conduit à une impasse institutionnelle et à la fin, démocratique, vous l'aurez compris la problématique de la représentation des communes au sein des conseils communautaires est un sujet qui retient toute mon attention. Face à ce problème bien identifié votre solution de bon sens. Madame la sénatrice Gatel émerge. Je souhaite à la soutenir. Aujourd'hui le texte que vous proposez un texte de bon sens, c'est pour cela que j'aimais émets un avis favorable sur ce texte. Je signale toutefois. Qu'il nous faudra. Dans la suite de la discussion parlementaire s'assurer et faire confirmer par la délibération collective que ce texte ne porte pas atteinte au principe de parité auquel je ne peux que réitérer mon plein et entier attachement je vous Première. Merci. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Jean il vaut pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, je pense que tout le monde salue les progrès effectués ces dernières années en matière de parité de mixité au sein des institutions publiques, bien sûr, il nous reste beaucoup à accomplir. Nous avons une marge de progrès indéniable au sein de la représentation politique et plus largement dans l'accès à toutes ses fonctions publiques, surtout pour des postes à responsabilité et je pense au-delà de la question du sexe à celle des origines sociales. Le sujet est connue depuis plusieurs décennies avec au départ la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 qui a complété l'article 3 de la Constitution imposant que la loi favorise l'égal accès accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. S'en est suivi très. Spécifiquement la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes, des hommes aux mandats au électoraux et fonctions électives. La loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, puis des dispositions aux scènes d'autres tests plus vaste. Je pense en particulier à la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des conseillers communautaires mais également à la loi du 27 décembre 2019 relatives à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique. Bref, même s'il reste beaucoup à faire, reconnaissant tout de même que le législateur n'a pas puis attache seulement chacun conviendra également que les mécanismes incitatifs voire coercitifs vue de rendre effective cette représentation paritaire ne doivent pas conduire à déblocage le droit aujourd'hui applicable au conseil communautaire a déjà été niquer, je le rappelle brièvement en citant l'article L 273 10 du cours d'électoral dans les communes de plus de 1000 habitants, lorsque le siège du conseil communautaire devient Vacca pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe et du conseil municipal. Le conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer, être élu. Les auteurs de la proposition de loi en raison de souligner que cette disposition pose pas avoir des difficultés d'application. Un particulier dans le cas où un seul siège est à pouvoir le candidat complémentaire qui figure un deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseil communautaire élu or puisque le remplaçant de plus être de sexe différent la personne figurera en 2ème position du fait de cette règle de parité de sexe différent de la tête de liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. C'est évidemment regrettable et il est nécessaire de rectifier ce dispositif. Il a été souligné par la rapporteure que les objectifs poursuivis par l'auteur de la proposition de loi était partagé quand même bien la rédaction du texte initialement présenté a dû être ajustés afin de le rendre au mieux opérante. Le texte initial prévoyait de s'appliquer seulement au terme de la première année suivant le renouvellement général des conseils municipaux. La nouvelle rédaction a écarté de décalage d'un an, de sorte que même dans les premières années du mandat aucune vacances ne pourrait pas se voir appliquer les dispositions de la PPL, tout cela me paraît aboutir à un travail de qualité. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont pris une part active aussi, vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe RDSE E votera en faveur de ce texte. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre monsieur le président de la commission des lois. Madame le rapporteur. Mes chers collègues si l'unité dans la diversité, la devise de l'Union européenne, ça pourrait être aussi celle de toutes les intercommunalités de France composé. Des plus de 34.000 communes. Elles sont toutes différentes plus ou moins grandes, plus ou moins riches plus ou moins vaste, elles se sont progressivement regroupées pour exercer leurs compétences dans un contexte de décentralisation leur regroupement a fait émerger une nouvelle gouvernance fondée sur la légitimité des élus municipaux au Sénat. Nous savons que l'intercommunalité est un outil de coopération au sein duquel chaque commune doit avoir sa juste représentation mais l'intercommunalité soulève des questions légitimes comme la représentativité de son conseil à la fois entre les oppositions et la majorité entre les communes selon la population et entre les hommes et les femmes ainsi un équilibre subtil et tu as trouvé entre l'exigence légale d'égalité homme femme et l'indispensable représentation juste et continue des communes au sein des conseils communautaires, selon les mots de notre collègue excellente rapporteure Nadine. Ainsi, la proposition de loi que nous examinons ce jour de notre estimé présidente de la délégation des collectivités territoriales. Françoise Gatel tend à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Je me félicite que notre collègue se saisissent de ce sujet important pour la démocratie locale et qui touche particulièrement les intercommunalités de la Seine-Maritime aujourd'hui nous débattons d'un cas sert particuliers et ponctuels mais qui n'enlève rien à son caractère problématique s'agit de la vacance d'un siège, faute de candidats du même sexe pour remplacer un conseiller communautaire démissionnaire des règles actuelles ont démontré leurs limites. La vacance durable de sièges communautaire conduit à un amoindrissement de la représentation des communes ou des droits de l'opposition ou encore d'un défaut de représentativité et de légitimité un siège durablement vide au conseil communautaire alimente un sentiment pernicieux dont nous ne pouvons faire l'économie, l'incompréhension tant on connaît l'impact des EPCI dans la vie de nos concitoyens. Le pragmatisme du Sénat et donc une fois encore exigé pour répondre l'insatisfaisante règles actuelles devant concilier le principe de parité et la représentation des communes. L'occasion nous est donc donné de mesurer les effets inattendus de l'exigence légale qu'est la parité. Plusieurs exemples dans mon département attestent de la nécessité de faire évoluer une règle générale et absolue qui résiste. Qui résiste pardon, À Turville sur Arc en Seine Maritime. Le maire a dû composer avec les volontés, les aspirations, les attentes de certains certains. Il a souhaité s'entourer de 2 adjointe car elles avaient vraiment manifesté leur souhait de s'engager dans cette commune de 1300 habitants. Eh bien non. La parité là interdit de recruter, enfin et de nommer ces 2 adjointe, il a fallu choisir un homme. Qui n'était pas forcément volontaires et une des 2 femmes a dû devenir simple conseillère municipale déléguée, vous savez l'engagement devient rare et il ne faut ne pas gaspiller les chances d'avoir des élus volontaire qu'il soit homme ou femme. Autre exemple, celui d'une commune que je connais particulièrement bien puisque j'y suis élu, c'est celle du Havre ou le conseil municipal siège dans sa totalité au conseil communautaire. Or, depuis le 3 janvier 2022 un siège est vacant au conseil communautaire car la conseillère municipale de la majorité du Havre dernièrement. Désigné un con c'est un collègue masculin ne peut pas siéger au sien du conseil communautaire. C'est la seule des élus du conseil municipal du Havre de ne qui n'a pas le droit de siéger au sein de l'instance inter-communal. C'est la même chose pour l'agglomération de Fécamp et voir celle de Bolbec ah sur laquelle nous échangions à l'heure avec notre collègue brûle en conséquence, en ce qui concerne la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et jusqu'en 2026. Eh bien nous avons un siège vacant quoi quand comment le comprendre il n'est pas nécessaire d'avoir effectivement un élu. De même sexe ainsi la place des communes n'est pas assurée au sein d'interconnecter dans leur intégralité et c'est là peut être particulièrement verrait dans les communes les plus rurales compte la parité prédominent sur la représentation démocratique. Il est donc urgent d'adopter cette très bonne proposition de loi particulièrement pragmatique. Qui. Correspond à une vraie difficulté on sert parfois mineurs, mais une autre difficulté réelle de terrain. C'est pour toutes ces bonnes raisons que notre groupe votera cette proposition de loi. Merci cher collègue. La parole est maintenant le ce Denis Wattebled pour le groupe les indépendants pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre. Madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Certaines communes sont confrontées à des situations durables de vacance de sièges au sein des conseils communautaires. Faute de candidats de même sexe pour remplacer le conseiller du ministre démissionnaire. Certes, il s'agit d'un dysfonctionnement exceptionnel. Mais ils peuvent être amenés à se multiplier. C'est pour pourquoi je me félicite de l'initiative, notre collègue Françoise Gatel afin de pallier ces difficultés déjà rencontrées par des élus locaux. En effet ces situations de vacances peuvent être à bien des égards dommageable pour les communes. Les intercomités et celui-là a été relevé à juste titre par la rapporteure. Affaiblissement de leurs plantations des communes au sein des conseils communautaires. Diminution des droits de l'opposition ou encore atteinte à la représentativité et à la légitimité des décisions. Afin d'apporter une ce sont pragmatiques, à situation certes ponctuelle mais portant toutefois atteinte à la démocratie. La proposition de loi prévoit, pour les seules communes de plus de 1000 habitants représentés par plusieurs leur siège au sein des Clotaire et lorsqu'il n'existe. Pas de conseillers municipaux fléché ou pas. De même sexe candidat à ce siège de le pourvoir par le suivant de liste fléché et élu au conseil municipal sans tenir compte de son sexe. Lorsque la liste concernés ne comporte plus de conseillers municipaux 10 fléchés. Le siège sera l'air alors pourvu par le 1er conseiller municipal élu sur la liste n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire sans compte. Tenir compte de son sexe. Ces ajustements apporte une réponse équilibrée au dysfonctionnement ponctuel constaté tout en préservant à la fois l'impérieuse impériosité de augmentation continue des communes au sein du conseil communautaire et l'obligation de reprendre sur l'égal. Égal des hommes et des femmes. Enfin. Je rejoins la position de la Commission, lorsque celle-ci a souhaité apporter une modification au texte initial, en précisant que le dispositif n'a s'appliquerait à compter d'une année suivant la date d'installation du conseil municipal afin notamment de tenir compte d'éventuels renouvelant municipaux et locaux. Monsieur le Ministre, chers collègues, la pression de loi qui nous est présenté constitue un texte correctif pertinents, répondant à une difficulté ponctuelle à laquelle plusieurs collectivités se sont déjà heurtés. La vacance durable au sein d'un conseil communautaire. Elle remédie ainsi à des soupions pouvoir porter atteinte au bon exercice de la démocratie. Ainsi le groupe les indépendants votera pour ce texte. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste pour 4 minutes. Madame la ministre madame l'auteur, chère Françoise madame la rapporteure, chers collègues. La représentativité, la parité la diversité dans les instances décisionnaires sont considérées de manière assez généralisé désormais. Comme bénéfique dans la conduite des affaires publiques et pas que d'ailleurs. Sans conteste les lois sur la parité hommes-femmes ont permis de faire progresser cette parité au sein des communes, puis les conseillers communautaires. L'application de cette contrainte paritaire à faciliter une entrée massive des femmes dans les conseils municipaux des villes de plus de 3500 habitants alors que leur proportion n'était que de 25,7% dans les conseils municipaux issu des élections de 2004, 2995. Celle-ci est grimpé. À 48,5% en 2008. Dans ces communes et la part des femmes dans les conseils communautaires a augmenté également et atteint 35 8 %. Après les élections de 2020. Cette obligation a donc des effets mais mais demeure encore indispensable. Comme la proportion des femmes a augment n'a augmenté que parmi les jeunes élus cela augure de renouvellement à terme encore plus paritaire. Parallèlement. La vocation des élus s'essouffle. Nous l'avons tous observé le nombre de démissions tend à déstabiliser les copies des travaux des EPCI les règles actuelles posent aux communes de plus de 1000 habitants, une règle de parité pour la constitution des listes de candidats au conseil communautaire. Elles obligent aussi à Lire la parité tout lors du mandat. Avec une femme représentant une commune au sein d'un EPCI assis ne pourra être remplacé que par une femme de cette pas liste à défaut le siège restera vacant le mécanisme vous a été expliqué par mes collègues précédemment. C'est bien ce problème de vacances que l'auteur a souhaité répondre. Les EPCI exerce des compétences essentielles pour la vie de la commune aussi l'absence de conseiller au sein des conseils communautaires peut être préjudiciable. La compréhension de nos élus locaux sur ses difficultés de représentativité. S'est installer de manière durable. Je pense d'ailleurs que personne sur ces bords ne pourra. Nous accuser d'être insensible aux questions de représentativité au sein des intercommunalités, y compris de statut pacifie spécifique et aux conséquences que cela aussi sur la compréhension de l'eau citoyen sur le comment ça marche. De la gestion des déchets, des routes jusqu'aux transports en commun. Et autres compétences exercées. La proposition de loi issu des travaux de la Commission cherche à répondre à cette incongruité qui voudrait qu'une commune aucune opposition ne puisse plus être présenté au Tchad le PCI auquel elle participe. Alors certes. La réponse de cette PPL et peut-être parfaite sur l'application de la parité et notre groupe restera très attentif aux utilisations qui sur en fait de cette loi qui n'entend répondre en fait initialement qu'à des situations ponctuelles qui doivent rester isolés, le restaurant. L'imagination de certains hommes politiques, est assez. Comment dire. Sans limite 10 rando, j'ai quelques exemples, j'aurai pas le temps de vous les donner. La rédaction semble apporter un certain nombre de garde-fous. En l'espèce avec l'instauration de délai de réserve d'un an, suivant la station de Causses municipaux afin d'éviter toute tentative d'effet d'aubaine post-élection mais toute atteinte à l'obligation de parité peut avoir des effets négatifs. Même si elle ne remet pas en cause les dispositions liées à la parité, mais permet leur adaptation en cas d'impossibilité matérielle de remplacer les conseillers communautaires. D'autres groupes a conscience de l'importance de la représentativité de l'ensemble des idées et des territoires au sein d'une assemblée et a toujours attiré l'attention sur les difficultés des positions minoritaires au sein des assemblées par exemple en terme de représentativité dans les commissions mixtes paritaires au Sénat. Dans sa grande majorité notre groupe de peut se satisfaire de ce type de solution pourquoi de pas permet. Bullock pourquoi ne pas limiter aux villes de moins de 3500 habitants et donc majoritairement d'Andrew voient dans cette mesure une solution moyen d'un vrai problème. Pour autant, certains d'entre nous dont je fais partie voteront ce texte en restant très attentif aux résultats de l'application de ces dispositions au regard des progrès obtenus dans une meilleure et plus juste représentativité des femmes au sein de nos institutions locales. La parole est maintenant au président Alain Richard pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Merci monsieur le président. Mais Monsieur et Madame la Ministre de monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. le sujet sur lequel nous avons à délibérer sur la proposition judicieuse de notre collègue Françoise Gatel résulte de la conjonction de 2 principes électoraux le 1er c'est celui du fléchage et de l'élection des conseillers communautaires à l'intérieur des listes municipales en gardant. Ce que j'appellerais un chaînage une solidarité permanente. Et une cohérence entre les représentations communes les représentations intercommunal. Ce système est parfois discutée et parfois confronté à d'autres. Et j'entends avec beaucoup d'irritation continuer à employer l'expression d'élection directe des conseillers communautaires pour parler d'autre chose qui serait une élection supra communal. Carrément extérieur aux conseils municipaux, ce qui serait à mon ce qui changerait fondamentalement la neige. Sur des intercommunalités mais dans le système où nous sommes il y a une cohérence, il y a une solidarité entre la liste municipale et les élus communautaires. Que ce soit dans la majorité ou dans la minorité. Et le second principe. Qu'il s'agit évidemment de faire de faire appliquer le plus efficacement possible, c'est celui de la parité qui s'applique dans le cas des élections communautaires. De façon assez spécifique. Car dans toutes les élections au scrutin de liste ou s'impose une composition paritaire des listes. Il n'y a que pour le l'élection interne à la municipale du conseil communautaire que s'impose une règle spécifique de remplacement, que ce soit pour le Parlement européen que ce soit pour les conseils régionaux. Que ce soit pour les conseils municipaux même. La succession d'un siège vacant se fait toujours par le suivant de liste. Quel que soit son sexe ou son genre et il faut bien dire que la précaution. Documentaire qui a été instaurée dans la loi de 2013, à propos du remplacement dans les conseils communautaires était probablement un coup d'épée dans l'eau car compte tenu du nombre de cas dans lesquels des communes n'ont qu'un nombre impair. De. 2 conseillers communautaires soit un soit trois avec une grande majorité de têtes de liste. Homme. Une règle de succession sans fléchage le sexe aboutirait probablement à l'arrivée en cours de mandat de plus de conseillère communautaire femme que la disposition actuelle mais enfin. On en fera le bilan à jour, c'est la seule. C'est le seul cas dans lequel ne s'applique. Il en résulte dans de de 2 types de situations qui ont été décrites celle décrite par Madame Canayer à propos des grandes villes qui occupe. Une très grande proportion du conseil communautaire et donc dont tous les conseillers ou pratiquement tous les conseillers son conseiller communautaire et au contraire, les cas de minorité. Mais également en général dans les communes centres où il y a une forte proportion de conseillers communautaires parmi les conseillers municipaux et dans les 2 cas il peut y avoir en effet un déficit. Présentation parce que le dernier poste vacant ne peut pas être remplacé par un conseiller. Communautaire ou. Ou municipal municipal de même sexe. Il me semble donc il nous a donc semblé en réfléchissant dans notre groupe que c'était un aménagement de bon sens à l'application d'une règle qui est une règle spécifique et qui n'a pas forcément démontrer sa plus grande efficacité en matière de respect de la parité, c'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra également, c'est une proposition de loi. Merci monsieur le président. La parole est maintenant monsieur Éric Kerrouche pour le groupe socialiste pour six minutes.

Monsieur le président, madame la ministre madame la rapporteure. Chers collègues. Parfois les règles qui s'appliquent aux collectivités territoriales peuvent relever du cabinet de de curiosité. Et il s'avère que notre collègue Françoise Gatel à des dons pour les débusquer. En même temps, il s'avère que parfois elle participe. De la création de ces bizarreries du vestiaire. Je pense par exemple à la commune communautés néanmoins néanmoins. Dans Dans les 2 cas, ce sont des mesures qui. Ont leur intérêt et il s'avère que en ce qui concerne ce le texte dont on discute ce soir. Il est évident qu'il convient de corriger ce qu'on peut appeler une bizarrerie parce que c'est de cela qu'on parle, on va pas dire que ce cas de figure. est le cas le plus courant au sein des intercommunalités. Néanmoins, on peut se demander pourquoi il existe encore et tout le monde a bien compris que ce texte concernés le remplacement. Pour les communes de plus de 1000 habitants. Des conseillers communautaires qui. En bout de liste. Serait toujours disponible mais ne pourrait pas être présent puisque, en effet, il ne pourrait plus y avoir d'alternance homme femme ou femme homme pourquoi laisser vacant c'est postes si il y a une possibilité de remplacement qui a priori participe du bon sens

l'exotisme, on va dire du scrutin de nos communes de moins de 1000 habitants. Je vous rappelle que, il n'y a pas si longtemps. On pouvait être élu à l'insu de son plein gré. Je vous rappelle les possibilités de panachage. Je vous rappelle aussi que ce scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants fait que ben d'une certaine façon on a un Tir au pigeon qui se fait souvent au détriment d'ailleurs du maire celui qui est identifié comme prenant les décisions l'autre point lié à ce scrutin. Des communes de moins de 1000 habitants concerne la parité puisque la parité ne lui est pas tu ne lui est pas applicable et donc d'une certaine façon. Il faudrait également unifier la question de. Ce mode de scrutin de telle façon à ce que, quelle que soit la commune dans laquelle on se trouve le mode de scrutin soit le même ce qui imposera de manière définitive la parité, y compris dans dans les communes de moins de 1000 habitants qui, si je ne m'abuse représente un peu plus de 18.000 communes françaises ce qui encore une fois là est complètement atypique. Le 2ème sujet touchés par cette PPL c'est celui de la parité parce que la proposition renvoie de fait à la question plus large de la parité femmes-hommes au sein des intercommunalités et des moyens d'y parvenir. Or je regrette juste même si je le comprends que l'amendement que nous avons porté sur. La parité aient été jugée irrecevable. Je vous rappelle juste que celui-ci reprenait une proposition de notre groupe formulées lors de l'examen de la loi Engagement et proximité et traduite dans une proposition de loi que j'avais été posée par ailleurs. L'idée c'était de faire en sorte, je vous le rappelle qu'il y a une parité miroir au sein de l'exécutif intercommunal, c'est-à-dire en gros que la proportion de femmes. Vice-présidente soit équivalente au moins à la proportion de ce que représentaient les femmes à l'intérieur du conseil communautaire, cet amendement avait été. Acceptée, je vous le rappelle, de haute lutte dans l'examen de loi engagement et proximité. Mais il avait été. Supprimé Madame la Ministre, vous n'en étiez pas encore responsable à l'époque par la majorité présidentielle de l'Assemblée nationale et cette suppression avait été entériné par la commission mixte paritaire. Malgré une proposition de rédaction pendant cette CMP. Je vous rappelle juste que la disposition qui avait été introduite est la suivante, avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiés pour étendre l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements. À ma connaissance, nous sommes le 15 mars 2023. Et ces dispositions ne trouve toujours pas à s'appliquer. Et donc la prise en compte de cet amendement aurait été une bonne chose et il aurait permis de réguler ce qui reste un problème. Néanmoins, dans l'attente parce que nous continuerons à porter cette proposition dans le temps et que d'une certaine façon elle dépasse donc le cadre de cette proposition de loi nous voterons pour une proposition qui nous sommes, de qui nous semble de bon sens, d'une part. Mais d'autre part, nous ne voterons pas pour l'amendement unique qui nous semble aller. Au-delà du périmètre de la correction proposée par Françoise Gatel je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Cécile Cukierman. Pour le groupe CRCE pour 4 minutes.

Bonsoir monsieur le Président Madame la Ministre. Mes chers collègues. On va y aller. Cette proposition de loi permet une continuité. Cela a été dit. De la représentation dans les conseils communautaires dans un contexte où les EPCI d'ailleurs exerce des compétences structurante de plus en plus hein. Part importante qui ont un impact fort sur le quotidien des communes et donc des habitants de ce fait à travers l'objet. L'article de cette proposition de loi, l'objectif est bien d'assurer la représentation continue des communes comme l'a rappelé. Françoise Gatel qui sont des collectivités territoriales au sein des groupements les EPCI via les élus nécessaires. Nous savons que cette proposition de loi n'est pas discuter pour remettre en cause le principe de parité mais au contraire certaines situations vécues par nos élus locaux qui mérite d'être entendus et nous devons compte cela est possible a porté bien évidemment les des solutions et des réponses concrètes. Alors. Je l'ai entendu également, il y a des inquiétudes. Je crois, c'est de faire en tout cas pas offense à l'auteur de cette proposition de loi ni au travail de la rapporteure que de dire que l'enjeu de cette proposition de loi concerne et cela a été bien rappelé quelques communes et donc ce n'est pas une remise en cause du principe de la parité et de la représentation, même si d'ailleurs Agnès Canayer le rappeler, je crois que nous avons tous des exemples parfois aussi. Comme on dans la constitution des exécutifs locaux, parfois on arrive à d'autres aberrations qui font qu'un adjoint homme a finalement assez peu délégation quand une con. Une femme conseillère déléguée se retrouve avec beaucoup de délégations. Pour gérer tout ceci tout cela n'est pas remis en cause à travers cette proposition de loi. Donc en amendant la règle de droit avec cette proposition. Nous permettons aussi et et je veux le souligner parce que finalement ce sont peut-être les plus concernés, nous permettant ainsi au groupe d'opposition. De faire valoir leurs voix au sein du conseil communautaire, là encore, cela vient d'être rappelé c'est souvent sur ces listes là. Factuellement, que le nombre d'élus fléchés pour siéger au conseil de communauté vient à manquer. Il ne dispose pas d'une liste suffisante de remplaçant ou de remplaçante pour assurer le remplacement de la personne démissionnaire du même sexe. Cela peut donc entraîner une non représentation et ainsi mettre en difficulté le droit d'expression en tant qu'élu d'opposition. Cette proposition de loi donc du sens elle permettrait une représentation pérenne au sein des conseils communautaires mais surtout corrigerait la législation qui n'a pas pris en compte des situations ponctuelles particulières qui peuvent exister. Ainsi, avec cette proposition de loi. Quand il n'existe, il n'existera pas de conseiller communautaire de même sexe sur la liste communautaire. On pourra nommer le suivant de la liste sans tenir compte de son sexe afin d'assurer la mission première confiée aux élus, celle de la représentation de leur commune et de leur population, et ce quel que soit leur sexe étant attaché au principe de démocratie d'et de représentation des communes au sein des EPCI nous voterons bien évidemment sa proposition de loi, qui permet comme je l'ai dit d'apporter une solution à des problématiques rencontrées au sein de nos collectivités et il nous reste devant nous l'éternel chantier fondamental jamais atteint mais qui. Mérite essentiellement beaucoup de débats et d'évolution de société qui est la question de la place des femmes et des hommes dans les la vie politique locale dans la vie politique nationale mais c'est une simple proposition de loi suffisait à régler des problèmes de société, cela se saurait. En l'état, nous voterons cette PPL. Merci cher connaît. La parole est maintenant madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union centriste pour six minutes. Monsieur le président. La c'est le président de la commission des lois, mes chers collègues arrivés 8ème dans ce débat qui ne pose strictement aucun problème. Je vais évidemment pas utiliser la totalité de mon temps de parole. Remercier Madame Gatel dont la évidemment la perspicacité encore frappé. Et plutôt dire que évidemment notre groupe soutient ce texte ce qu'il répond à un problème ponctuel que tout le monde est d'accord. Nos collègues à l'Assemblée nationale, le gouvernement donc vraiment aucune aucune espèce de difficulté. Vous dire Madame le Ministre comme c'est important d'avoir cette délégation aux collectivités locales tellement attentive même pour régler des problèmes qui peuvent sembler insignifiants sauf pour les gens qui sont directement concernés parce que c'est toujours, c'est toujours évidemment. Le cas donc moi je n'ai absolument rien d'autre à ajouter. Que il faut évidemment écouter le Sénat et que le principe des niches parlementaires et d'autant plus importante qu'il qu'il peut porter évidemment des solutions pour ceux qui en ont besoin. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Très bien, cher collègue, la parole est maintenant madame Laure Darcos pour les républicains pour cinq minutes. Madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires présentée par notre collègue Françoise Gatel, président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales à la décentralisation. Je tiens à saluer nos son initiative hein particulièrement judicieuse ainsi que le travail de notre collègue. Rapporteur Nadine. Comme vous le savez, la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux des conseillers communautaires a prévu que pour les communes de plus de 1000 habitants. La liste des candidats au siège de conseiller communautaire soit composée alternativement de candidats de chaque sexe elle a contribué à améliorer la féminisation de la vie politique locale et nous nous en réjouissons grâce aux lois adoptées depuis plus de 20 ans l'engagement des femmes a considérablement progressé dans les assemblées élues des collectivités territoriales, même si nous pouvons déplorer que la parité réelle ne soit toujours pas atteinte. La part des femmes dans les conseils municipaux s'élève à ce jour à 48,5%. La composition des organes délibérants et des exécutifs des intercommunalités reste en revanche en parfaite et les EPCI représente sans aucun doute une zone blanche de la parité. Ainsi que le relevé le Haut Conseil à l'égalité, en 2020 dans les conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre. La part des femmes a certes augmenté de 5,7, des vice-, présidents de. 6 points et c'est des présidents de 2 points en absolu, cependant elle n'atteint respectivement que 36 pour 125,6% et 11% de la composition générale de ces instances. Bien entendu il ne saurait être question de mettre en cause ces avancées dont la portée est loin d'être symbolique puisqu'elle favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Ce n'est d'ailleurs pas l'intention de la proposition de notre collègue Françoise Gatel. Pour autant, l'obligation de parité institué par le législateur peut conduire à des situations incongrues qui n'avait pas été identifiée à l'origine et que le texte examiné aujourd'hui a pour objectif de courses La possibilité de remplacer une conseillère ou un conseiller communautaire démissionnaire par un élu du même sexe n'est pas sans conséquence puisque les rend le siège vacant pendant toute la durée d'un mandat. Pour les communes concernées. Une telle situation est susceptible de créer un effet d'éviction du pouvoir intercommunal d'autant plus préjudiciable que nous connaissons tous ici l'étendue des compétences acquises au fil du temps par ces EPCI. En outre, elle peut avoir en effet pour effet de donner à la commune la plus importante de l'EPCI un poids et une représentation qui ne serait démocratiquement pas justifié là que le risque de voir les décisions de cette intercommunalité entaché d'un défaut de légitimité. Notre rapporteur signale le cas d'espèce que représente le recours gracieux formé en 2021 par le préfet de la Nièvre contre la délibération d'un conseil communautaire qui avait procédé au remplacement d'un conseiller démissionnaire de son mandat municipal par une conseillère municipale de sexe féminin, faute de candidats masculins, la délibération contestée ne pouvait être que rapporté puisque la désignation à laquelle et procédé n'étaient pas conformes au droit en en vigueur. j'ajoute que l'avenir nous ne pourrions être de plus en plus fréquemment confronté à ce type de situation en raison de l'augmentation constante des démissions d'élus locaux oui, mes chers collègues, nous ne devons pas ignorer la désaffection croissante des élus pour l'exercice d'un mandat qui s'avère à bien des égards difficile à assurer. Sur le le temps long. Les mots sont connus, les élus assument toujours plus heureux sous sa responsabilité dans des conditions d'insécurité juridique et financière grandissante. Tout le mérite de la proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel et de tenir compte de cette réalité de proposer une solution qui, sans porter atteinte à la règle de parité prévue par le code électoral permet de nous de laisser aucune commune son représentant au sein d'un conseil communautaire. Il est ainsi proposé d'inscrire dans le droit positif de facultés subsidiaire de désignation d'un conseiller municipal en remplacement d'un élu démissionnaire. La première consiste à pourvoir le siège par le 1er conseiller municipal fléché de même liste et de sexe opposé. Ou à défaut par le 1er conseiller municipal non fléchés de même liste et de sexe opposé. Une telle dérogation ne serait possible qu'à compter de l'année suivante. Suivant la date pardon d'installation du conseil municipal afin d'éviter des stratégies électoralistes inopportune visant à contourner le principe de parité, indéniablement, cette solution est de nature à répondre aux inquiétudes des élus locaux et de leur association représentative qui nous avait alertés. Elle est marquée du sceau du pragmatisme et ne porte pas atteinte au principe de parité qui je le rappelle l'institut pas un droit ou liberté que la Constitution garantit. C'est la raison pour laquelle je voterai sans réserve comme groupe en faveur de la proposition de loi qui nous est soumise. Je vous remercie et désolé d'avoir pris tout mon temps. La discussion générale est Close, nous passons la discussion du texte de la commission et avant l'article hein, j'ai un amendement hein rectifier bis. Madame Sollogoub. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement de notre collègue Hervé Maurey vise à modifier les modalités de désignation des remplaçants des conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'Ordre du tableau du conseil municipal. Si l'application de cette règle paraît opportune en ce qu'elle garantit aux maires d'être le représentant de sa commune au sein de l'intercommunalité. Les règles de remplacement du conseiller communautaire en cas de vacance définitive sont insatisfaisantes. Le code électoral prévoit ainsi que le conseiller municipal, appelé à remplacer un conseiller communautaire et le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mon mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau. Or le maire et, plus largement, le conseil municipal peuvent souhaiter qu'un autre élu et même l'élu lui-même que celui désigné en application de cette règle puisse représenter la commune au sein de l'intercommunalité pour diverses raisons, il n'est pas non plus satisfaisant que le suppléant qui a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement temporaire soit désigné selon la même règle dans les communes de moins de 1000 habitants avec un seul conseiller communautaire, le premier adjoint est ainsi obligatoirement suppléant du maire, sans possibilité d'y déroger. Or, pour un certain nombre de raisons, notamment de disponibilité, il pourrait être souhaitable que cette fonction échoit à un autre membre du conseil municipal ainsi cet amendement prévoit que le remplaçant puisse être désigné par le conseil municipal je remercie. Merci monsieur le président. Les conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants sont désormais désignés. Selon l'Ordre du tableau du conseil municipal. Cette règle vous le savez, a été adopté en 2013 par analogie avec le système du fléchage dans les communes de 1000 habitants et plus puisque, en dehors du maire et des adjoints le rang des simples conseillers municipaux dans l'Ordre du tableau dépend du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus aux élections il y a donc un lien établi avec le suffrage universel et remettre en cause le tableau et le le le suffrage universel me semble quelque peu. Dangereux. Il me semble donc pas opportun de revenir en arrière. Au risque donc de fragiliser l'équilibre retrouvé en 2013 par ailleurs s'agissant de la suppléance l'Ordre du tableau du conseil municipal qui régit la désignation des conseillers communautaires titulaire doit également être respectée dans la mesure où le conseiller suppléant a vocation à devenir conseiller titulaire si celui-ci cesse d'exercer ses fonctions. Je veux également préciser ce que j'ai dit pendant mon intervention. Cette proposition de loi vise les vacances de sièges communautaire des vacances pérenne. Or pour des communes de moins de 1000 habitants, il est peu probable qu'il y a absolument personne. Et deuxièmement cette proposition vise les communes de plus de 1000 habitants ayant plusieurs conseillers communautaires, elle ne vise pas les communes de moins de 1000 habitants qui ont donc un seul siège. Voilà, on a voulu une proposition circonscrit sur ce sujet et on ne souhaite pas aller au-delà. Donc je suis défavorable à cet amendement. Madame la Ministre. Je nous sommes le gouvernement défavorable aussi à cet amendement pour les mêmes raisons que madame la rapporteure. Ah non non d'abord Madame ce logo. Oui merci madame la rapporteur, j'ai bien écouté vos explications malgré tout moi je suis très favorable à l'amendement de Monsieur Maurer parce que. Il y a des cas je vais reprendre les mots de madame la ministre, elle nous a dit il faut porter une attention particulière aux situations particulières. J'ai noté plusieurs phrases que vous nous avez indiqué nous on a eu le cas d'une commune de moins de 1000 habitants, le maire était gravement malade, hospitalisé pendant de longs mois, c'est son suppléant. Donc le premier adjoint qui devait siéger sauf que lui-même y travailler la nuit, il a pas pu mettre en péril sa situation et pendant de longs mois. Cette commune n'a pas été représentés au conseil communautaire. Donc je reprends ce que vous nous avez dit, il y avait un vrai enjeu de continuité de représentation. Il faut veiller à ce que chaque commune peut garantir à chaque commune qu'elle puisse être participer effectivement et activement fonctionnement de son EPCI. Donc il faut que dans un cas, le premier adjoint lui-même demandé à ce qu'on puisse désigner quelqu'un d'autre pour remplacer le maire ou comment conseil communautaire, il existe des cas il faut il faut pouvoir avoir une toute petite souplesse dans des cas très particuliers pour que il y a une représentation effective au conseil communautaire. Très bien. Non j'ai plusieurs demandes alors chacun va prendre son tour rassurez-vous. Il y a pas le feu. À l'heure sur cet amendement, j'ai plusieurs demandes d'explications, monsieur Kerrouche.

mêmes, on n'est pas exactement dans la perspective. L'Avantage du texte de Françoise Gatel, c'est qu'il via solutionné une difficulté dont on sait qu'elle peut se manifester, essentiellement dans les communes de. Plus de de plus de 1000 habitants et elle résout un problème en trouvant j'allais dire une solution comme je l'ai dit de, de, de bon sens. Sur l'autre sur l'autre proposition qui est faite, je comprends tout à fait le. Le raisonnement mais pour autant, effectivement, l'Ordre du tableau n'est pas indifférent dans les communes de de moins de 2000 habitants. Et puis par ailleurs je veux dire c'est pas très compliqué parce que si on veut que ça ne soit pas.

tant qu'on n'aura pas changé le mode de scrutin. Dans ces dans dans ces communes me semble me semble pas adéquate et il me semble qu'on est pas dans la même perspective que dans la solution trouvée par Françoise Gatel, parce que dans un cas on est dans une logique palliative et dans l'autre cas on vient on vient corriger les règles. c'était le fait de remettre en cause pour une raison de souplesse supposé mais. Éric Kerrouche la très bien il suffit de démissionner dans ces cas-là de mettre en cause en fait le, les résultats de vente et donc du suffrage universel, donc je, je, ça je je. Nous nous opposerons. Ce qui nous concerne à cet amendement. Merci madame Hermann.

pour le coup je je reste toujours très prudente. Deuxièmement, il me semble et et j'entends les, les arguments qui pourraient être évoqué mais il ne faudrait pas aller sert à penser que à travers cette proposition de loi nous. Avons volontairement laissé de côté les communes rurales de moins de 1000 habitants, bien au contraire, elles sont soumises. De fait, à des réalités totalement différente dans les communes de moins de 1000 habitants. D'abord il c'est le la désignation se fait selon le tableau ça été rappelé et sans obligation d'alternance de sexe donc dans le cas que vous évoquiez, si on va jusqu'au bout de la logique, ça voudrait dire que si on n'est plus en capacité de pouvoir désigner un représentant au conseil communautaire. Même si la commune au sein de très petites intercommunalités aurait de sièges ça voudrait cependant dire qu'on aurait plus de la moitié du conseil municipal. En fait on est dans une situation de fait on a des démissions en masse on a des démissions en masse et une réélection de conseil municipal anticipé. Donc je je veux bien vraiment qui est un cas d'école qui le contredisent. Mais normalement, telles que la loi est aujourd'hui prévu pour les communes de moins de 1000 habitants. La difficulté évoqué ne concerne pas les communes de moins de 1000 habitants. En revanche, et ce pour ça que je vous le disais également comme d'autres l'ont dit, la question n'est pas de remettre en cause le principe de parité mais il impose d'autres règles d'autres contraintes du scrutin de liste et de l'alternance et du respect des sexes sur lequel, là effectivement on vient apporter une dérogation pour assouplir permettent la continuité politique et de la représentation communal mais parce que l'on est dans une autre réalité qui d'ailleurs répond à une autre désignation donc en l'état, moi je ne voterai pas à certains moments, ce qui avec tout pour autant tout un souci est une problématique des communes rurales de moins de 1000 habitants à traiter, mais en tout cas pas dans ce cadre-là. Madame alors. Madame Gatel. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président. Madame la rapporteure moi j'entends parfaitement. La question qui est évoqué ou présenté par notre collègue. Nadia sur le coup je tiens toutefois dire que on ne se retrouve pas dans le même contexte, puisque je rappelle que, il a été prévu pour les communes de moins de 1000 habitants qui souvent n'ont qu'un représentant qu'on aille prendre dans l'ordre du tableau fera mesure des démissions et qu'on oblige pas à la parité. La question elle est là mais sincèrement je pense que ça n'est pas la bonne arme si je puis dire, ou le bon outil pour régler le problème est que la proposition de loi qui a été faite elle est très étroite. Je l'ai dit très humble et elle ne vise que les communes de plus de 1000 qui elles peuvent se retrouver sans solution pendant 5 ans ou 5 ans et demi. Et que si on retient cet amendement. Ça veut dire qu'on vient toucher Cécile Cukierman lundi au code électoral. Et moi j'ai le code électoral, c'est exactement comme la constitution, on y va prudemment n'ayant mesuré l'impact. Moi j'entends la question de Nadia Sollogoub. Il faudra qu'on traite ça sachant que je pense qu'on a déjà des solutions mais que je pense que venir. Mettre cet amendement c'est venir. Peut-être même empêché. Le règlement des gros problèmes sans solution, qu'il y a dans les communes de plus de 1000 donc et on ne réglera rien et que par contre moi je pense que ça, ça nous amène à réfléchir. Un sujet dont on parle beaucoup, c'est la diminution du scrutin de liste en deçà de 1000 habitants. Et que je pense que ça vaut la peine de débat de ça alors je vois que certains hoche de la tête horizontalement et pas verticalement. Ça doute mais je pense qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus mais sincèrement chers Nadia et mes collègues, vous avez un problème, c'est pas le bon outil. Et ça va faire capoter lorsqu'on essaie de régler pardon. Merci. Exceptionnellement, Madame Sollogoub. Je ne vous redonne la parole, que si vous retirez sinon vous ne pouvez pas l'avoir. Donc vous ne la prenait pas très bien madame la. Rapporteure. Juste pour compléter ce que vient de dire Françoise Gatel. En effet il y a un sujet en dessous de 1000 moins 1000 habitants et il y a une vraie réflexion à avoir sur le scrutin. Des moins de 1000. Voilà donc on peut avoir des avis divergents, mais enfin en tout cas il y a un vrai sujet

Qui est contre. Il est rejeté. Je vais mettre aux voix l'article unique mais naturellement le vote sur l'article valant vote sur l'ensemble de la proposition de loi, il y a l'explication de vote de Monsieur le questeur. Merci monsieur le le président, madame la Ministre, mes chers collègues. Je, j'aurais voulu. Pouvoir défendre et soutenir les excellences amendement présenté par mon collègue et ami Éric Kerrouche. Malheureusement ce n'est pas possible puisque l'article 45. Tel que nous le vivons au Sénat ne le permet pas. Donc je me permets de dire Madame la Ministre qui serait vraiment très heureux que nous puissions avancer sur ce sujet. De la parité au sein des exécutifs intercommunautaires. En effet, comme mon collègue là expliqué cela a été voté par le Sénat. Et donc il est regrettable mais c'est l'affaire de l'Assemblée nationale. Que cela n'ait pas prospérer et que cela n'ait pas pu être inscrit dans la loi. Or chacun voit que la parité est maintenant considérée comme juste nécessaire pleinement légitime. Et qu'il n'y a pas d'obstacle. À mettre en oeuvre cette parité dans les exécutifs. Il y a assez de d'élus des 2 sexes dans la très grande majorité presque l'unanimité des métropoles des communautés d'agglomération et même communauté de commune pour que cela devienne effectif et même si on ne le pouvaient pas, il y a le second amendement qui a été également présentée qui consisterait à ce que de ce point de vue de la parité. la composition de l'exécutif soit homothétiquement à la composition de l'Assemblée donc Madame la Ministre j'espère que vous nous soutiendrez de manière à ce qu'on puisse inscrire cette avancée très attendue par un certain nombre d'associations et beaucoup d'élus dans la loi, je vous remercie. Merci monsieur le questeur jeu mais aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vais suspendre la séance elle sera reprise à 21h 30 pour le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 23 et 24 mars 2023. La séance est suspendue.